La séance est ouverte. Bonjour, chers collègues. Bonjour, madame la Ministre, le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, y a-t-il des observations. Je n'en vois pas le procès-verbal et donc adopté sous les réserves d'usage. Mes chers collègues par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande d'inscription lors du jour du mardi 9 mai des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, après l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. Acte et donner de cette demande. Le délai limite pour les inscriptions de parole sera fixée au vendredi 5 mai 15h, y a-t-il des observations non il en est donc ainsi décidé l'ordre du jour appelle le débat sur le thème l'avenir de la ressource en eau comment en améliorer la gestion. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartis pour une minute. Madame le Ministre vous pourrez donc si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé une place, sa place de préférence dans l'hémicycle. La parole et tout d'abord à l'orateur de la délégation qui a demandé ce débat. Notre collègue Jean Sol au nom donc de la délégation sénatoriale à la prospective chargeant vous avez 8 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Qui dites oh santé assainissement hygiène et prévention des maladies d'et du du Développement durable, lutte contre la pauvreté. Soutien au système alimentaire et création d'emplois c'est prospérité. C'est pourquoi l'eau doit être au centre de l'agenda politique mondial. C'est par ces mots qu'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations-Unies. Conclut et la conférence des Nations-Unies sur l'eau le 24 mars dernier. En France aussi. L'eau est au coeur du développement de nos territoires de notre agriculture de notre système énergétique puisqu'il faut beaucoup d'eau pour refroidir les centrales thermiques. L'eau est également essentielle à l'équilibre des écosystèmes et quand elle vient se dégrader, il en manquait ou à l'inverse, à être en trop. Les conséquences sont dramatiques. Plus trivialement, l'eau est au coeur de notre vie quotidienne. Nous ne faisons même plus attention à la prouesse que constitue le fait d'avoir tout le temps à notre disposition une eau de qualité. Simplement en ouvrant le robinet et pour un coûte relativement modeste de 4 euros et 30 centimes en moyenne pour 1000 litres, assainissement compris mais cela sera-t-il toujours le cas. L'année dernière plus de 2000 communes ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable. La sécheresse s'installe comme une situation non plus exceptionnelle mais habituelles et récurrentes dans un pays tempéré comme le nôtre c'est un choc culturel. Sur l'Hexagone, nous recevrons chaque année plus de 500 milliards de mètres cubes de précipitations dont un bon tiers c'est un filtre dans le sol ou vont dans nos rivières. C'est ce qu'on appelle les pluies utiles 200 milliards de m3 en toute en toute logique, nous ne devrions pas avoir de difficultés puisque nous n'utilisons de l'ordre de 30 à 32 milliards de mètres cubes par an, 15 pour le refroidissement de l'eau centrales cinq pour l'alimentation des canaux cinq pour l'eau potable trois pour l'agriculture et un peu moins de trois pour l'industrie. Bien sûr il faut laisser une partie de ses taux dans les notes dans les rivières et plus largement dans les milieux mais nous devions pouvoir répondre à tous nos besoins. Malheureusement, le réchauffement climatique change la donne. L'étude explore 2170 nous dit que le débit de nos rivières va baisser de 10 à 40% d'une année sur l'autre. Nous pouvons connaître des variations importantes de précipitations. La sécheresse explique maman forte que nous avons connu en 2022. Qui vient après d'autres étés secs a fait prendre conscience que nous n'avons pas échapper à une remise en cause de nos modèles au 1er mars de cette année 80% des nappes phréatiques sont encore à un niveau considéré comme bas par le Bureau de recherches géologiques et minières. Aucune région n'échappe au phénomène. L'année dernière ce sont la quasi totalité des départements qui ont été touchés par des arrêtés sécheresse. Pour l'eau l'été entre juin et août devient de plus en plus critique et à l'heure où nous parlons les perspectives estivale 2023 sont particulièrement sombres. La délégation à la Prospective du Sénat avait déjà tiré le signal d'alarme en 2016 avec l'excellent rapport au urgences déclaré de nos collègues Jean-Jacques Lozach et Henri Tandonnet depuis 2022 nous avons lancé de nouveaux travaux pour actualiser on nous donner affiner notre analyse avec pas moins de 4 rapporteur au nom desquels je parle aujourd'hui Catherine Bell Rithy Cécile Cukierman Alain Richard et moi-même notre rapport articulée autour de huit question s'intitule comment éviter la panne sèche, car sans être alarmiste. Il faut être lucide. Nous pouvons gérer l'eau dans la nouvelle période qui s'ouvre mais il va falloir s'en donner les moyens, ces moyens existent. Nous avons en effet depuis 1964 une gouvernance de l'eau par grands bassins Hydro-Jo Le hydrologiques pardon reposant sur les agences de l'eau, une planification pluriannuelle à travers les stages des moyens financiers mobilisés. Grâce aux redevances plus de 2 milliards d'euros par an. Nous avons des collectivités territoriales impliquées dans le petit con me que le grand cycle de l'eau qui se sont parfois regroupées dans des établissements publics de bassin pour gérer en commun les ressources et les milieux avec comme philosophie la démocratie de l'eau. Bref, nous sommes armés pour faire face aux défis de l'avenir de l'eau mais nous sommes aussi en difficulté pour définir ce que nous voulons pour mieux gérer notre. Sur le plan qualitatif. Nous continuons aux à poursuivre un objectif d'excellence fixé d'ailleurs par les textes européens comme la directive la directive-cadre sur l'eau. Malheureusement le bon état des masses d'eaux souterraines et de surface. Ne sera pas atteint à l'échéance de la directive qui a pourtant déjà été repoussée à 2027. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer nos efforts. Lutter contre les pollutions organiques les nitrates. Les résidus de pesticides. Les résidus médicamenteux les pollution plastique ou les péages. Ça c'est, c'est un enjeu de santé publique non négociable sur le plan quantitatif, l'équation se Corse. La priorité doit être la sobriété. C'est ce qu'a dit en tout cas le président de la République en présentant le plan eau du gouvernement en 53, mesure le 30 mars dernier. Nous, les 10 ans aussi dans notre rapport. Mais cela ne doit pas se faire en partant d'un dogme d'interdiction de toute nouvelle retenues d'eau. Gérer l'eau est consubstantielle à la civilisation. Refuser par principe de le faire c'est se condamner à des difficultés futures pour tous, à commencer par les agriculteurs. La première recommandation de notre rapport et de permettre de nouvelles retenues dès lors que le service environnemental et économique rendu et de positif. La seconde est de mettre en oeuvre les solutions de gestion de l'eau. Fondée sur la nature. Nous proposons aussi d'accélérer la transformation des pratiques agricoles pour faire face aux tensions hydrique. Disons-le tout Net, faire de l'agriculture sans eau et impossible mais améliorer les systèmes d'irrigation, les pratiques culturales. Mieux gérer la ressource. C'est possible à condition d'accompagner les agriculteurs. La recherche et l'innovation peuvent aussi être mobilisées pour avancer par exemple en encourageant la réutilisation des eaux usées traitées particulièrement utile dans les zones côtières en bout de bassin. Cette proposition de notre rapport figurent dans le plan eau du gouvernement. La question des moyens financiers Madame la Ministre ne peut être éludée. Notre rapport juge indispensable de euros aussi les moyens des agences de l'eau notamment, point sur lequel le plan eau apporte aussi une réponse. Notre rapport préconise également de davantage. La décision publique sur l'eau et de repolitiser les instances de l'eau qui ne doit pas être une affaire unique de technicien. Enfin, nous préconisons de faire davantage de pédagogie auprès du grand public pour faire connaître les enjeux de l'eau et faire prendre conscience des efforts que nous allons tous devoir faire. Je terminerai en disant que les principes de la politique de l'eau ne doivent pas nous faire perdre notre bon sens en vous parlant de nos vieux canaux d'irrigation des Pyrénées-Orientales au nom des débits réservés aux n'empêche l'audit circuler. Or il contribuer à recharger la nappe. À ralentir l'écoulement d'une autre fleuve la tête vers la Méditerranée. Il faut vivre hein maraîchage local vertueux vous en conviendrez. Tuer nos agriculteurs ne résoudra pas no souci d'eau. Alors je formule un voeu. Que l'on trouve des solutions raisonnables comme le faisaient nos anciens. Car si l'eau est plus rare. Elle n'a pas disparu et la France ne sera jamais le savoir. Notre Intelligence collective doit nous permettre d'éviter la panne sèche. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le président de la la délégation à la prospective mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur, seul. D'abord je je vous remercie pour vos propos introductif et je profite de ces 2 minutes de temps de parole pour pour vous répondre. 3 mois nous séparent du précédent débat sur l'eau au Sénat. Le 10 janvier dernier, nous étions en effet réunis sur cet dans cet hémicycle et nous partageons les enjeux justement dans les territoires d'une gestion résiliente et concertée de la ressource en eau, Précis, j'avais déjà pris connaissance avec beaucoup d'attention de votre rapport, et je tiens à saluer à nouveau la qualité de votre travail. J'ai plaisir à revenir aujourd'hui sur ce sujet. Quelques jours après la présentation du plan eau par le président de la République, un plan très complet, avec 53 à mesure des moyens inédits qui je crois apporte des réponses concrètes à vos préoccupations et auprès. Préoccupations des des collectivités. La politique de l'eau, elle est structurée. Elle est bien outillée mais le président l'a confirmé. Nous devons aller plus loin pour être à la hauteur des enjeux environnementaux. Nous avons donc travaillé pour définir un plan d'action collectif à partir d'une concertation notamment des comités de bassin et du comité national de l'eau et des représentants aussi des collectivités. Nous avons désormais la méthode le chemin pour parvenir aux aux engagements pris aux assises de l'eau et dans le cadre aussi du Varenne agricoles de l'eau et l'ambition est bien de garantir à long terme, un accès à l'eau pour tous, une eau de qualité et des écosystèmes préserver. Le thème de votre débat s'inscrit dans l'avenir. Je m'en félicite car je souhaite que nous soyons très concrets. Quant aux solutions à apporter pour nous adapter aux bouleversements climatiques. Il en va également de notre avenir. Les questions que vous célébrez lors de ce débat appelleront à ce que je puisse entrer plus dans le détail du plan eau donc je vous remercie et donc je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci la parole est à présent à Monsieur Alain Joyandet du groupe les républicains en attendant votre monter je salue madame Lemaire de Sainte Terre et son conseil municipal des jeunes. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le président, mes chers collègues. La longue histoire de la gouvernance de la gestion de l'eau en milieu rural. C'est sur ce sujet que je voudrais exclusivement concentré mon mon propos Madame la Ministre une majorité de communes rurales veulent conserver la gestion de l'eau et c'est sans doute l'intérêt général. Mais le parcours du combattant épuisant. Ici nous sommes leur porte-voix. Pas seulement parce que nous portons aussi des textes. Étape après étape. J'espère que nous finirons par obtenir satisfaction mais à quel prix et quel temps perdu. Juste un rappel de ce parcours qui commence en 2015 avec. La fameuse loi notre ou. C'est, c'est selon, qui oblige le transfert de l'eau et de l'assainissement des communes vers les communautés de de communes des propositions de loi, notamment en 2017, j'en avais déposé une ici avec un certain nombre de collègues. La proposition de loi de loi Retailleau en 2017 qui a été adoptée, qui remettait la compétence de l'eau dans les compétences optionnelles, 2018 avec une nouvelle loi. Qui permet de passer de 2020 à 2026 ce qui veut bien dire quand même qu'il y a un problème puisque le gouvernement accepte ce report d'autres étapes avec une autre proposition de loi en 2020 d'un certain nombre de collègues ici dont je faisais.

Nouvelle preuve qu'il y a véritablement problème, notre excellent collègue Mathieu Darnaud dépose à nouveau une proposition de loi le 22 juin 22. Et puis en 1900 en 2023 une proposition de loi qui ici est à nouveau voter qui permet également de passer dans la catégorie des compétences Madame la Ministre 329 voix, 329 suffrages exprimés. 259 voix pour, 70 voix compte. Vous voyez qu'ici sur tous les bancs. On dit bien qu'il y a un problème et qu'il faut trouver une solution enfin enfin 9ème étape. Il y a quelques jours, j'allais dire quelques semaines. Le ministre-votre ministre. Qui est en charge. Et qui nous déclare ceci Madame la Ministre c'est important parce que c'est ma question si vous avez la possibilité de répondre le ministre ici en que âgé, il y a une quinzaine de jours à la question. Qui est la même question, il répond, je cite, j'espère fidèlement ce n'est pas forcément l'intercommunalité. Je rappelle que dans le texte actuel, c'est l'intercommunalité. Donc il nous dit je répète ce n'est pas forcément l'intercommunalité mais il ajoute aussitôt, ce n'est pas non plus la commune seul. Alors vraiment ma question madame Annie c'est qu'est-ce que ça veut dire des milliers de communes attendent de savoir ce qu'ils doivent faire avant 2026. Certaines qui ont anticipé. Pensant que ça allait arriver de toute façon que, constate-t-elle. Elle constate que pour un grand nombre d'intercommunalités. Je je je précise bien en milieu rural, c'est absolument ingouvernables. On embauche des dizaines de fonctionnaires territoriaux supplémentaire avec la conséquence de l'augmentation des prix dans mon département, il y a même une interco qui n'a pas pu envoyer les factures d'eau. Aux concitoyens depuis un an et demi. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je fais juste partie de ceux qui disent qu'il faut remettre ses de compétences dans les compétences optionnelles et surtout laissez les élus décider. Nos collègues élus locaux ont du bon sens du sérieux bien sûr qui sont attachés à la quantité de l'eau, ils sont attachés à la qualité de l'eau. Mais quand des mesures venues d'en haut s'impose à tout le monde est que la conséquence dans une commune rurale, c'est que le prix de l'eau est multiplié par par trois par 300 clos n'changé en quoi que ce soit, je pense que c'est intolérable que l'eau que le tarif de l'eau augmente quand on a fait des travaux sur les réseaux. Quand on a fait des travaux dans la filtration dans la qualité, tout ça s'explique tout ça est normal le service public s'il coûte plus cher. Il doit correspondre à une amélioration. Donc on est vraiment. Madame la ministre, dans une situation pour laquelle un certain nombre d'entre eux d'entre nous se battent pas pour nous mais pour défendre l'intérêt de nos concitoyens. Vous savez en zone rurale. Quand on a déjà tellement, tellement de, d'inconvénients au quotidien et ce qu'on doit dire aux gens, c'est la mode, il faut augmenter le prix de l'eau parce que l'eau c'est notre avenir. On m'a même répondu parfois dans mon département, une représentante du gouvernement, m'a dit c'est la c'est la qualité de l'eau et la santé de nos enfants qui est en jeu, je peux vous dire que chez nous dans une petite commune où tout va bien, où l'eau est bonne ou il en a assez, ou le Fontagné souvent bénévoles depuis 25 ans en fait un travail extraordinaire. Pourquoi casser ce qu'il marche bien parce qu'il faudrait que tout soit exactement pareil quelles que soient les territoires et l'importance de nos collectivités. Voilà donc moi je vous supplie. De nous expliquer, de faire l'exégèse des propos du ministre et le plus vite possible de nous donner un texte pour que des milliers de communes sache ce qu'elle doit faire ou ne pas faire avant 2026 dollars. Je vous remercie pour vos réponses. Merci madame la présidente,

Déjà, je tiens à rappeler que 88% des des communes, c'est déjà l'intercommunalité qui porte la compétence eau et assainissement et la mutualisation sous la forme de l'intercommunalité et donc largement enclenché pour ses 88% des des communes qui porte, seuls la compétence sont concentrées dans certains départements et c'est d'ailleurs par exemple le cas des Hautes-Alpes où était le président de la république lorsqu'il a fait les, les annonces du plan eau. Ça a été d'ailleurs l'occasion pour le président de la République de rappeler l'importance de la mutualisation. Dans la capacité justement d'ingénierie la capacité d'investissement également la capacité d'innovation. Je crois que c'est essentiel pour garantir un service public, efficace et surtout aussi un niveau de service qui mérite que mérite justement nos nos usagers, vous avez donné des exemples de communes où ça fonctionne bien. Bien sûr qu'il y en a mais il y a aussi 2000 communes qui ont connu des tensions sur l'approvisionnement en eau potable et la large majorité était des communes isolées et des travaux de sécurisation sont nécessaires pour améliorer justement leur résilience et les 170 communes qui ont 50% de rendement seulement sont des communes isolées. Donc il y a bien un lien entre les communes isolées et le fait qu'il y a une baisse de rendement. Donc des moyens financiers sont apportées justement pour soutenir les collectivités en difficulté et l'État a engagé 100 millions d'euros complémentaire des agences de l'eau en 2022 et 100 nouveaux millions d'euros en 2023 et ça suffira pas et il faut que les collectivités face et de la capacité d'ingénierie nécessaire. C'est pourquoi le gouvernement ne souhaite pas revenir sur le transfert des compétences eau et assainissement au niveau communal, le ministre et je tient les mêmes propos que le ministre-Béchu ici même, j'étais présent donc je me rappelle très très bien des aussi des propos qu'il a qu'il a tenue. Il pouvait y avoir une remise en cause de l'intercommunalité, mais que par contre la mutualisation n'était en aucun cas remis en cause et donc le niveau communal ne semblent pas correspondre aux besoins surtout des communes qui aujourd'hui sont en manque d'eau, particulièrement sur les périodes estivales. Donc il a été. Notamment. Annoncé qu'une mission parlementaire allait être lancée prochainement et justement pour examiner les solutions ou l'intercommunalité ne répond pas justement aux besoins du territoire et uniquement dans ce cadre. Par contre, il est évidemment possible de revoir l'intercommunalité mais pas la mutualisation c'est l'esprit même de ce qui a été défendu par le ministre une majorité. Madame la Ministre, nous allons poursuivre. vous avez émis. Oui je vous en prie. Merci madame la présidente. Bon ça répond pas à ma question, puisque c'est un arbitre pas mais je je je je n'en suis pas surpris savez quand même que dans le texte de loi aujourd'hui une interco peut prendre la compétence puis décidé dans la mine dans la demi-heure qui suit de leurs délégué aux communes. C'est possible de le faire. Donc à ce moment-là, on va faire comme ça, on va dire à nos Interco vous prenez la compétence vous délibéré. Vous prenez la compétence et de la demi-heure qui suit, vous leur délégué aux communes. Madame la Ministre, c'est ça. Le texte, pourquoi nous, pourquoi ne pas clarifier les choses et moi ce que je dis c'est je je ne bande d'obligation ni dans un sens si dans l'autre, je demande juste de redonner aux élus locaux le pouvoir de décider. Bien sûr que dans certaines communes où il y a plus d'eau, il faut faire des choses, ils le font, ils nous ont pas attendu ça fait dans mon département, j'ai des syndicats avec 17 18 communes depuis 30 ans donc nos élus locaux. Faisons-leur confiance. Madame la Ministre, pourquoi vouloir faire encore un truc alambiquée qu'est-ce que ça veut dire pas l'Interco mais pas la commune. Alors on va refaire une mission parlementaire. Alors que ce serait tellement facile de dire pour l'eau dans les communes de moins de je sais pas de 20.000 habitants, on remet ça dans les compétences optionnelles voilà enfin si, un peu de simplification et de bon sens. Venez faire un petit séjour en Haute-Saône. Je vous invite vous seraient reçus cordialement. La parole est à présent à Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. Yassine d'Ardern ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande, lors de son dernier discours devant son Parlement. A déclaré que le changement climatique défini notre génération de politiciens. Je crois cette infirmation vrai. Sur tous les bancs de cet hémicycle. Ou de celui de la rue de l'Université malgré nos sensibilités différentes. Nous essayons de lutter contre le dérèglement climatique et ses effets. nos visions pour y parvenir sont clairement différentes. Mais les conséquences sont déjà là nous les subissons et essayons de nous adapter. C'est en cela que quoi que nous pensions. Même si vous avez beau ne pas vous occuper du changement climatique. On peut dire que le changement climatique s'occupe de vous. L'avenir de la ressource en eau, en est l'exemple parfait. Je ne pense pas me tromper. Nous souhaitons tous une gestion. Ça a été dit améliorée de cette ressource vitale. L'eau régule l'ensemble du cycle de vie et notre environnement, nos mers et océans abritent une biodiversité qui est essentiel à la vie et absorbe une part importante de notre pause pollution en CO2. L'accès à l'eau à travers le monde et l'un des principaux enjeux pour nombre de population et bien souvent, on le sait malheureusement la source de conflit meurtrier. Face à cette rareté les solutions implique de travailler à l'échelle mondiale à la chaîne d'approvisionnement global en haut, à commencer par les glaciers. La qualité de l'eau et tout aussi importante évidemment les récentes détection dans notre eau potable d'un pesticide interdit depuis des années relance ce sujet. Madame la Ministre quelles sont les pistes envisagées en termes de gestion pour juguler ce type de risque. Comment s'attaquer aux causes de ces pollutions. Madame la Ministre je sais que vous êtes sensible à ce sujet les homologations de nouveaux produits comme les bio-contrôle en substitution aux pesticides chimiques, sachant que. Et ses homologues européens sont sur saturés. Le stress hydrique que nous subissons depuis l'été dernier et par période. Et toujours plus fréquentes participe de nos questionnements sur l'état de cette ressource. Si nous faisons le point sur la qualité de l'eau, son manque sur certains de nos territoires. Ainsi que sur les hausses de sa consommation. Nous devons inévitablement par les gestion. C'est là que la vision libérale de l'écologie que défend le groupe les indépendants prend tout son sens. Il est impossible de revenir en arrière. Avec les méthodes d'autres siècles pour gérer une ressource qui est confrontée à de nouvelles problématiques. Nous sommes simplement trop loin dans l'avancée du changement climatique et les solutions qui compte viendront de la recherche et de l'innovation. Nous ne pouvons nous adapter qu'en regardant devant avec un devoir d'anticiper et de prévenir. Il faut faire les investissements nécessaires dans nos réseaux, cela a été dit dans un pilotage optimisé et aussi une gestion intelligente de nos trop. Le système a besoin de clarifications quant aux responsabilités qui incombent à chacun, notamment au sein des collectivités. Celui-là a été rappelé. Je salue le plan sobriété que vous avez lancé madame la ministre, avec certains de vos collègues. Nombre de ces propositions rejoignent ce en quoi nous croyons et sur quoi nos actions de notre travail. J'évoquais à l'instant, la recherche et l'innovation. Il est pertinent d'actualiser nos projets hydrologiques et d'évaluer les perspectives. Nous serons plus réactif dans une gestion que je conçois comme flexible pour une adaptation rapide. je suis à cet égard particulièrement sensible aux outils qui nous permettront de prendre en compte l'aménagement de nos territoires dans leur spécificité. La ressource en eau effectivement n'est pas la même que l'on soit en Aveyron, dans l'Aube ou en Corse. Nous devons partager nos bonnes pratiques et trouver les solutions et les meilleurs instruments en fonction de nos besoins propres qui sont Haddock en fonction des territoires dans lequel nous sommes, vous le savez, je crois aussi beaucoup en la sensibilisation et la formation Madame la Ministre. Nous avons besoin de gens formés dans la gestion de l'eau et de sa préservation, qu'envisagez-vous concernant la formation notamment d'ingénieurs en ce domaine. Sur le volet financement votre plan met en lumière une nouvelle génération d'Aqua prêt à un taux bonifié pourrez-vous nous expliquer les évolutions que vous prévoyez. Quid du crédit d'impôt sur les récupérer les récupérateurs d'eau dans les zones en tension. Nous avons besoin aussi de vos éclairages sur ce sujet. Enfin et parce que je ne pouvait conclure sans évoquer ce sujet la tarification progressive de l'eau sur laquelle le 16 sera saisi. Je forme le voeu que le plus d'acteurs possible mais notamment et surtout des praticiens soient associés à cette réflexion. La gestion de notre ressource en eau sera de plus en plus complexifié par le changement climatique. Une bonne gestion impliquera un pilotage fin qui devra allier flexibilité et adaptabilité pour répondre à tous les enjeux de nos territoires. La recherche et l'innovation devront nous y aider. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame le Ministre vous avez 2 minutes. Merci de le repréciser madame la présidente. Parce que je, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir répondre à tous et j'ai profiter de toutes les questions. Et c'est justement le manque de temps, donc je me plaignais monsieur le sénateur, parce que j'ai bien envie de de vous répondre à toutes vos à toutes vos questions. Donc vous vous répondre madame la sénatrice Paoli. Agen. Déjà vous dire que vous avez raison sur le sujet de l'eau c'est un sujet mondial et je suis très heureuse d'avoir participé à la conférence des Nations-Unies qui s'est tenue à New York il y a maintenant une quinzaine de jours, où on a pu aborder justement la question de l'eau se laver. 46 ans qu'il n'y avait pas eu de conférences et ça permettait justement de reparler de ces sujets, avec beaucoup de pays à travers le monde et on voit que c'est un sujet en effet éminemment important pour, pour les prochaines prochaines Évidemment fournir une eau de qualité, c'est une nécessité pour la santé évidemment de de toutes les personnes au niveau mondial mais aussi et bien sûr pour la santé des Français et on observe en effet une tendance à la dégradation de la qualité chimique des eaux souterraines. Je rappelle tout de même que le dépassement du seuil de potabilité est une alerte, mais qui n'implique pas un danger éminent pour la santé des Français. C'est un signal sur la nécessité d'agir pour inverser la tendance. L'eau potable vient au 2 tiers des nappes. Il convient donc de mieux prévenir les pollutions diffuses, à l'échelle des aires d'alimentation de captage. Pour cela, nous allons accompagner des évolutions de pratiques agricoles, pour utiliser moins de pesticides, moins d'engrais chimiques sur ces zones particulièrement sensibles et vous avez raison, la question du biocontrôle m'apporter et ce sont des solutions qui peuvent justement. Permettre de moins utiliser des produits chimiques, il y a eu notamment des enveloppes ont été déployés sur le précédent mandat pour justement boosté la recherche parce que il faut bien chercher en fait pour annuler retirer. Une molécule, il faut bien qu'il faut qu'on trouve justement une solution alternative biocontrôle et c'est justement l'utilité ce fonds c'est justement faire les recherches nécessaires. On souhaite également accompagner les nouvelles générations pour favoriser l'installation en bio est également en agro-écologie. Nous allons aussi apporter 100 millions d'euros supplémentaires pour soutenir financièrement les agriculteurs qui utilisent justement moins d'intrants. Au niveau des négociations européennes parce qu'on sait qu'il y a aussi évidemment le niveau européen qui compte. On est en pleine négociation sur le règlement pour un usage durable des pesticides le règlement sur et nous allons porter une ambition de meilleure protection des captages, nous allons aussi agir plus vite en cas de dépassement d'un seuil sanitaire si la molécule en question est toujours utilisé, il y aura automatiquement des mesures mises en place par le préfet en complément du plan de de gestion de la collectivité. vous m'avez interrogé sur le crédit d'impôt pour les récupère récupérateur d'eau de pluie. Nous sommes en train d'instruire les conditions de de sa réactivation. Et je ne manquerai pas de vous tenir évidemment informé de de l'avancée de de nos travaux sur le sujet et vous avez également abordé le sujet de la formation. Nous avons en France la chance d'avoir des établissements d'enseignement supérieur reconnu est réputé pour la qualité de leur formation sur le sujet de l'eau. Madame Merkel. Disons que je crois que j'ai profiter de la prochaine. Chen réponse parce que là j'ai laissé plus d'une minute de plus. La parole est à présent à monsieur Daniel Breuiller du groupe écologiste pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre. Merci à Jean Sol et à la délégation prospectives de ce débat. J'ai écouté comme tous ici les déclarations du président de la République à propos de l'eau j'étais d'ailleurs satisfait d'entendre que des propositions que nous avions défendu un projet de loi de finances et qui avait été rejetée étaient reprises Madame la Ministre dans votre plan, je pense au plafond mordant dans des agences à la tarification progressive de l'eau à l'augmentation des financements à l'agriculture biologique et pour la sortie des engrais azotés de synthèse ou encore le développement de paiement de services environnementaux. Même si, pour ces 3 mesures, nous proposions un accompagnement sur tout le territoire et pas seulement sur les aires de captage. Madame la Ministre pour accélérer votre action contre les dérèglements climatiques pour une gestion durable de l'eau, n'hésitez pas à consulter nos amendements. Et nos propositions actuelles en voici quelques-unes. La première concerne la qualité de l'eau. Enjeu essentiel évoqué de façon trop superficiel dans le plan présidentiel. La moitié des masses d'eau sont pollués par des plastiques des nitrates des herbicides et des pesticides sur ce sujet rien ou presque pire au lendemain de l'annonce du plan eau. Le ministre de l'agriculture et des pesticides demande à l'Inde cesse de revenir sur l'interdiction de l'herbicide S- métolachlore remarquable sens des priorités puisque 2 jours après de nouvelles études été rendu public sur la non-conformité d'un tiers de l'eau distribuée en France en raison de la présence du métabolites chlorothalonil R 400. R 400. 811 pour la qualité de l'eau. Nous revendiquons un plan d'appui à la transition de l'agriculture vers l'agroécologie un plan massif et vers l'agriculture biologique car elles reposent sur des pratiques sobre en haut et permettent de retenir l'eau dans les sols par les les couverts végétaux les prairies les rotations. La nature a ses propres solutions et des agriculteurs ont toujours été au rendez-vous des demandes de la nation. Encore faut-il les engager sur ce chemin plutôt que de défendre un modèle qui craque face aux pénuries mais qu'il reste rentable pour l'agro-industrie. La seconde suggestion concerne la gestion quantitative. Les assises de l'eau avait fixé en 2019 un objectif de réduction de 10% des consommations à échéance 2024 vous le reprenez met à échéance 2030, madame la Ministre, la situation se dégrade vite, on ne peut retarder les échéances. Ni en extraire l'agriculture qui consomment 56% de la ressource, ni l'industrie dont les développements. Peuvent être très consommateurs. Je n'irai aussi des tensions comme l'illustrent le projet de développement de STMicroelectronics à Crolles, le groupe écologiste solidarité et territoires souhaite également un moratoire sur les projets à fort impact sur les cycles de l'eau et non compatible avec les bouleversements climatiques mégabassines réserve d'eau pour canons à neige ou le Lyon-Turin. Il est aussi primordial de concert de considérer les évolutions de la ressource en eau dans nos choix énergétiques et notamment les risques liés à la baisse du débit d'étiage des fleuves de 20 à 40% d'ici 2050 et de combien d'ici 2100, date de fin de vie de vos potentiels futurs EPR sans oublier leurs impacts sur les milieux aquatiques, la biodiversité et la qualité de l'eau l'été, il faudra choisir entre la fourniture d'eau potable, la préservation des milieux la fourniture pour l'électricité et pour l'agriculture qui arbitrera et comment elle le fera-t-on sans conflit. Pour nous, ce doit être la science partagée et la démocratie qui doivent arbitrer. Nous demandons la mise en place d'études académiques en amont de tout projet impactant le cycle de l'eau et le partage des ressources. Madame la ministre, il y aura de plus en plus de conflits d'usage au fond ce qui s'est passé à Sainte-, Soline n'est qu'une illustration de tension beaucoup plus nombreuses et parfois moins visible et moins médiatisés. L'agriculture a besoin d'eau mais elle en a besoin dans les sols plutôt que dans des méga-bassines, elle en a besoin dans des systèmes d'irrigation vertueux pour que les conflits d'usage ne deviennent pas des conflits violents, il faut trouver des réponses démocratiques plutôt que des réponses sécuritaires au plan territorial. Les commissions locales de l'eau, les projets de territoire pour la gestion de l'eau doivent être généralisé mais surtout réellement ouvert à tous sans omission des associations environnementales ou de la Confédération paysanne comme c'est le cas ici ou là, au plan national. Le groupe écologiste solidarité et territoires vous propose d'organiser une Convention citoyenne de l'eau sur les chemins de sobriété et les priorisation en temps de sécheresse. La Convention citoyenne sur la fin de vie et la preuve heureuse que les Françaises et les Français ont envie d'une démocratie ouverte et sont capables de trouver un consensus éthique et profond sur des sujets complexes. Si cette démarche peut éviter des affrontements dramatiques osons ce chemin en France et dans le monde, nous vivons à présent cette crise de plein fouet. Faites donc confiance aux citoyens. Écoutons les ONG des scientifiques et même les parlementaires écologistes ou la prochaine mission au. Dans le rapporteur et notre collègue Hervé Gillet. Ce sera utile pour être à la hauteur des enjeux. René Dumont prédisaient la raréfaction de l'eau dans l'indifférence généralisée voir sous les sarcasmes des partis de gouvernement en 1974, il avait pourtant raison et nous sommes dans la crise. Merci madame le Ministre, si vous avez. Un peu de temps pour répondre toujours un petit peu de temps j'en prends moi madame la présidente. Monsieur le. Le sénateur Breuiller vous avez donné beaucoup d'éléments simplement peut être revenir déjà vous remercier pour les 10 propositions et ça montre qu'on a aussi fait un travail de concertation de qualité parce que vous avez souligné qu'on a repris quelques-unes et d'ailleurs quelques-unes, enfin même de nombreuses. Vous dire que. Ce que nous souhaitons, évidemment, c'est parvenir à ces 10% de prélèvements en moins d'eau pour ça. Il est vrai que si daté à 2030 mais maintenant on donne vraiment la manière dont on va y parvenir jusque-là on avait donné l'objectif sans se donner les moyens, aujourd'hui on arrive avec un plan qui est complet et qui permet justement à chacun de se donner les moyens. Quand je dis chacun sait que toutes les parties prenantes prennent leurs responsabilités. C'est évidemment les collectivités, les particuliers, mais également les industriels et aussi les agriculteurs, chacun va justement contribué à la baisse de 10% de prélèvements. C'est vrai qu'il est pas facile de faire cette, cette modification dans le domaine agricole c'est certain quand on regarde, il faut bien sûr vous l'avez souligné le sujet de l'irrigation. Mais le sujet d'irrigation concerne que 7% des eaux utilisées par le secteur agricole, il faut qu'on revoie aussi les cultures qui sont aujourd'hui. Mises dans certains territoires qui doivent être. Peut-être oublié de certains territoires pour être planté plutôt ailleurs parce que elles sont aujourd'hui trop gourmandes en eau. Il faut qu'on arrive justement à faire les investissements nécessaires pour la réutilisation des eaux usées traitées, chose qu'on n'a pas assez fait dans notre pays. Je rappelle qu'on est à moins d'un pour 100 d'. Dans notre pays alors que on a nos voisins par exemple espagnol qui, qui avoisine les 13%,

ne nous laisse pas le temps d'aller à un rythme de sénateur, madame la Ministre et il convient donc plutôt d'aller à un rythme qui prennent en jeu cette accélération, des débats démocratiques dès aujourd'hui parce que j'ai peur que les conflits d'usage se développe, je prends note de vos engagements et je vous redis que nous sommes disposés à participer à ce travail parce qu'il s'agit du futur de notre pays comme de la planète. Merci la parole est à présent madame Nadège avez du groupe RDPI pour six minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le président de la délégation Madame la Ministre, mes chers collègues. Au cours de l'été 2022. 93 départements ont été soumis à des restrictions de consommation d'eau du fait de la sécheresse, plus de 1000 communes ont dû être ravitaillés en eau par bouteille. 32 départements sont actuellement en état de vigilance ou d'alerte renforcée et la faiblesse et la faible pluviométrie observée ces derniers mois sur l'ensemble du territoire national interroges déjà notre gestion de cette ressource fondamentale au cours des prochains mois. Depuis 20 ans la France métropolitaine a perdu 14% de ses ressources en eau renouvelable, renouvelable par rapport à la période 92.001 notre accès à l'eau et celui et ceux-là est rappelé dans le rapport fait au nom de la délégation de la prospective et rendue de plus en plus difficile avec les effets du changement climatique, déjà visible. Oui, le cycle de l'eau en France se modifie et va encore évoluer avec plus y réduire hilarité dans les précipitations. Les débits des cours d'eau vont être ralentis le stress hydrique va s'accroître, là où encore récemment, cette problématique n'était pas première. La répétition des chaleurs et leurs conséquences et à l'inverse la survenue d'épisodes d'extrême de pluies violentes va impliquer une meilleure gestion quantitative de l'eau sur toute l'année. Anticiper les événements et s'adapter aux aléas pluviométriques à leur soudaineté mais toujours aussi dans le respect des impératifs sanitaires ce défi, je dirais du volume et de la quantité. Il nous faut nécessairement le relevé en favorisant et en appelant à la mobilisation de tous industriels monde agricole et particulier en matière de sobriété dans les usages de compréhension partagée des enjeux et des progrès techniques à sortir. Face à cet état de fait qui n'est pas cons feu conjoncturelle des mesures ont déjà été prises. Un nouveau plan de sobriété visant à réaliser 10% d'économie d'eau en 2030 est désormais l'objectif que nous nous fixons dans le cadre du programme d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Les moyens mis en oeuvre se feront par secteur par territoire. Chaque sous-bassin hydrographique en fonction de ses spécificités, sera doté d'une trajectoire particulière. Parmi les annonces effectuées. Cela a été rappelé la mise en place d'un EcoWatt, de l'eau et de plan sectoriel de sobriété. La hausse du budget des agences de l'eau et la suppression de leur plafond de dépenses afin de lutter contres les fuites dans les réseaux, la mise en place d'une tarification progressive de l'eau et aussi le soutien à la réutilisation des eaux usées. Ma question portera sur ce point précis, car il s'agit en réalité pour nous de faire un véritable bond en passant d'approximativement 1% actuellement à 10% d'ici 2030, ce que font nos pays les pays proches tels que l'Espagne qui irait emploie 14% et l'Italie oui pour impulser ce mouvement essentiel plusieurs leviers vont être actionnés lancement 2000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser l'eau lancement par l'État en partenariat avec la. D'un appel à manifestation d'intérêt spécifique à destination des communes littorales sur la faisabilité du projet. Mise en place d'un observatoire national accélération des procédures administratives. Car si aujourd'hui la réutilisation des eaux usées traitées et rendu possible dans quelques part cas précis comme pour l'arrosage des espaces verts, il est nécessaire d'accélérer. C'est le sens de la 6ème recommandations transpartisane établi par les 4 rapporteurs encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de l'eau que ce soit dans la recharge artificielle des nappes dans le développement de la télé-, surveillance des réseaux dont le recours aux données numériques et à l'imagerie satellitaire pour mieux connaître en temps réel l'état de la ressource où justement dans l'arrêt utilisation des eaux usées traitées pourquoi parce que les autres traitées ne constitue pas une ressource nouvelle mais une alternative au prélèvement de l'eau dans la nature. Cela représente un intérêt certain, en période estivale dans les zones littorales touristiques là où les consommations d'eau et les besoins de l'agriculture sont importants on été. cet intérêt. L'Union européenne a voulu se doter en mai 2020 d'un nouveau règlement qui sera bientôt en vigueur visant à faciliter cette réutilisation en particulier pour l'irrigation agricole. Selon la Commission européenne. Plus de 40 milliards de mètres cubes d'eaux usées sont traitées chaque année dans l'Union européenne mais moins d'un milliard et réutiliser ces avancées comme les autres mesures précédemment évoqués iront de Pair avec une plus grande pédagogie sur l'eau, notamment auprès du grand public fin août lors des rencontres des entrepreneurs de France. Élisabeth Borne avait abordé la notion de planification écologique de l'eau avec l'objectif d'identifier les actions dont nous avons besoin pour accélérer la transition écologique et atteindre les baisses de prélèvements. La gestion de l'eau se doit d'être plus résilientes plus fiable dans les 3 domaines principaux topo que son industrie la décrit culture et les usages du quotidien. Pour ce faire il paraît indispensable de parvenir à un consensus sur l'eau, ce qui représente un enjeu national et territorial. Cela passe par un effort de démocratisation, d'éducation et de communication ciblée et continue sur les usages et leur priorisation. Madame la Ministre quelles sont les nouvelles décisions réglementaires qui pute arrête être prise rapidement en la matière et je pense aussi au secteur industriel et comment entendez-vous accélérer la procédure existante ce qu'un grand nombre d'acteurs du monde tout en rassurant sur les évolutions souhaitables je vous remercie. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice avait. Et d'ailleurs monsieur le monsieur le sénateur brouillé. Je vous le disais tout à l'heure aussi c'est que on a seulement moins d'un pour 100 de de de réutilisation d'eaux usées traitées et vraiment c'est pas assez alors que nos voisins. Vous l'avez dit. 13% en Espagne, 8% en Italie. Donc on peut on peut faire mieux et on vise les 10%. Donc ça veut dire 10% mais aussi développer jusqu'à 1000, projet. De réutilisation sur le territoire d'aucune animation et un accompagnement des porteurs de projets seront évidemment notre priorité, vous l'avez. Dit madame la sénatrice. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui sera lancée. Par l'État en partenariat avec la pour financer sans étude de faisabilité parents donc tous les cas il y a il y a un grand. Un grand soutien de la part de de Yannick Moreau sur ces sujets. Et donc ils nous souhaitons particulièrement valoriser ses projets sur les communes littorales parce que nous pensons qu'il y a évidemment un avenir et que c'est plutôt venu sur des communes qui relâchent leur eau douce dans de l'eau de mer, donc autant la récupérer. Vous parliez des évolutions réglementaires nécessaires. Vous avez raison, il y a de nombreux chantiers qui sont où se sont ouverts dès cette année. Et notre objectif évidemment c'est bien de lever les freins à la la valorisation des eaux non conventionnelles pour les usages les plus pertinents en matière d'économie d'eau tout en garantissant bien sûr la sécurité sanitaire et c'est bien ça qui a empêché nombreux plus. Jusque-là. Le décret relatif à la réutilisation des eaux dans les industries agroalimentaires est actuellement en consultation publique et l'objectif est de sortir ce texte aussi rapidement que possible. Nous engageons régulièrement des discussions avec les filières agroalimentaires qui attendent ce texte avec impatience car des des projets sont prêts à sortir. Merci à vous. Merci la parole est à présent à notre collègue Monsieur Hervé Gillé du groupe socialiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, madame la ministre. Notre groupe socialiste écologique et républicain a proposé une mission d'information sur la gestion durable de l'eau, l'urgence d'agir pour nos usages nos territoires et notre environnement. J'ai le plaisir d'en être le rapporteur. Alors à cette mission vise à réaliser une évaluation des politiques publiques de la gestion de l'eau, mise en oeuvre en France au regard des enjeux environnementaux, sociaux et économiques et cette approche sociétale est importante. Cette mission s'inspire évidemment des travaux réalisés par la délégation à la prospective et son rapport et nous remercions la, la délégation. Pour ce débat. La mission s'appuie sur 3 axes, le premier, l'enjeu de la qualité de l'eau de la lutte contre les pollutions en effet notre approvisionnement en eau potable, mais aussi pour l'équilibre des milieux de la faune et de la flore aquatique est essentielle, il nous faut disposer d'une eau non polluée. près de la moitié des masses d'eau de surface sont impactés par des pesticides. Le rapport de lancer ces ces récentes révélations sur le chlorothalonil et le S-métolachlore démontre à quel point nos quelques progrès sont insuffisants et que ce sujet doit être abordé avec humilité ce constat de la contamination est d'ailleurs relativement absent du plan eau et nous le regrettons notons néanmoins que la protection de 500 points de captage prioritaires semble porter ses fruits. Madame la Ministre, Ne faudrait-il pas étendre leur nombre pour améliorer à moyen et long terme, la qualité des prélèvements. Quels sont vos objectifs en la matière, ma collègue Florence. Reprendra d'ailleurs ce sujet notre 2ème axe concerne l'enjeu de la gestion quantitative de l'eau puisqu'en 2050 effectivement il y a une diminution prévue prévue importante des cours d'eau de 10 à 40% et les épisodes extrêmes tels que les sécheresses et les inondations seront beaucoup plus fréquent. Ainsi, nous devons optimiser les ressources disponibles, le stockage naturel bien sûr mais voir aussi créer de nouvelles ressources multi-usages et vertueuse pour l'environnement. La démarche est la méthode des. Va dans le bon sens mais où le au-delà d'un consensus territorial. Nous nous heurtons souvent à des recours tardif réduisant les négociations à néant, également, que comptez-vous faire sur ce sujet pour le faire évoluer. Nous sommes tous d'accord, nous devons prioriser une politique de sobriété de cette manière explorons toutes les pistes pour atteindre l'objectif de baisse d'eau prélevée fixé à 10% d'ici 2030, 30 millions d'euros pour les retenue agricole 180 millions pour les réductions des fuites les plus prioritaires. 50 millions pour la préservation des zones humides et l'infiltration des nappes, mais également un plan pour la réutilisation des eaux traitées ou bien la récupération des eaux toiture le plan donc propose des pistes intéressantes mais comment seront réellement financer ses chantiers. Allez-vous créer de nouvelles fiscalité ou des redevances supplémentaires pour l'avenir. Quelles sont vos réponses également sur ce sujet, il faut clarifier pour éviter les effets d'annonce. L'application de la tarification différenciée est une mesure souhaitable mais sa mise en oeuvre interroge la mise en place de ce dispositif est discuté depuis de nombreuses années, cependant il faudra engager un travail partagé approfondi avec le Parlement, les syndicats des eaux et les élus pour s'assurer d'un développement optimal. À l'instar des déchets chaque nature d'activité devra profiter d'une tarification différenciée en fonction des consommations. Ce doit être le cas également pour les ménages pour une famille nombreuse, ne soient pas lésés par rapport à un couple sans enfant. Il faudra donc créer des adaptations. Comment le gouvernement re-sur à faire de la tarification différenciée. Un dispositif efficace adaptée à chaque usage. Notre mission parlementaire. Madame la ministre est disponible pour travailler sur le sujet. Notre 3ème axe a trait au rôle des collectivités territoriales la gouvernance qui doit agir et avec quels moyens. Nous devons le rappeler sans cesse le rôle des collectivités en première ligne dans la gestion de l'eau, des fuites de la baisse d'approvisionnement l'assainissement et la Gemapi pas toujours bien financer mais également l'importance de l'échelle des bassins versants effectivement est essentiel et ses bassins versants permettre d'optimiser la ressource au Sénat, nous le savons mieux que quiconque l'échelon territorial doit être préservé et renforcé dans le cas d'une gouvernance affirmer à l'échelle du bassin versant ainsi la revalorisation financière conséquent des agences de l'or et bienvenue. 475 millions par an, mais elle ne sera pas mise en oeuvre avant le 12ème programme donc pas avant 2025. Madaule le Ministre pour atteindre nos objectifs, nous pourrions étudier la mise en place de contrats d'objectifs et de performance avec l'ensemble des parties prenantes, ou encore le conditionnement des aides et des financements des objectifs partagés pour sécuriser la ressource. Il serait donc normal de partager ses objectifs de performance et de sobriété. Chers collègues, la gestion de l'eau est un sujet éminemment politique. Il est multidimensionnelle et doit être travaillé en cohésion interministérielle avec les acteurs agricoles environnementaux économiques et sociaux ça mériterait pratiquement un ministère ou au moins un secrétariat d'État. J'en appelle de mes voeux, travaillons ensemble à des solutions concertées investissons nos instances hé ros politisant les au sens noble du terme. Je vous remercie. Madame la Ministre. Si vous souhaitez terrible. Cliquez, vous avez. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Gilles et je souhaite être évidemment la plus exhaustive possible tout en étant la plus rapide. Déjà ça, votre travail en cours. Je sais que vous menez un certain nombre d'auditions et donc je voulais saluer le travail que vous réalisez. Vous avez rappelé les engagements financiers. Je vous confirme qu'il n'y aura pas de nouvelle fiscalité mais il s'agit bien. De Réau se des taux de redevance existantes. Donc en aucun cas de nouvelle fiscalité sur le sujet de la gouvernance parce que peut-être que je peux peut-être davantage répondre à ce à ce sujet parce que nous on a abordé des des nombreux C'est une compétence décentralisée, et il n'y a aucune et vous l'avez vu aucune volonté du gouvernement de revenir se là dessus c'est ancien hein depuis les années 60 à l'échelle des bassins et des sous-bassins. On a l'objectif en effet. D'avoir une gestion de l'eau qui associe l'ensemble des acteurs pour une gouvernance ouverte et plus efficace. 54% c'est le pourcentage du territoire qui est doté d'une commission locale de l'eau et d'un document de planification et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc les clés et les sages et des simplifications réglementaires seront apportées justement pour accélérer et généralisée à l'échelle de chaque sous-bassins versant la mise en place d'une instance de dialogue, donc la clé et d'un projet de, de politique de de territoire au plus tard en 2027, selon le principe un territoire un projet politique pour l'eau. Je crois que c'est important parce que ça va nous permettre justement de répondre à toutes les exigences du plan eau notamment sur les 10% de prélèvements. En moins parce qu'il va falloir évidemment discuté par territoire. Il n'y a pas mieux évidemment que ces échelles et les parlements de l'eau pour pouvoir les décidé évidemment par secteur, donc c'est pour ça que j'invite évidemment et vous les les sénateurs représentants des des collectivités a impulsé. Si si si la création en tous les cas de de ces sages de ses clés évidemment aussi des péter GE qui sont trop peu nombreux encore sur notre territoire. Je vous remercie. Vous avez une minute. Chers collègues de répliques. Merci madame la présidente. Merci pour vos réponses. Madame la Ministre, vous, vous nous confirmez qu'il aura quand même un relèvement des redevances existantes bien, il faut bien effectivement lactée. Je vous laisse vous indiquer que personnellement je suis très favorable à un renforcement de la planification des établissements publics de bassin joue un rôle essentiel, il faut essayer de les développer, de les conforter. Sur le plan de de territoire avec les EPAGE effectivement mettre en place des sages et faire en sorte que les clés soit aussi les parlements locaux et territoriaux de l'eau, c'est absolument important, il y aura sans doute aussi une attention il me semble à avoir sur une intégration dans les politiques d'urbanisme de la gestion de l'eau. Sans doute que les Scott les schémas de cohérence et d'organisation. Territoriale mériterait un de, d'approfondir encore plus ce sujet-là et les PLU et les PLU. Ils pourraient être concernées sur la gestion de l'eau, la gestion du fil de l'eau au bénéfice notamment du pluvial et des zones humides. Je vous invite à réfléchir sur cette proposition. Merci. Merci la parole est à présent notre collègue Madame Marie-Claude var alias du groupe communiste. Merci madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, le monde est engagé dans une nouvelle ère qui le voient confrontés à la vulnérabilité de ces écosystèmes et à des tensions accrues sur ses ressources naturelles. 40% de la population mondiale souffre de pénuries d'eau au moins une fois par an et 1,4 milliard de personnes sont privées d'accès à l'eau potable. Ces pénuries qui nous concerne aujourd'hui très directement sur notre sol nous oblige à nous saisir de l'enjeu de la gestion de l'eau durant. 32 jours d'affilée en plein hiver, la France a été pris les de pluie, ce qui va induire probablement une pénurie cet été dans de nombreuses communes en 2022 l'été le plus chaud depuis les années 50, 93 départements étaient soumis à des restrictions et plus de 1000 communes ont subi des coupures d'eau nous n'intervenons pas la situation continuera à se dégrader le GIEC l'affirme sans réduction immédiate des émissions de CO2 au niveau mondial. Tous les scénarios indique une augmentation de la température globale de 2 degrés d'ici 2050. Depuis, les assises de l'eau en 2018 en passant par le l'Avare le Varenne, de l'eau en 2021 2022, le plan sur l'eau, du président de la république aujourd'hui avant le rendu ce jour d'ailleurs du rapport de la Commission interministérielle la longue litanie des annonces faites débouche sur tout ce qui aurait dû être anticipé qui s'impose à nous, aujourd'hui le rapport travailler par nos collègues de la délégation, la porte effective auquel a participé d'ailleurs ma collègue Cécile Cukierman a le mérite d'aborder très largement la problématique de l'eau et d'apporter plusieurs solutions utile que je salue. Il est dit notamment que la mise en oeuvre concrète des actions en faveur de l'eau repose sur les acteurs locaux, les élus ont effectivement un rôle essentiel à jouer dans la gouvernance de l'eau en France dans les comités de bassin dans les agences de l'eau dans les clés en matière de fourniture d'eau potable des gestion des milieux aquatiques avec la Gemapi est encore en matière de travaux d'assainissement à cet égard, j'ai noté aussi que la question du transfert obligatoire instauré par la loi notre de la compétence eau et assainissement aux EPCI en 2026 n'est d'ailleurs pas clairement évoquée dans le plan du président de la République, malgré l'opposition de très nombreuses communes. Nous avons gagné en efficacité, en renforçant l'échelon local de prise de décision enfin de mieux intégrer la réalité des bassins de vie dans l'élaboration des GE notamment il faut redonner à nos collectivités à nos agences de l'eau qui sont la clé de voûte de la politique de l'eau, la capacité financière d'agir si la suppression du plafond mordant. C'est-à-dire du plafonnement des recettes Madame la Ministre des agences de l'eau est supprimé, on peut s'interroger sur cette annonce et 475 millions d'euros de rehaussement des moyennes des agences et leur provenance puisque leur budget n'est pas abondé par l'État, mais par les redevances des uns des Les collectivités à vous me répondrez peut-être d'ailleurs sur ce sujet. Les collectivités n'ont pas directement de capacité d'intervention sur tous les secteurs consommateurs d'eau et tout ne peut pas non plus reposer sur les usagers. Même si la sobriété s'impose. Ce n'est pas l'installation de Muster sur les robinets qui permettra d'amener un accès durable à l'eau alors que, alors même que nous perdons à cause des fuites dans les réseaux à rénover l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions d'habitants, c'est énorme. Nous ne pouvons pas opposer les usages de l'eau l'agriculture, l'industrie, le tourisme. Nous avons besoin de toutes ses activités les épisodes Selve Nole vont se multiplier, savoir retenir cette eau avant qu'elle ne ravage habitations routes équipements sera un enjeu important, même si la question fait rage en matière de récupération de l'eau, nous devons sur ce sujet, avoir un débat apaisé. On ne vole pas plus l'eau avec une retenue colinéaire qu'avec nos installations de récupérateur dans nos maisons individuelles. C'est un fait. qu'il nous faut accélérer vers l'agroécologie et Generali et généralisée, une agriculture de conservation des sols qui permet d'augmenter la rétention d'eau. Il est par ailleurs regrettable que notre pays manque d'ambition réelle pour faire en sorte que l'eau soit enfin traitée comme le bien commun qu'elle constitue et non plus comme une marchandise constituant, il faut bien le dire au marché juteux et opaque pour les multinationales. Je me souviens pourtant des paroles sages prononcé par le président de la République lors de la crise sanitaire, je le cite, il disait il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. La gestion publique de l'eau par la création d'un service public dédié doit guider notre action avec une intervention particulière et prioritaire dans les outre-mer où l'état des réserves d'eau et des réseaux d'approvisionnement est très préoccupant et je pèse mes mots, enfin la tarification sociale de l'eau visant à assurer l'accès à tous via la gratuité des premiers mètres cubes comme le préconisait la proposition de loi que j'ai porté pour mon groupe en 2021 doit, pour moi, être un objectif pour garantir ce droit inaliénable. Je vous remercie. Oui merci madame, la la présidente mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice a déjà rappelé ce que vous avez évoqué un certain nombre de de sujets rappeler les grands axes de ce plan le 1er c'est la sobriété. J'ai évoqué notamment la baisse de 10% de prélèvements. L'optimisation, le fait qu'on favorise la réutilisation des eaux usées traitées également qu'on fasse appel aux solutions fondées sur la nature. On a parlé également de la qualité, la qualité de l'eau évidemment, c'est très important avec la protection des des captages, et aussi le renforcement. De la gouvernance locale avec notamment la multiplication des des sages des clés et puis aussi des GE, tout ça, ça va nous permettre bien sûr d'aller. Définir la la politique de l'eau au niveau local et c'est bien comme ça que va être. Décidé les engagements pris, qui doivent évidemment répondre aux 10% de prélèvements en moins mais ça va permettre en tous les cas à tous les acteurs de pouvoir le décider au niveau local, vous avez parlé de la contribution qui va payer. C'est l'ensemble des usagers qui vont payer. On a été extrêmement vigilants justement à faire porter la responsabilité sur les ménages sur les agriculteurs sur les industriels. Également le secteur de l'énergie, c'est très important parce que je pense que lorsque c'est partager, c'est beaucoup mieux acceptée. On le sait par l'ensemble de la, de la population, ce sont 475 millions d'euros supplémentaires qui sont. Engagés, ça représente 20%. De, de budget complémentaire. Je crois que c'est évidemment indispensable de le rappeler, vous m'avez interrogé également sur la tarification sociale de l'eau. Vous dire que, évidemment, le sujet de la tarification sociale tarification tout court d'ailleurs c'est un sujet qui est porté directement par les collectivités. D'ailleurs, David Lisnard nous l'a rappelé, juste après la, la, l'annonce du plan eau du président de la République mais vous dire que. L'État sera aux côtés évidemment des collectivités pour accompagner cette tarification sociale de l'homme et tout ça ça doit être décidé évidemment par territoire en aucun cas l'État viendra imposer une tarification. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Jean-François Longeot du groupe Union centriste, président, vous avez quatre minutes. Il y a madame madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues. Les sécheresses et les canicules de ces dernières années l'ont assez prouvé le temps de l'abondance et de l'insouciance hydrique est révolu. Face à la raréfaction de la ressource nous savons désormais. Que nous devons changer de modèle de gestion de l'eau. Il ne faut pas être docteur en mathématiques pour poser l'équation tant elle est simple, faire mieux avec moins. La nouvelle donne hydrique nous impose de repenser notre modèle de gestion durable de l'eau d'accroître la sobriété de nos consommations et de nos prélèvements de trouver des voies pour prévenir à apaiser les conflits d'usage. Mais également d'anticiper les conséquences. D'étés plus secs pour ne pas les subir. Angle mort des réflexions d'un pays que l'on a souvent comparé à un château d'eau, la ressource en eau peut devenir dans la France de 2023 et des années à venir, un facteur de tensions, voire de conflits. Ne pas nous y préparer serait suicidaire. Les assises de l'eau et le variant de l'agricole agricole de l'eau ont préparé le terrain mais également les esprits. Le plan au conclut cette séquence de réflexion et de concertation par une série de mesures que les élus, les acteurs et les citoyens attendaient depuis longtemps. On peut certes regretter que la cible de 10% d'économie d'eau prélevée dans tous les secteurs ne soient qu'indicatives mais si toutes les toute politique est perfectible. Je sais aussi que l'action est préférable à l'immobilisme. Je note avec satisfaction la appelant le l'annonce du plan de lutte de 180 millions d'euros par an contre les canalisations fuyards de pour les collectivités ayant des rendements de réseau inférieur à 50%. Ainsi que je l'avais appelé de mes voeux en novembre dernier dans une tribune largement cosigné par des parlementaires et des élus locaux. Je suis néanmoins inquiets quant à la conditionnalité des aides qui sera appliquée car je ne voudrais pas que les collectivités les plus fragiles soient pénalisés par des excès des exigences qui serait hors de leur portée. Les élus locaux et c'est important, doivent être accompagnés, ils ne doivent pas être. Pouvez-vous me rassurer sur ces aspects et nous dire en plus sur la manière dont les aides seront attribués et seront évalués. Ces dernières semaines des articles de presse ont ravivé les préoccupations relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Les nouvelles molécules chimiques mises sur le marché, dont les effets à long terme sont mal évalué finissent par se retrouver dans les milieux aquatiques et quoi fier. Et par conséquent l'eau distribuée aux usagers. Quelles actions comptez-vous mettre en oeuvre pour rassurer sur la potabilité de l'eau du robinet et son absence de danger pour la santé à long terme. En matière d'action publique, l'État doit être exemplaire et s'appliquer à lui-même les efforts qu'il demande aux collectivités qui demande aux entreprises comment comptez-vous instaurer dans les administrations publiques, une gestion de l'eau irréprochable et mettre fin au gaspillage. Je rappelle que le parc immobilier de l'État comprend plus de 190.000 Badie et bâtiments représentant une surface d'envion 94 millions de mètres cubes. Un rapide calcul me fait arriver à un montant financier vertigineuse. Il ne s'agit pourtant que d'une mesure sur les 53, comment comptez-vous la financer et comment communiquer autour de cette exemplarité. Ses réflexions m'amène à la conclusion de mon intervention, je n'apprendrai à personne dans cet hémicycle, que sans moyens financiers adéquates. La parole publique. Les programmes d'action reste lettre morte. Vous augmenter le plafond mordant des agences de l'eau mais dans le même temps vous. Une grande partie de ces augmentations vers des mesures que vous avez identifié par ailleurs. Même si les montants annoncés par le président de la République paraissent importants les besoins annuels identifié pour le petit et le grand cycle de l'eau se chiffrent en milliards. Madame la secrétaire d'État. Ma question est toute simple. Que comptez-vous faire pour que le plan oh ne soit pas un plan qui prennent l'eau. Madame la Ministre. Monsieur le Président Longeau. Merci. Vous avez abordé longuement notamment la la conditionnalité des aides aux collectivités et rappelé que l'objectif c'est bien de soutenir bien sûr les collectivités pour atteindre une gestion performante du Patrimoine des services eau et assainissement et la conditionnalité des aides sera dimensionné pour être incitatives. Sans laisser les collectivités les plus en difficulté sur le bord du chemin. Nous ciblons dans le plan eau plus particulièrement de profil de collectivités, celles qui présentent des risques de sécurité d'approvisionnement en eau potable. Nous en avons identifié 2000 et celles qui présentent de graves défauts d'entretien des réseaux. Avec plus de 50% de fuite, j'en parlais tout à l'heure et nous en avons listé 171. ce sont celles qui ont été répertoriés et nous savons en réalité qu'il n'y en a bien plus et l'enjeu, il est d'entraîner toutes celles qui ont des performances moyennes des performances de renouvellement des infrastructures vu leur durée de vie et cette accélération sera soutenue principalement à juste prix de l'eau et la mobilisation des quoi. Prêts à taux bonifiés. De la banque des des territoires concernant le conditionnement des aides. Ce sont les agences de l'eau qui fixeront les critères selon les principes généraux posées par l'État et ses principes porteront notamment sur la conformité au regard des cibles de fuite et de qualité des rejets des eaux usées traitées et bien sûr l'idée n'est pas de pénaliser les collectivités les plus en difficulté. C'est la raison pour laquelle ces dernières qui n'atteignent pas ces critères de conformité pourront prétendre. Ah des aides si elle présente un plan correctif vous m'interrogiez, c'est la dernière question. Comment on fait en sorte que le plan eau ne prennent pas l'eau, Essayé justement de regarder la problématique et la gestion de l'eau dans son ensemble et quand on on a. On répond aux objectifs de baisse de prélèvements canton. Renforce la la gouvernance canton permet aussi d'autres utilisations, je pense à la réutilisation des eaux usées traitées, je pense également à la favorisation des solutions fondées sur la nature. Et que on est évidemment attentif aussi à la qualité de l'eau. Je crois qu'on répond à l'ensemble. Des des besoins tout en n'oubliant pas évidemment les moyens financiers. Je vous remercie. Monsieur le Président une minute pour répliquer. Oui merci merci madame le Ministre persuadé la présidente, je n'aurais pas besoin d'une minute. Je voudrais simplement effectivement rappeler une chose importante, les moyens financiers pour les collectivités. Les collectivités les attendent. Mais je crois qu'elles attendent aussi des conseils qu'elles attendent des aides parce que en matière d'assainissement en matière de structures pour traiter les eaux hé bien chaque maire et j'ai été maire je peux vous dire que c'est pas facile de prendre une décision parce que aujourd'hui il y a des nouveaux traitements à faire et il faut effectivement qu'on puisse accompagner, je ne suis pas sûr que. Et surtout. Notre collègue. Louis-Jean de Nicolaï, je ne suis pas sûr que la. Soit en capacité d'accompagner complètement pour que un conseil municipal une commune prenne une décision bien adapté pour le traitement de ces eaux usées. Merci la parole est à présent notre collègue monsieur Éric goal du groupe RDSE. Et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Madame la Ministre, monsieur le président de la délégation de la prospective, chers collègues. Après les affrontements de Sainte-, Soline le 25 mars. Ce débat sur la gestion de la ressource en eau s'avère cruellement d'actualité. Sainte-, Soline n'est pas une affaire d'écologistes et d'ultragauche, mais doit amener la manifestation d'un débat de fond et d'une véritable inquiétude. Dans un contexte de pénurie croissante. L'eau va-t-elle enfin être gérée comme un bien commun à préserver. Jusqu'ici, nous vivons dans un pays où l'eau coulait en abondance. Elle nous permettait de prélever jusqu'à 35 milliards de mètres cubes par an sans avoir à remettre en cause notre modèle. Mais après plusieurs épisodes de sécheresse et la confirmation d'une trajectoire inquiétante du réchauffement climatique. Des tensions autour du partage de cette ressource font surface. Cependant qu'on ton réellement la situation et à mesure de quête de quantifier l'état de la ressource en eau. Le sentiment général Madame la Ministre et qu'on se réveille quand c'est déjà trop tard alors que les cours d'eau sont à sec que les nappes phréatiques sont au plus bas et que les prévisions à moyen terme ne sont pas plus optimistes. Sous l'effet du réchauffement climatique, les précipitations vont diminuer d'évaporation va s'accentuer dans le même temps, l'augmentation de la population mondiale accroît les besoins en eau les pressions qui s'exercent sur les gestionnaires de l'eau en ville s'intensifie en zone rurale, c'est le partage et les conflits d'usage qui pose des problèmes croissants. Parallèlement, les besoins en énergie et en alimentation augmente, alors que le refroidissement des centrales nucléaires et l'agriculture sont de très gros consommateurs d'eau. Alors qu'est-ce qu'une gestion durable de l'eau. C'était en capacité de reconstituer les stocks chaque année. C'est ne pas puiser plus que l'alimentation annuelle des réserves souterraines et de surface et ce alors même que les glaciers fondent ça se reconstituer. Pour cela, nous avons d'abord tout un modèle à revoir le modèle économique des agences de l'eau déjà qui n'incitent pas suffisamment une utilisation rationnelle de l'eau. Le plan au prévoit le déplafonnement des dépenses des agents. À élargir les contributeurs pour conserver une logique de pollueur-payeur. C'est une tarification progressive et responsabilisante de l'eau peut aider à faire baisser la consommation des ménages, le financement de la politique de l'eau ne peut continuer à reposer entièrement sur eux. L'objectif de réduction de 10% des prélèvements par rapport à 2019 dans tous les secteurs semblait une première accroche. Nous regrettons toutefois que cette ambition affichée pour 2025 lors des Assises de l'eau se reporter en 2030. Dans tous les cas. Un objectif ni rien s'ils ne s'accompagne pas de moyens à la hauteur. Le plan oh nous apporte quelques réponses avec 500 millions d'euros supplémentaires chaque année pour les agences de l'eau, 100 millions pour les pratiques vertueuses agriculteur ou encore 100 millions du Fonds Vert pour des projets de renaturation des collectivités. Une grande campagne de sensibilisation et d'accompagnement des particuliers viendra compléter cet arsenal pour couvrir l'ensemble de la chaîne de consommation. Pour ma part je défends un modèle ou l'État fixe un cap ambitieux associée à des moyens suffisants tout en laissant la main aux collectivités territoriales. C'est un modèle unique. Car un modèle unique ne saurait être appliquée sur tout le territoire, il nous faut des approches intégrées par exemple avec une gestion par bassin ou par écosystème. Il nous faut achever l'évolution de la gouvernance de l'eau pour que tous les acteurs définissent ensemble les priorités de leur bassin pour éviter les conflits et garantir une utilisation de la ressource, en fonction des besoins prioritaires. Sur la question très sensible l'irrigation riziculture les quantités autorisées, doivent être définis par les agences de l'eau en lien avec les chambres d'agriculture, mais aussi les associations locales pour faire baisser le niveau de tension, de tels projets de territoire. Pourrait nous éviter de nouveaux Sainte-Soline. Il nous faut également mieux accompagner les élus locaux parfois démuni face aux enjeux, notamment dans les petites communes hors syndicats. Il faut les aider à mieux identifier financer et mettre en oeuvre leur projet. Enfin des solutions très concrètes sont évidemment à développer la technologie nous offre des opportunités intéressantes dans tous les secteurs où et l'irrigation, de précision, le goutte-à-goutte enterré ou les drone en en capteur en agriculture. La réutilisation des eaux usées doit faire figure Le président a fixé l'objectif de passer de un à 10% d'eaux usées réutiliser notamment le vent certains verrous administratifs. Quand on sait qu'Israël réutilise 80% de ses eaux usées et que nous continuons à utiliser de l'eau potable pour arroser le jardin, il y a aussi une absurdité a levé je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes.

c'est que en fait ça a permis de que tout le monde prenne conscience. Ça permet évidemment de, de sensibiliser les les les citoyens sensibiliser les élus, je vois qu'on a jamais eu autant de débats sur le sujet de l'eau et moi je m'en réjouis et bien sûr que le sujet est remonté et fait la préoccupation du gouvernement, donc c'est aussi pour ça que on agit. Les 10% de prélèvements avaient été anticipée parce que nous avions déjà c'était la la ministre Emmanuel wagons qui avait déjà à l'époque. Annoncé la baisse de 10% de prélèvements, maintenant moi je nous venons annoncé la manière dont nous allons-y parvenir. Je crois que. L'effort partagé et bienvenue. Le fait que ça puisse reposer sur l'ensemble, l'ensemble des acteurs. Il y a aussi des des solutions techniques qui peuvent être apportées à cela pour justement atteinte, c'est 10% de prélèvements en moins, c'est d'utiliser une eau qu'on a déjà utilisé, et donc c'est la réutilisation des eaux usées traitées, ça a été dit, nos voisins savent très bien le faire il y a pas de raison et surtout qu'on a les entreprises françaises qui le font à l'étranger, alors pourquoi pas chez nous donc le la participation de l'ensemble des collectivités aussi de l'ANEL pour favoriser ces solutions sur les communes littorales. Et bienvenue, parce que ça va nous permettre d'accentuer évidemment cette dynamique et le fait de. Faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de contraintes réglementaires va aussi nous permettre d'accélérer parce que je sais c'est ce qui remonte des territoires c'est que l'envie de bien faire mais maintenant c'est donner aussi les moyens et notamment les moyens réglementaires pour ne pas être empêché de mettre en place ces solutions sur les territoires. Merci. Vous avez une minute, chers collègues. Je vous remercie madame la présidente, madame la ministre, je vous remercie évidemment pour votre réponse. J'en profite pour vous dire qu'au vu des tensions croissantes autour justement de la ressource en eau. Peut-être une mise à jour de la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques serait utile, c'est-à-dire une mise à jour sur la priorité des usages pour rappeler à chacun que dans un contexte de pénurie l'accès de la ressource pour tous et la biodiversité seront nos priorités. Merci la parole est à présent rapporteur Monsieur Jean-François Husson. Madame la présidente, madame la Ministre, Monsieur le président de la délégation, mes chers collègues. Effectivement été 2002 historiquement sec qui a donné l'occasion de controverses récurrentes liées tantôt partage de l'eau mais aussi. Si on regarde le printemps aux inondations à répétition, la question de la gestion de l'eau cet invité s'invite plus que jamais dans le débat public. Ce dont je me réjouis. Cette eau nous devons préserver l'intégrité et la pérennité et la préservation ne pourra se faire qu'avec la mise en place d'une gouvernance. Bonsoir. Et donc. Fort d'un regard rétrospectif. Il m'apparaît qu'il serait bien venu tout d'abord. De recréer des services d'ingénierie de l'eau dans tous les territoires. Sans aucun doute la dégradation de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau et d'assainissement et réel, la disparition de l'ingénierie publique j'ai regardé dans mon territoire, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. C'est sur la période 2012 2022, 25% de suppressions de postes en conséquence c'est c'est assez logique. Les collectivités locales connaissent aujourd'hui des difficultés dans leur choix d'un mode de gestion et d'assainissement. Étant d'ailleurs trop souvent livrées à elles-mêmes. Il est donc essentiel de reconstitue une ingénierie territoriale spécialisé dans le domaine de l'eau qui soit à la fois facilement mobilisables par le plus grand nombre des collectivités. C'est d'abord une question d'équité entre les territoires. La piste d'une ingénierie de proximité. Articulé entre les acteurs. peut être d'ailleurs en leur bien sûr laissant le choix mutualiser au niveau des structures intercommunales méritent d'être explorées pour aboutir à des. Propositions d'amélioration fonctionnelle mais également de performance de service l'émergence d'une nouvelle ingénierie et me semble-t-il la condition nécessaire pour améliorer la gouvernance du service public de l'eau. Ah si et c'est mon 2ème point nous pourrons stimuler les mécanismes de solidarité pour rattraper le retard d'équipement en matière d'eau et d'assainissement. Et notamment en mi-rural. Sans revenir d'ailleurs sur le caractère obligatoire de la loi. Il serait utile de faciliter la remise à niveau des infrastructures d'eau et d'assainissement en cas d'intégration d'une commune à une intercommunalité trop souvent le rattrapage d'investissement est telle que cela freine l'adhésion soit le ticket d'entrée est trop important, soit la solidarité forcée de l'intercommunalité d'accueil trouve ses limites. Or l'intercommunalité en matière d'eau, grâce notamment aux mécanismes du budget annexe qui permet de programmation pluriannuelle et dans l'absolu, un bon vecteur de modernisation des infrastructures et de professionnalisation des services nous pourrions imaginer un contrat de transition permettant de réaliser dans des conditions apaisées soutenable des adhésions volontaires à des structures intercommunales. À la fois par des logiques de performance de service et dans lesquels les agences de l'eau trouveraient naturellement leur place. Occasion c'est le 3ème point dès lors de fixer les conditions d'une transformation des usages. Et d'un partage des ressources en eau grâce à un dialogue territorial renouveler que j'appellerai en vision à 360 degrés. Le changement climatique impacte et impactera durablement les ressources en eau. Les projections donnent une baisse moyenne de la pluviométrie dans la plupart des régions de France, à part le Grand-Est, d'ailleurs avec une variabilité interannuelle très forte le sage issu de la loi de 92. Porter une ambition claire et ambitieuse, permettre aux élus mais pas seulement à eux de prendre en considération la nouvelle situation climatique pour définir dans leur bassin, les scénarios prospectifs d'aménagement. Là où les conflits d'usage était prégnant cette forme de démocratie locale était pionnière et a montré son intérêt. Elles permettent en effet de concilier les usages au disponibilité en eau et aux aléas. Il faut certainement Madame la Ministre lui donner un souffle nouveau. C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui réinventer les sages en imaginant des formes plus souple de gouvernance en tirant les enseignements de leurs échecs ou de leurs limites en gros en ayant un plan d'action opérationnelle. Dès lors, et pour terminer nous devons réinvestir dans l'innovation, parce que nous devons nous poser une question, comment en étant arrivé à couper les ailes de nos entreprises spécialisées dans la gestion de l'eau et qui incarnait une excellence technologique à la française. en retard par rapport à nos voisins européens. Je vais parler d'l'Italie de l'Espagne en terme de réutilisation et ça a été dit des eaux grises et des eaux usées. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un volet au au sein du programme. France 2030. Or c'est bien dans ces territoires que le renchérissement du coût de l'énergie. Ah les effets les plus marquées sur les services d'eau et d'assainissement ou qu'il existe les pressions non traitable du fait de la faiblesse des services. Moins intégrée, madame le Ministre, j'ai évoqué 4 orientations à propos desquels le gouvernement je le devine par votre voix va et j'en suis certain, faire connaître la suite qu'il entend y donner. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre, vous avez Dominique de répliques. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le le sénateur Husson déjà je tenais à vous remercier pour les propositions que vous venez de faire. J'espère que vous aurez l'occasion de réitérer et de les compléter dans le cadre de la mission parlementaire qui va être lancée. Je pense que c'est l'occasion de pouvoir aborder notamment la possibilité justement de, de renforcer la gouvernance locale sur le sujet de l'eau. Je crois qu'elle est appelée. Des voeux de, de tous les, de tous les élus locaux et de tous ceux qui participent justement au Parlement de l'eau je il y a une la nécessité de renforcer la gouvernance locale. Vous avez abordé de sujet, le sujet des moyens et également l'ingénierie d'État et l'ingénierie publique. Sur les moyens. Je rappelle quand même que les agences de l'eau sont dotés de 2 2 milliards d'euros le plan eau vient y ajouter 475 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Je l'ai dit tout à l'heure, ça représente 20% d'augmentation. Ah ça, il y a une, une enveloppe de 180 millions d'euros par an supplémentaires qui est là pour aider justement les communes en difficulté pour sécuriser. Leur approvisionnement en eau potable via des travaux d'interconnexion de résorption de de fuite ou encore de de forage de de de secours. 100 millions d'euros qui ont été renouvelés cette année pour justement répondre au risque de sécheresse et encore 400 millions d'euros qui correspondent justement à une nouvelle génération d'Aqua près qui vont pouvoir être déployés. Sur plus de d'un d'un milliard d'euros dans les territoires.

d'où l'intérêt, et je réitère mon propos par rapport à la première question qui m'a été posée l'intérêt de mutualiser, même si le sujet n'est pas forcément l'intercommunalité mais bien de mutualiser pour pouvoir justement. d'avoir les moyens nécessaires pour assurer l'ingénierie. Il reste malgré tout une oeuvre d'ingénierie d'État. C'est l'intervention du CEREMA la gouvernance de l'établissement a connu d'importantes évolutions de en 2022 en application justement de la loi 3DS c'est aujourd'hui un établissement partagée par l'État et les collectivités et l'établissement pourra apporter justement un appui pour accompagner les projets les plus complexes. Je tiens à souligner avant de de de qu'on a obtenu également que les ETP du pôle ministériel ne baisse pas pendant les 5 prochaines années. Vous savez que c'est pas toujours simple de l'obtenir, il nous sommes très heureux de l'avoir fait avec Christophe Béchu. Merci monsieur le rapporteur. Vous avez une minute de répliques. Je ne sais pas ce sera suffisant mais Madame la Ministre j'ai écouté vos 2 éléments de réponse le premier j'ai l'impression qu'on était à Gravelotte. Il tombe, il pleut des millions ou des milliards. Je ne suis pas sûr que. Pour nos concitoyens et pour les élus se soit le seul élément de réponse. Et accessoirement, vous avez oublié signaler que ici nous avions obtenu au moment du budget, 50 millions d'euros supplémentaires. De la part de l'État ce si vraiment décaisser contrairement aux 100 millions que la ministre. La Première ministre avait demandé de débloquer. Au niveau des agences de l'eau et puis le 2ème sujet qui touche à l'ingénierie. Je pense que vous vous trompez d'abord le CEREMA rencontre de grandes difficultés pour pouvoir intervenir dans les communes de moins de 2000 habitants parce qu'il a un problème de ressources techniques. C'est la même chose pour les agences de l'eau, il ne faut pas qu'on se renvoie la balle. Vous parlez d'un parlement de l'eau, hé bien je pense, je le redis qu'il faut avoir une vision à 360 degrés qu'il faut regarder objectivement les choses. Il y a une solidarité urbain rural qui joue d'ailleurs dans le prélèvement des recettes au bénéfice des territoires ruraux. Mais il faut il faut pardon, aller plus loin et ne pas se à mon avis se contenter de de bien n'exprimer les choses dans notre assemblée mais voir concrètement sur le terrain les efforts qui doivent être déployés pour remédier à la situation de d'une gestion publique de l'autre qui ne me paraît pas tout à fait au bon niveau aujourd'hui. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Madame. Marta de si. Si drague pardon du groupe Les Républicains Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues. Autrefois abondante dont marché est disponible la ressource en eau, fait face à une situation d'une gravité historique. Sous l'effet du réchauffement climatique, elle se raréfient. Selon l'étude explore 2070 le dérèglement du climat aura pour effet de réduire la pluviométrie en été, de 16% à 23%. La France ne sera pas épargné, baisse des débits des cours d'eau, temps de recharge des nappes allongé sécheresse des sols. Notre pays connaît déjà des périodes de stress hydrique inédite dans son histoire. Pourtant rien ne nous prédisposait à connaître une telle situation ni notre climat ni notre. Hydrographie depuis plusieurs années, nous aussi on en traiter caniculaire et sécheresse précoce avec des conséquences parfois dramatiques. Cette ressource fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses tensions qui demande en tant que législateur, toute notre vigilance. Stocker l'eau à des fins agricoles ou laisser les nappes phréatiques se recharger sans retenue. Un exemple parmi tant d'autres, comme à Sainte-, Soline où une véritable bataille pour l'eau a eu lieu et qui illustre au-delà des postures une problématique parmi de nombreux autres et qu'il est impossible d'ignorer. Dans ce souci de projections et d'anticipation. Je salue le travail des rapporteurs de la délégation sénatoriale à la prospective pour leur excellent rapport sur l'eau qui est clair, un sujet danse et brûlant. On observe à quel point la question de l'eau en France est devenu un sujet qui nous concerne tous et nous n'avancerons pas en tenant nos concitoyens à l'écart de toute forme de démocratie locale autour de l'eau. Je sais que la tentation est forte de rester sur une approche purement technique et technocratique, mais nous devons développer une approche pédagogique et citoyen du problème tout en étant attentif aux territoires et à leurs besoins. La loi de 1964 qui font notre modèle français de gestion de l'eau institut un principe bien connu l'eau paye l'eau, or aujourd'hui un tel principe n'est plus respecté pour reprendre les mots de mon collègue Mathieu Darnaud que je salue. Aujourd'hui l'eau paye l'État face aux nouveaux enjeux climatiques. C'est toute une stratégie qu'il faut repenser et accompagner. Oui mais il y a le plan d'eau, me direz-vous. Madame la Ministre. Plusieurs fois reportée, il a finalement été présenté par le président de la République le 30 mars dernier. Et permettez-moi de saluer ceux dont les travaux de réflexion d'auditions et de prospective ont de longue date préfigurer ce plan d'eau. Notre délégation sénatoriale bien sûr mais également l'association nationale des élus des bassins les collectivités concédantes et régies. Le comité national de l'eau ainsi que le Centre d'information sur l'eau le plan présidentiel n'arrive pas de nulle part et tant mieux, il dresse un certain nombre des problèmes identifiés de notre gestion de l'eau et propose différents axes. J'ai été particulièrement sensible au 3ème intitulé investir massivement dans la réutilisation des eaux usées. 90 sont très en retard en la matière, notamment en comparaison des pays d'Europe du Sud, confrontée depuis plus longtemps que nous aux problématiques de l'eau. Les logements français doivent pouvoir réutiliser les eaux grises et les eaux pluviales notre pays comporte des champions mondiaux du traitement des eaux. Nous devons les associer pleinement et encore plus à cet effort et ne pas les déstabiliser, comme ça a pu être fait par le passé. Notre modèle de gestion de l'eau a besoin de transformation pour coller aux enjeux climatiques et environnementaux mais doit conserver certaines spécificités françaises. Une eau potable disponible pour tous sans distinction sociale mais où chaque citoyen doit être contributeur à hauteur de ce qu'il consomme. Certains grands pays comme les États-Unis voient la potabilité de l'euro reculait dans certains États. Face au coût de traitement. La vétusté des réseaux, le manque de moyens des problèmes que nous connaissons, hélas également dans nos territoires, madame la Ministre, soyons exigeants et économe et rappelons-nous d'adapter chaque ou à son usage. Cela a été rappelé par beaucoup de mes collègues, mais également chaque usage à la disponibilité de l'eau. Je vous remercie, cher collègue. Merci. Madame la Ministre. Vous avez 2 minutes pour répliquer. Vous avez rappelé un certain nombre d'éléments, peut-être pour éviter d'être d'être redondantes. Davantage peut-être parler d'un sujet que je n'ai pas évoqué notamment le sujet de la réutilisation des des eaux de pluie. C'est un sujet qui est important parce que c'est quelque chose que nous souhaiterions non pas généraliser mais en tout le cas permettre qu'il puisse y avoir un déploiement beaucoup plus important sur les logements, ce que vous avez abordé cette question. Jusqu'à aujourd'hui, il était très difficile de le mettre en place pour un particulier, alors que c'est quelque chose qui pourrait très facilement en fait être être déployés et pour ça il faut qu'on simplifie en fait un certain nombre de de de pratiques. Et que on a d'ailleurs travaillé avec un soutien politique important de la part de d'Agnès Firmin Le Bodo, pour faire en sorte auprès des des services du ministère pour faire en sorte justement de faciliter. Cela et donc il sera possible beaucoup plus facilement de récupérer les eaux de pluie pour pouvoir alimenter les chasses d'eau. Par exemple des des des logements. Je pense que ça c'est important parce qu'en fait, ça peut paraître assez anecdotique mais malgré tout une quand c'était une quantité d'eau importante pour les ménages et donc ça permettra en tous les cas, de faire en sorte que chacun participe notamment à la sobriété. Vous avez appelé près sur les autres sujets a rappelé les grands enjeux, notamment la réutilisation des eaux usées traitées, le fait qu'il ait 10% de prélèvements en moins. Et que ce soit de façon beaucoup plus partagés. Et que chacun participe en fait à son niveau et je crois avoir eu l'occasion d'y répondre dans les différentes questions vous dire que c'est un plan. Oh ambitieux en effet il a été retardé, mais je crois qu'il est à la hauteur et qu'il a il pense pas la

avec notamment le renforcement de la gouvernance locale. Le fait qu'on travaille à l'optimisation justement de la ressource. La la sobriété. Tous ces sujets qu'il faut qu'on arrive à à engager et c'est vrai que c'était prévu fin janvier on a décalé légèrement. Courant fin fin mars début avril. Mais je crois que c'était nécessaire pour justement aussi obtenir les arbitrages financiers indispensables merci pour justement réussir. Pardon, vous vouliez répliqué chers collègues au sujet de cette ressource qui est précieux. Cela a été rappelé par l'ensemble des collègues qui se sont exprimés avant moi et qui sans doute continuera à s'exprimer. Dans ce sens donc je souhaitais simplement attirer votre attention sur cet aspect-là un bon usage et pour préserver, toujours cette eau qui nous est si précieuse, merci. Merci la parole est à présent à Madame. Florence Blétry compta du groupe socialiste, vous avez quatre minutes, chers collègues. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, je remercie la délégation à la prospective d'avoir initié ce débat. L'été 2022 s'est caractérisée par des records de chaleur et de sécheresse. L'hiver 2023, quant à lui se classe déjà parmi les hivers les plus sec avec un déficit de pluviométrie de 50% L'été 2022 a compté près de 500 communes concernées par des problèmes d'approvisionnement en eau potable, selon les dires du ministre de la transition écologique et l'été 2023 risque d'être pire si l'on en croit le le rapport mais interministériel de ce jour sans action forte et déterminée des pouvoirs publics. La gestion de la ressource en eau devient crucial pour la satisfaction d'un besoin essentiel que l'on croyait définitivement acquis, l'accès à l'eau potable mon interpellation portera sur la gestion du petit cycle de l'eau et en particulier sur la question des captages et leur protection nombre de collectivités sont aujourd'hui concernés par des problématiques de qualité des eaux brutes prélevé la protection des captages est une préoccupation croissante des gestionnaires de de services publics d'eau potable car la détection de pollution diffuse et de plus en plus fréquentes. Suite au Grenelle de l'environnement en 2009 un peu plus de 500 captages ont été désignés comme prioritaires sur la base notamment de l'état de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses et du caractère stratégique de la ressource en 2013 500, nombreux ouvrages prioritaires ont été identifiés. L'intérêt de cette classification résidait dans la gestion concertée de Césaire et la prévention des pollutions diffuses des diagnostics permettent de mieux connaître les vulnérabilités les modes de contamination subis par ces captages et des programmes d'action adaptées aux objectifs d'amélioration de qualité des eaux sont élaborés en partenariat avec avec les chambres d'agriculture. Ils comprennent la plupart du temps des mesures agro-environnementales. Cette stratégie qui a démontré son efficacité devrait être étendue. Alors qu'elle ne concerne que 1000 captages sur les 35.000 recensés en France. Par ailleurs, la directive eau potable sera transposé prochainement par ordonnance. L'ordonnance que nous aurons à examiner vise le déploiement d'une démarche préventive pour garantir la qualité de l'eau jusqu'au robinet du consommateur avec l'obligation de réaliser un plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau pour les personnes responsables de la production de la distribution de l'eau, c'est d'ailleurs une des mesures du plan eau du gouvernement. Donc première question, comment les collectivités, madame la Ministre seront-elles accompagner dans cette Par ailleurs, l'ordonnance vise également à une rationalisation des périmètres de protection de captage en réformant la politique de préservation de la ressource en eau des captages sensible aux pollutions par les pesticides, mais aussi prévoit la possibilité de contribuer à la mission de préservation de la ressource en eau pour pour les collectivités qui le souhaitent, en liaison avec le préfet afin d'établir un programme d'action encadrant les pratiques qui dégradent la qualité des points de prélèvement ses programmes d'action. En général, sur les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines. D'occupation des sols ou certains entrant. S'agit-t-il comme nous le souhaitons d'une. Extension de la politique des captages prioritaires les préfets disposeront-t-il de moyens pour interdire l'utilisation d'entrants notamment les pesticides et comment les agriculteurs danser seront accompagnés dans cette transition et surtout comment développer les baux environnementaux qui sont encore trop peu utilisé. L'eau est le miroir de nos sociétés les Liens que l'on montre que l'on entretient avec elle disent en creux ce que sont nos sociétés. Ces mots sont d'Erik Orsenna. Notre engagement dans la préservation de l'eau dira qu'elle ne société nous voulons-nous. Dans le cas de la mission, nous nous attacherons à y contribuer. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame la la sénatrice. Je peut être vous répondre sur davantage sur le le le sujet des de la baisse des pesticides. Qui qui évidemment souhaité par. Une grande partie d'entre nous en tout cas, je peux dire. Que quasiment sur tous les bancs. Parce que on a déjà commencé, cette baisse depuis depuis 2017 parce que là il y a une baisse. Notamment des de la vente des des produits phytosanitaires et c'est aussi les résultats concrets de de de la mise en oeuvre des plans Ecophyto le gouvernement. Il travaille notamment activement à ce changement de méthode pour qui consiste en fait à à anticiper le retrait des des substances actives potentiellement problématiques également renforcer le le pilotage et l'adaptation des techniques de protection des cultures pour soutenir nos agriculteurs dans dans les transitions et pour ça, ça passe par 3 principes d'action simple le 1er c'est je crois de, de pouvoir aligner les calendriers français et européens et défendent la mise en place des clauses miroirs parce que nous ne souhaitons pas évidemment consommer des produits qui entrerait sur notre territoire qui. Aurait été cultivée avec des produits phytosanitaires qu'on aurait nous-mêmes interdit sur le nôtre, je crois que c'est une exigence sanitaire et également une exigence. Environnementale qu'il nous faut arriver il faut qu'il y ait une concordance le 2ème principe c'est de mettre en oeuvre. La recherche de de solutions alternatives j'évoquais notamment le sujet du du du biocontrôle mais il y a aussi le évidemment des recherches qui sont réalisées par l'INRA et et les instituts techniques qui développe justement des des solutions, il faut qu'on continue à accompagner nos nos nos agriculteurs qui vont connaître la suppression d'un certain nombre de produits encore à venir et on doit être en capacité de les accompagner 3ème principe c'est bien sûr la gouvernance. On assume d'avoir refusé la réintroduction de de substances actives interdites et en même temps d'avoir. Aussi. Fait en sorte de d'accompagner la décision qui a été prise sur les néo-que thyroïde ça ne voilà. L'un n'empêche pas l'autre et sur le sujet des des captages, j'ai déjà répondu à la sénatrice Paoli et et le temps me manque pour pouvoir vous répondre. Merci madame la ministre. Bien entendu, on a vu avec le dernier rapport de l'an 2 cesse. La rémanence de certaines molécules après leur interdiction impose vraiment une anticipation. Et si on veut éviter d'être dans une logique curative qui sera très coûteuse pour nos collectivités et donc pour les consommateurs, il faut davantage anticiper et dans ce sens-là la préconisation de l'de cesse de retirer le S-métolachlore semble être utile et ce sera une très mauvaise idée pour le gouvernement de revenir sur le sur ce retrait et d'ailleurs nous insistons beaucoup sur. L'indépendance de cette agence et de ses décisions plus généralement il faut accélérer à accélérer la transition de notre agriculture vers l'agro-écologie en accompagnant bien entendu les agriculteurs ce qui permettra de concilier résilience de notre agriculture et préservation de notre source. Merci la parole est à présent à notre collègue. Monsieur Pierre Louvot du groupe Union centriste. Et vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues. Je voudrais aborder. La fin de ce débat sur la gestion de l'eau comment retrouver une ressource plus abondantes, les autres sujets ont été abordés pas fait lui. Je crois qu'aujourd'hui le niveau des rivières baissent les nappes s'épuise et depuis 70 ans on accumule un certain nombre de fautes dans les années 60 70 on a créé des fossés profonds on a approfondi et mis affecte les ruisseaux. Dans les années 2000. Nouvelles directives européennes qu'on a interprété à la française avec une loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Appeler de manière pompeuses, la continuité écologique continuité. Seulement pour les poissons migrateurs mais enfin, relever les 20 Fidan. En même temps il y a eu une sur-interprétation administrative qui fait pratiquement jurisprudence. Aujourd'hui, on a supprimé les feuilles sur les cours d'eau on abaisse le niveau de l'eau, on vide les rivières très souvent. On vidange les nappes phréatiques. On vidange les nappes phréatiques. Allez je suis paysan c'est le système de l'Abreuvoir a poulet. Vous enlever 50 centimètres d'eau, les nappes se vidange. L'abreuvoir a poulet de centimètres d'eau retiennent un mètre d'eau des nappes phréatiques. C'est exactement le même système. Et si bien que dans le même temps, les prairies humides sont devenus des vrais paillasson. Les zones humides sur notre territoire qui étaient des. Sont en train de disparaître. Et on continue maintenant après avoir pratiquement et. Épuisé les feuilles de rivière. On est en train de vouloir supprimer les étangs qui ont quelques fois, plus de 5 ans, 500 ans d'existence à la bonne raison que le cours d'eau passe au milieu de l'étang. Je crois qu'à travers. Tous ces systèmes mis en cascade. On épuise les réserves d'eau. Les rivières, les ruisseaux sont de plus en plus abondants l'hiver quand il pleut. un Avantage c'est que ça contribue pour sa part à rehausser le niveau des océans qui en ont grand besoin. Et on a de moins en moins d'eau l'été. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui c'est un défi, un vrai défi et je puis vous dire que par un certain nombre d'expériences que j'ai mis en place sur ma commune et mon territoire, tout simplement en rétablissant des feuilles sur Desfossés créée dans les années 60, on a retrouvé des sources qui ne coule pas que l'hiver mais qui coule toute l'année et on a rétabli des ruisseaux. Je voudrais vous dire également que je ne suis pas. Un anti-écolo. Je fais partie de quelques fois. Je voudrais vous dire que sur ma commune en 20 ans j'ai planté 7 kilomètres de rivière j'ai recréé de toutes pièces des zones humides et on retrouve de l'eau toute l'année dans des endroits qui étaient à sec. Mais par pitié arrêtons. Au nom de je sais pas quelle idéologie de vouloir mettre à tout prix les rivières à sec. Sans. La moindre expérimentations. par principe on supprime les feuilles. Au lieu de les rétablir dans une continuer écologique ou les poissons migrateurs pourrait passer. C'est tellement plus simple de les supprimer. Et voilà où va la moitié de l'argent de l'Agence Ça n'est plus possible et je voulais tout simplement vous alerter sur ce problème qui. S'il perdure. Hé bien aggravera encore un peu plus. La capacité de nos rivières, la capacité de nos nappes de ce rachat recharger aujourd'hui nos nappes se vide, l'hiver et n'ont plus rien à donner. L'été c'est une vraie réalité. Alors c'est sans doute trop compliqué pour la haute technostructure. Mais je crois qu'il va être temps d'y jeter un coup d'oeil. Ça va. Merci de vous inquiéter pour moi, bonjour. Merci madame la présidente. Vous avez abordé la politique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau. une est une politique évidemment qui qui vise en fait à, à limiter la fragmentation des habitats naturels. C'est une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité. dans ce ministère nous défendons évidemment les continuités écologiques et au-delà d'avoir cette pensée que vous appelez technocrate quelque part. Moi j'ai envie dire que j'ai envie de défendre l'avis scientifique et l'avis scientifique, il est assez clair sur le fonctionnement des des systèmes hydro-hydrologiques. Je pense que on n'accorde. Et même sur l'ensemble de ces bancs, justement. Une importance de l'avis scientifique et j'ai avec moi et je pourrais vous le donner. Un avis qui est produit par le conseil scientifique de l'OFB qui date de 2018 et qui, face aux multiples interventions sur la gestion de de des cours d'eau et des ouvrages avaient procédé justement à certaines clarifications j'invite d'ailleurs toutes les personnes intéressées à en prendre de connaissance. Cet avis il il tend à infirmer les conséquences que vous avez décrite notamment. Et moi je ne pose pas. Cette politique de restauration du grand cycle de l'eau avec l'idée de stockage pertinent. Dans l'espace et le temps et les ouvrages font partie du panel de de solutions de la gestion de l'eau et peuvent répondre des besoins locaux. Moi je crois qu'il faut pas opposer les projets et c'est juste que les projets doivent être regardées au cas par cas et en tout cas la la voix du du ministère de la transition écologique, c'est et surtout les continuités écologiques et aussi regardons les réserves de substitution on les réserves collinaires qui peuvent être adéquate pour les territoires. Merci monsieur eau une minute pour répliquer. Oui madame. Défendiez vos services mais. Est-ce qu'on peut qualifier les agents de l'OFB de scientifiques. Et ce qu'on aurait le droit. Quand même dans ce pays d'expérimenter. Au lieu et de regarder ce qui se passe réellement. Quand on a des rivières qui était pleine avec des prairies humides qui sont secs comme des paillassons avec des roses qui disparaissent. Est ce que l'OFB vous à quelques fois parler de ça non parce que ça les dérange. Par contre l'OFB a fait une interprétation une sur-interprétation de la loi elle ne regarde que ce qui est dans la bonne lignée. Elle pénalise ce qui est contraire à la lignée qu'ils ont interprété et ne font rien d'autre. Aujourd'hui on va dans le mur, mais ça n'est pas grave, je commence à être âgés. Je ne m'en apercevrait peut être pas, mais je crois qu'il vaudrait mieux y regarder d'un peu plus près. près. La parole est à présent à Madame. Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le président de la délégation à la prospective mesdames et messieurs les les sénateurs tout d'abord je voulais vous dire merci, merci pour la richesse de ses échanges. Merci encore pour la qualité aussi des travaux qui sont réalisés. Par la la délégation sénatoriale à la prospective qui sont toujours des travaux dont je prends connaissance, avait beaucoup d'intentions bien sûr aussi tous les travaux. Qui sont réalisés par par les sénateurs parce que le sujet de l'eau est un sujet qui a été. Particulièrement aborder depuis le début de de cette année. En tant que député, moi-même je considère le le travail parlementaire comme une source de d'inspiration et de réflexion et je crois en l'Intelligence collective d'autant plus que, face aux grands défis de l'adaptation au changement climatique. Je crois que c'est dans cet esprit que nous avons construit le plan eau nous allons d'ailleurs continuer j'espère ensemble à co-construire que ce soit dans la mise en oeuvre du plan ou dans le cadre de la mission parlementaire qui a été annoncé la ressource en eau est un enjeu de souveraineté nationale. Une eau en quantité et de qualité est essentielle pour notre environnement pour notre. Ressentez pour notre économie. Ça a été dit et je pense qu'aujourd'hui, notre société est prête pour échanger pour engager, je veux dire là un changement de rapport à l'eau. La trajectoire collectif de sobriété, de moins 10% à horizon 2030, nous allons la déclinés par territoire avec les élus, avec les acteurs locaux et par secteur avec le représentant des filières, c'est un plan qui engage l'ensemble des acteurs particuliers, industrie, agriculture, tourisme, secteur public dans une même dynamique. Le débat que nous avons eu aujourd'hui qui est le reflet du contenu de votre rapport montre à quel point le sujet est vaste et aussi complexe. J'ai noté particulièrement vos questions sur les moyens pour les collectivités d'agir dans la préservation du grand cycle de l'eau. J'ai également pris en compte la question de la mise en cohérence des échelons de gouvernance et la nécessité d'avoir un dialogue renforcé entre les instances de définition des politiques publiques territoriales. Enfin, et cela me tient à coeur tant les marges de progrès sont importantes, mais aussi réjouissante. Vous avez mis au rang de priorité la levée des freins parfois réglementaires à l'innovation, comme sur le sujet de la réutilisation des eaux usées. J'ai pu, je l'espère vous montrer que le plan eau apporte des réponses concrètes et ambitieuses à l'ensemble des préoccupations que vous avez exprimé aujourd'hui. Je suis assez fier, oui, je dois dire du résultat. Qui a été réalisé un travail interministériel qui a été intense. C'est le premier exercice de planification écologique qui a piloté par la Première ministre et qui a démontré justement l'intérêt de cette méthode. Je suis encore plus fier des moyens qui sont apportées en faveur de la politique de l'eau, nous avons beaucoup consulté nous avons été à l'écoute, notamment des collectivités et la capacité d'intervention des agences de l'eau, principaux financeurs de la politique de l'eau aux côtés des collectivités est augmenté de 20%. Je crois qu'on peut souligner que c'est un effort inédit et qui s'était appelée des voeux de l'ensemble des acteurs. Ces moyens permettront d'accompagner les collectivités les plus en difficulté pour rénover et sécuriser les infrastructures d'eau potable. Le sujet a été largement évoquée. Aujourd'hui, nous allons changer d'échelle en matière de recycler, réutiliser des évolutions réglementaires ont été travailler pour libérer les projets, nous allons aussi soutenir les collectivités qui ont envie d'approfondir, justement le potentiel que pourraient représenter la réussite pour leur territoire comme je l'ai dit lors de notre débat et un partenariat avec l'année elle sera justement noué en ce sens la semaine dernière je remettez les trophées des aux commère. J'ai vu des projets très inspirant notamment sur la préservation de de l'eau des projets participatifs élaboré par et pour les citoyens. Ce sont de véritables pépites je crois fondamentalement aux initiatives de terrain et nous devons encourager. Tout cela pour ensuite les porter justement à l'échelle. Ce plan traduit une conviction commune la ressource en en haut en France et précieuse précieuse pour nos écosystèmes précieuse pour notre santé précieuse pour notre économie. Dans cet élan d'Europe repolitisation des enjeux de l'eau. J'attends aussi des élus locaux, une mobilisation pleine et entière en particulier sur les questions de partage de la ressource. Nous devons nous réunir autour d'une ambition forte pour porter des solutions d'adaptation dans nos territoires. Le 10 janvier dernier lors du 1er débat sur la ressource en eau. Nous avions eu ensemble. Je vous donner rendez-vous pour vous présenter plus en détail le plan eau et je vous remercie à nouveau de cette opportunité qui m'a été faite aujourd'hui pour vous présenter les mesures les plus structurante pour les collectivités et j'aurais plaisir à poursuivre ces échanges individuellement évidemment ou à l'occasion d'autres débats que je suis certaine qu'ils seront tenus au sein de de cette chambre. Merci à tous. Merci, madame la Ministre. Pour conclure le débat. La parole est à monsieur Mathieu Darnaud, président de la délégation. Sénatoriale à la prospective. Merci madame la présidente. Madame la Ministre je veux à mon tour saluer l'excellence du travail de nos 4 rapporteur et de la délégation qui a pu mettre justement en lumière les défis qui sont devant nous et qui nous attendent. Jamais je crois un exercice de prospective. N'aura autant collé avec une réalité que les uns et les autres vous êtes. Concentré. Essayer à à dépeindre la première chose que je souhaitais vous dire c'est que, à l'aune des hein différentes interventions c'est qu'il ne faudrait pas, selon moi, tomber dans une opposition entre le nécessaire effort. De sobriété et la mobilisation de la ressource, la sobriété je réponds cela notre collègue brouillé, on peut y travailler d'ores et déjà nul besoin de renvoyer à des travaux à des conventions et le département que je. Représente ici l'Ardèche avec l'établissement public de bassin a produit un document qui s'appelle Ardèche 2050 et qui est exemplaire sur le plan de la sobriété qui a mis tous les acteurs autour de la table et qui. Permet d'ores et déjà d'avancer sur ce sujet, y compris dans la dimension pédagogique. Mais nous avons besoin de mobiliser la ressource. Vous demandiez tout à l'heure madame la Ministre, pourquoi nous n'allons pas suffisamment vite sur la réutilisation. Des eaux usées traitées, je vous invite tout simplement à prendre angle et la tâche du président de l'Association des maires de France David Lisnard que vous avez. Cité tout à l'heure et qui se désespère parce que depuis 10 ans sur sa commune, il essaie de mettre en place un projet de cette envergure qui n'aboutit pas, on le sait, pour des raisons qui sont essentiellement administrative. Beaucoup ont ici parler de la question du stockage des réserves collinaires là aussi je veux porter témoignage dans mon département, les projets se succèdent pour répondre aux problématiques de notre agriculture du tourisme pour répondre aux problématiques de la défense incendie pour tout ce qui permet de répondre au sujet de de notre territoire. Nous avons multiplié les études environnementales, nous sommes appliqué à être le plus vertueux. L'État a signé des conventions avec la chambre d'agriculture avec le département aujourd'hui, aucun projet ne sort. Voilà la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui Je le dis réalité. Un mot sur le plan au oui, nous avons heureusement d'ailleurs des convergences sur certains points qui figure d'ailleurs dans. Le rapport de la délégation. Nous vous remercions de de l'avoir souligné mais le bât blesse. Sur le volet financier, je le dis très directement. On a salué le fait vous-même d'avoir. Demain la possibilité d'injecter 475 millions d'euros. Mais c'est oublier au passage que depuis plusieurs années. Nos agences de l'eau se voit dans l'obligation de restituer 400 millions d'euros pour financer l'Office français de la biodiversité. Donc quand vous faites l'addition et la soustraction, il reste peu d'argent pour porter et répondre aux défis qui sont devant nous et je le dis avec un. Parce que je crois que si on n'a pas compris l'enjeu financier qu'il y a. Pour pouvoir prendre à bras le corps. L'ensemble de ces sujets. Alors nous n'y arriverons pas. Vous avez évoqué l'enveloppe sur les réseaux fuyards très bien mais aujourd'hui. Je prends quelques exemples, le préfet de mon département vient d'interdire la délivrance à 26 communes de permis de construire pour que celles-ci puissent se conformer à des obligations en matière de réseau. C'est oublier que aujourd'hui sur ces communes l'Agence de l'eau n'a pas. Pu soutenir financièrement la la mise en place de schémas directeurs renvoyant aux finances des départements. Donc il y a la oui. Une avancée mais qui à mon avis est largement insuffisante pour pouvoir être au rendez-vous. Des efforts qui sont devant nous beaucoup de choses ont été dites, qu'il me soit permis de finir sur la question de la gouvernance. Oui il faut une gouvernance territorialisée. Oui, il faut vraiment parler et sollicité l'ensemble pardon des des élus de nos territoires pour venir autour de la table, discuter et faire avancer. Tous ces sujets, mais je crois aussi qu'il y a besoin d'agilité et je n'ai toujours pas compris après une question d'actualité au gouvernement après que vous nous ayez. Suite à l'intervention de notre collègue Joyandet. Comment vous voyez voyez l'avenir de la gouvernance sur nos territoires. Par rapport à une gouvernance qui soit intercommunal qui passe par le biais des syndicats ou d'une forme de mutualisation là encore je crois qu'il faut être clair vis-à-vis de celles et ceux qui doivent être. Les pionniers en matière de gouvernance de l'eau, c'est-à-dire l'ensemble des élus de nos territoires. Il faut leur faire confiance, il faut redonner un caractère facultatif, notamment pour permettre à des syndicats de porter ce sujet des syndicats qui revenons-en à l'essentiel, madame la Ministre épouse ces bassins versants qui finalement préfigure la gestion de la politique de l'eau sur notre territoire. Alors nous avons entendu les objectifs qui sont les vôtres. Nous sommes prêts à en débattre, nous sommes prêts à avancer car aujourd'hui le temps est venu de l'action. Je vous remercie.

La séance est reprise l'ordre du jour appelle le débat sur le thème harcèlement scolaire qu'est le plan d'action pour des résultats concrets à la demande du groupe Les Républicains. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit d'répartis pour une minute. Monsieur le Ministre, d'abord bonjour. Vous pourrez donc si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle la parole et tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat madame Alexandra Borchio-Fontimp pour le groupe. Les républicains et vous avez 8 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Harcelé. Tu. 2 verbes côte à côte pour désigner ce phénomène dramatique qui traduit un mal français, un laxisme sans précédent face à un fléau de société qui tue. Le harcèlement, mes chers collègues touche en France un million de jeunes, chaque année, c'est-à-dire un jeune sur 10 qui sont autant de citoyens. Dès la socialisation né le rejet. Et c'est lorsque l'enfant apprend à grandir à l'école primaire dans sa fragilité qui l'est davantage concernée à l'âge de ses premiers apprentissages. Le harcèlement scolaire concerne également leurs familles, leurs proches leur entourage, autrement dit au sein de notre assemblée, par exemple, ici et maintenant. Des dizaines de nos enfants ou de nos petits enfants subissent ce qu'aucun enfant ne devrait subir. C'est la raison pour laquelle notre groupe politique Les Républicains a souhaité inscrire ce débat à l'ordre du jour. Dès le plus jeune âge, un nombre de plus en plus conséquent de mineurs est amené à connaître de la cruauté humaine et à perdre foi en autrui ce lien de confiance pourtant fondamental dans l'épanouissement d'un individu. Une réalité qui dépasse souvent l'entendement une réalité trop régulièrement traité comme un simple fait divers mais chaque prénom de victimes leur histoire, leur souffrance et leur douleur. Nous ne pouvons les oublier. Suicide ou homicide. On ne s'est finalement jamais vraiment qualifié, comment qualifier l'acte d'un enfant qui se donne la mort car poussés à bout par leurs camarades. Que ce soit dans le cadre éducatif ou par le biais des nouvelles technologies ou des réseaux sociaux. Pourtant, le camarade à l'origine est un terme militaire qui renvoie au partage et à la fraternité. Il n'est de camarades que s'ils s'unissent dans la même cordée disait Saint-Exupéry, l'école et ce lieu où la société a décidé de confier à des adultes. La transmission des valeurs de savoirs de savoir-vivre et de savoir-faire à ses enfants. C'est là que la société dessine son avenir en formant les adultes de demain. Aller à l'école ne doit jamais devenir une contrainte émotionnelle mortifère qui ne laissera que des séquelles, voire des stigmates chez ceux qui ont été victimes de harcèlement ce débat et donc l'opportunité de poser des mots sur des incompréhensions que victimes par an mais aussi une forte majorité de nos concitoyens ne peuvent plus supporter. Et il est donc urgent de tout mettre en oeuvre pour remédier à cela. Comment ne pas être choqué lorsque l'on sait que l'enfant harcelé et donc brisé dans sa construction identitaire doit quitter son école tandis que celui qui a fait du mal peut y rester impunément. C'est ce qu'a conduit notre collègue Marie merci a déposé une proposition de loi visant à poser le principe d'une mesure d'éloignement du harceleur pour protéger la victime afin qu'elles ne subissent pas cette double peine. Une mesure de bon sens, Monsieur le Ministre, puisque vous l'avez retenu, si l'on en croit vos annonces dans la presse ce matin. L'impunité dans laquelle vivent les auteurs des faits de harcèlement doit cesser impunité qui les mène à reproduire leurs actes de victimes en victime à ne pas comprendre et mesurer l'impact et la gravité de leurs agissements. Il faut donc les prendre en charge de manière appropriée et n'oublions pas les témoins qui peuvent être traumatisés par la violence qu'ils ont observé et peuvent développer un sentiment d'impuissance. L'école a bien évidemment un rôle à jouer dans la lutte contre le harcèlement mais c'est avant tout l'éducation qu'on donne à son enfant qui va déterminer la personne qu'il sera envers les autres. Ne nions pas cet élément sans qu'il ne soit toutefois fait de faux procès en accusation aux parents afin que l'état des lieux dressé ne soit pas une équation dont il manquerait une inconnue. Les parents doivent également être impliqués dans la prévention en des temps sensibiliser et informer sur les différentes formes de harcèlement scolaire et en étant encouragés à Dia gauler avec à dialoguer avec leurs enfants. J'ai l'espoir que chacune des 17, prise de parole au sein de cet hémicycle aujourd'hui favorise le déclic afin que nous parvenons enfin à protéger nos enfants harcelés. Au Sénat, la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement estime qu'il est temps de détecter et traiter ce fléau autour de ce qui doit constituer désormais une grande cause nationale et non pas une journée nationale instauré un jeudi de novembre comme un rappel annuel où chacun dénonce le harcèlement scolaire, 24h durant, avec tout le pathos. Ce que l'on connaît. Faisons-le pour les parents de Lucas dans les Vosges. Ou encore pour la famille d'ombre dans la Drôme. Pas pour leurs propres enfants puisque c'est déjà trop tard. Ils ont préféré mettre fin à leur calvaire en se donnant la mort parce que notre pays n'a pas su les écouter. Ni les protéger. Nous devons donc aller plus loin dans la prévention et la formation auprès des acteurs de l'éducation nationale et des familles. Malgré les avancées de la loi du 2 mars 2022 et du programme phare de tels drames. En 2023, traduisent un terrible échec collectif. Une injustice inacceptable. Les chiffres montrent que ces mesures sont insuffisantes et relance les défaillances du système. L'autorité judiciaire doit faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité de sa politique pénale afin de se saisir de la nouvelle infraction définie les signalements doivent être pris au sérieux le harcèlement scolaire ne doit plus être considéré comme une histoire entre gamins qui a d'agrandir ou des jeux d'enfants sans importance à Menton dans mon département des Alpes Maritimes. Anna, je cite, n'en peut plus d'aller au collège chaque matin avec la boule au ventre et ça fait 6 mois que ça dure ce combat ne se mène pas seule. Il est temps que nous prenions tous ensemble des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre le harcèlement scolaire. Mais il est primordial de lever le voile sur ce phénomène et d'oser en parler car on a beau mettre en place tout un arsenal de mesures. Si les gens ne veulent pas voir alors tout cela ne servira à rien. Et dont les à détecter les victimes les prendre en charge et gérer les harceleurs. L'école est aussi ce lieu privilégié d'observation de repérage d'évaluation des difficultés scolaires personnel sociale familiale et de santé des élèves. Enfin pour conclure je veux saluer toutes les personnes qui s'engagent au quotidien dans la lutte contre ce fléau. Leur engagement est essentielle pour que nous puissions avancer ensemble dans la bonne direction avec, comme seul et unique objectif, l'intérêt de l'enfant pour que l'école ne soit plus une zone de non- de non- droit et pour que l'enfance ne rime plus jamais avec violence. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Borchio-Fontimp. Vous avez souhaité inscrire à l'ordre du jour, un débat sur le harcèlement scolaire, et je vous en remercie car j'ai placé la lutte contre le harcèlement scolaire comme une priorité de mon action indispensable à la réussite scolaire. Longtemps dans l'angle mort du système scolaire, il faut bien le reconnaître, la lutte contre le harcèlement scolaire, et depuis 2017, un enjeu fort du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui se mobilise très fortement et je m'inscris dans la continuité de l'action qui a été engagé. Vous je rappelle bien sûr la loi du 26 juillet 2019. Dite loi sur l'école de la confiance qui inscrit le droit à une scolarité sans harcèlement, la loi du 2 mars 2022 qui pénalise. Le fait de harceler et puis à la rentrée dernière, la généralisation du programme phare dont nous aurons l'occasion de reparler. Qui permet une mobilisation des communautés scolaires. Nous en sommes. C'est un chiffre que je vous donne à 60% des écoles qui sont engagés dans ce programme et 86% des collèges, ça n'est pas encore. 100%. Nous avons encore évidemment du chemin à parcourir. Nous avons aussi du chemin à parcourir. Du côté des lycées puisque j'ai annoncé que de. Du côté des lycées le programme phare sera étendue à partir de la rentrée 2022, nous avons beaucoup à faire. À tous égards et dans les échanges que nous allons avoir, j'aurai l'occasion de préciser un certain nombre de mesures. L'extension du programme phare, je l'ai dit et puis par ailleurs je l'ai annoncé également ce matin dans certains cas et en dernier recours la possibilité de scolariser l'élève harceleur dans un autre établissement pour ce qui concerne les établissements du 1er degré. Nous aurons l'occasion d'y revenir, je vous remercie. La parole est à présent à notre collègue monsieur Alain. Du groupe les indépendants et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Chaque année ce sont près d'un million d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Personne ne n'est épargné. Si chaque situation de harcèlement est unique. Les conséquences sont nombreuses et se ressemblent. Baisse de l'estime de soi isolement progressif des camarades, troubles du sommeil défiance envers les adultes décrochage scolaire honte et culpabilité si chaque situation de harcèlement est un drame. Il arrive même bien trop souvent que les cas de harcèlement vire à la tragédie. L'actualité se charge de nous le rappeler cruellement. On compte environ 20 suicides d'enfants par an. J'ai bien entendu une pensée pour le jeune cas décédé le 7 janvier dernier. La récurrence de ces drames souligne notre échec collectif à enrayer définitivement le fléau du harcèlement à l'école. Aujourd'hui, la situation se complique, car les frontières entre le cadre scolaire et la sphère familiale privée se brouille. avec l'avènement des réseaux sociaux, les jeunes victimes non plus un instant de répit. Le harcèlement vécu en classe se poursuit à la maison jusque dans la chambre, censée être le refuge intime et protecteur par excellence, les moqueries, les humiliations, les insultes continuent à pleuvoir. Par message privé ou bien à la vue de tous dans des publications, devenant parfois virale la peur doit changer de camp. C'était justement le signal envoyé par la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement en juin 21 dans ma collègue Colette Mélot était la rapporteure. Et dans notre collègue Alexandra suis au monde. Il vient de rappeler les principaux éléments. Le constat est sans appel, aucun établissement scolaire aucun département n'est épargné. On estime aujourd'hui entre 800.000 et un million le nombre d'enfants victimes de harcèlement scolaire chaque année. Cela représente un enfant sur 10. Ces chiffres sont effrayants et nous engage à réagir urgemment. Ce rapport a présenté une série de pistes d'actions concrètes. Elle s'organise autour de 3 axes clairs destiné à guider l'action publique, la prévention, la détection précoce, il y a enfin le traitement des cas de harcèlement. Le rapport, insisté notamment sur la gravité du cyber harcèlement face auquel les parents et le personnel éducatif reste bien souvent démunis, la prévention des jeunes est cruciale, la formation des adultes et essentiel. Nous devons développer collectivement de nouveaux réflexes de protection pour intervenir dès l'apparition des premiers signaux d'isolement ou de persécution. C'est d'autant plus important à l'école républicaine. Elle doit être un lieu d'épanouissement et d'apprentissage pour nos jeunes et non le théâtre de brimades, d'humiliations et de violence physique ou verbale. Tout le monde doit se mobiliser, éducateurs, parents, enfants, pouvoirs publics, l'État joue un rôle essentiel pour impulser une vaste stratégie de lutte contre ces violences dont souffrent nos jeunes aux à l'école. Nous devons tous être au rendez-vous. Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous énoncé avec précision vos ambitions et votre calendrier pour lutter avec efficacité contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre pour répliquer. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Marc. Je vous remercie de vos propos et nous sommes évidemment en accord sur la gravité des conséquences du harcèlement. Vous avez rappelé les drames que nous avons connu et j'ai une pensée bien sûr pour les victimes. Que ce soit les élèves qui meurent chaque année de harcèlement ou que ce soit les élèves qui plus silencieusement je dirais sont affectés sur le long terme par des des pressions ou par des trajectoires scolaires enrayer. La question du cyber harcèlement est évidemment très importante. Je rejoins les propos que vous avez tenus. Je rappelle à cet égard, l'existence d'un numéro le 30 18, numéro gratuit, qui est très efficace, j'ai visité la plateforme. Qui permet de répondre y compris à des messages de de panique. De collégiens ou de leur famille lorsqu'il s'agit de bloquer telle ou telle photographies intimes ou telle ou telle boucle de messages on y arrive très bien et je veux saluer évidemment l'existence de ces deux numéros, dont je signale qu'ils seront désormais systématiquement présents dans les carnets de correspondance des élèves à partir de la rentrée, le programme phare auquel vous avez indirectement fait allusion à donner ses preuves ou a fait ses preuves dans les 6 académies où il était expérimenté jusqu'à l'année dernière. Il est donc généraliser à partir de la rentrée dans les proportions que j'ai indiqué, nous avons encore du chemin à faire. De quoi s'agit-il. Il s'agit d'abord de former au moins cinq adultes référents par établissement scolaire plus des élèves ambassadeurs ce sont souvent les élèves qui sont à même de détecter. Les changements de comportement, de leurs camarades ou telle ou telle situation de harcèlement et de rapporter les faits auprès des adultes formés. Nous sommes en en dans un vaste programme de formation des adultes et puis ensuite il y a le traitement des situations de harcèlement. Où l'on essaye puisque ce sont des enfants et que nous avons une mission pédagogique de. D'amener le l'élève harceleur à reconnaître ses torts et enfin la possibilité de sanctions, que ce soit par le biais de conseils de discipline où que ce soit par la nouvelle disposition que j'ai indiqué un instant. Madame la présidente, monsieur Ministre, mes chers collègues, je vais commencer par une petite digression puisque nous allons passer le reste de la journée à parler de l'école et de ce qui l'entoure et alors que nous aimerions qu'elle soit un sanctuaire préservé des violences de notre société la semaine dernière, ce sont les violences policières qui se sont invités dans un lycée. De Conflans Conflans-Sainte-Honorine où un élève a été plaqué au sol par 4 policiers, menotté, emmené au commissariat relâché sans poursuites pendant que d'autres élèves étaient menacés par des agents les visant avec des flash ball. Nous aurions aimé Monsieur le Ministre, une réaction de votre part devant cet usage manifestement disproportionné de la force. Mais revenons au débat du jour, et nous sommes aujourd'hui une nouvelle fois réunis pour débattre d'un fléau national le harcèlement scolaire. Ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, mais il convient comme à chaque fois de faire état des chiffres pour bien mesurer l'ampleur du phénomène. D'après le rapport de la mission d'information porté par nos collègues la sénatrice Colette Mélot et Sabine bande Egg, la situation est absolument dramatique, entre 800.000 et un million d'enfants en sont victimes chaque année, ce qui représente 2 à 3 élèves par classe, et 6 à 10% des élèves ils font face au moins une fois durant leur scolarité. en fait une menace et une souffrance particulièrement difficile à vivre et à cerner, c'est qu'elle ne se cantonne pas aux enceintes des écoles le harcèlement rattrape les élèves jusque dans leurs foyers via les réseaux sociaux et toute la sphère numérique. Le cycle des violences ne s'arrête jamais. Les victimes ne connaissent aucune pose aucun répit dans leur souffrance et cela échappe à la sphère parentale, tout en se passant parfois au domicile. Il convient de s'attaquer aux causes de nombreux élèves sont harcelés en raison de leur genre de leur handicap de leur couleur de peau ou de leur orientation sexuelle et les conséquences sont parfois terribles définitive en janvier dernier, le suicide de Lucas, 13 ans, harcelée, en raison de son homosexualité montre à quel point l'homophobie et la discrimination continue de tuer. À la rentrée 2022, le programme de lutte contre le harcèlement scolaire phare qui prévoit notamment aux différentes actions de prévention, vous l'avez dit, a été généralisé à l'ensemble des écoles élémentaires et des collèges. vous venez de le réaffirmer que ce programme avait obtenu d'excellents résultats, nous aimerions vous croire sur parole mais nous avons un problème en ce moment avec la sincérité de la parole de l'ensemble du gouvernement. Sur quels critères. Sur quels éléments vous basez-vous alors que le programme phare prévoit un mécanisme d'évaluation aucune évaluation détaillée n'a jamais été communiquées publiquement de leur côté, plusieurs associations et syndicats pointent du doigt de nombreux dysfonctionnements, notamment le déploiement inégal du programme sur le territoire, la formation superficielles, l'absence de communication sur le numéro d'urgence le manque cruel de moyens humains et financiers. Le collège du jeune Lucas qui s'est ôté la vie avait d'ailleurs mis en place ce dispositif au sein de son établissement en vain le manque de moyens humains et financiers dédiés à la lutte contre le harcèlement scolaire va au-delà du programme phare, prenons l'exemple de la médecine scolaire j'alertait déjà sur ce point l'année dernière au moment de l'examen de la proposition de loi sur le harcèlement scolaire. L'état de la médecine scolaire dans notre pays est un scandale il y a environ 900 médecins scolaires et 7700 infirmiers et infirmières scolaires pour 12,5 millions d'élèves dans notre pays soit un médecin pour 14.000 élèves et un infirmier ou infirmière pour 1600 élèves, cela représente une chute des effectifs de 15% en 5 ans, la pandémie n'a, n'a pas été un déclic. Le quoi qu'il en coûte s'est arrêté à la porte de l'école. Voilà des professionnels au contact des élèves qui pourrait identifier des situations à risque, engager le dialogue est alerté, mais avec les moyens humains aussi dérisoire il nous est impossible de leur confier ces missions. Enfin vous avez récemment annoncé monsieur Ministre plusieurs mesures contre le LGBT phobies à l'école comme le déploiement de campagnes de sensibilisation et la généralisation d'observatoires, de lutte contre les LGBT phobies. C'est une première étape, que je salue, mais qui est loin d'être suffisante pour endiguer le débat le dès le fléau des discriminations LGBT fort à l'école. Je m'interroge également quant aux moyens qui seront dédiés à ces dispositifs et leur pérennité. lutter efficacement contre le harcèlement scolaire LGBT phobies. Si les moyens mis en place ne sont pas à la hauteur des enjeux, nous le savons, il n'y a pas de solution simple pour lutter contre le fléau protéiforme du harcèlement scolaire. Nous avons bien conscience que les solutions sont multiples et au croisement de l'école et de la société qui l'entoure. Mais il faut passer à la vitesse supérieure. Investir plus dans la lutte contre le harcèlement scolaire, que ce soit à travers la médecine scolaire ou des politiques de prévention contre la montée des haines, c'est investir dans l'apaisement de l'école et de la société en général. Il en va de notre responsabilité. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, vous avez 2 minutes pour répliquer. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur de Vous avez raison, ça n'est pas le 1er débat qui se tient dans cet hémicycle sur la question du harcèlement mais nous avançons et comme vous l'avez dit à l'instant, il n'y a pas de solution simple. Nous sommes sur un chemin un chemin de progrès mais il n'y aura pas de baguette magique qui d'un seul coup fera disparaître ce fléau. Vous avez justement dit que souvent le harcèlement pèse sur un élève ayant une vulnérabilité réelle ou supposée une différence réelle ou supposée. Le cas des élèves LGBT est un bon exemple. Nous avons eu des drames terribles. Il y a quelques semaines et je suis très mobilisée sur cette question, nous préparons activement la journée internationale du 17 mai, ce sera l'occasion d'une grande campagne vous avez mentionné la création des observatoires notre partenariat avec l'association SOS homophobie et d'autres associations qui sont très mobilisés sur la question, vous avez posé la question des évaluations en. De l'évaluation des expérimentations qui ont eu lieu dans 6 académies pendant 2 années Ces expérimentations sont en évaluation. Il y a une équipe de chercheurs qui travaillent sur la question. On sait déjà de manière empirique que le règlement des cas. De harcèlement a donné de bons résultats pas tellement la baisse du nombre de cas puisque précisément le fait de se mobiliser, fait que ça fait apparaître des cas qui sinon resteraient sous la ligne de flottaison. Nous sommes mobilisés, y compris via la médecine scolaire le point que vous indiquez sur la médecine scolaire est intéressant parce que un bon tiers des postes de de médecine scolaire ne sont pas pourvus. Je pourrais nous pourrions doubler le nombre de postes de médecine scolaire que ça ne changerait rien au nombre de médecins. C'est pourquoi nous préparons activement avec le ministre de la Santé. Un plan de médecine scolaire. Nous attendons pour cela. Le rapport qui viendra deux 3 inspections générales qui sera l'occasion de mettre à plat cette question importante. Merci, monsieur le Ministre. La parole est à présent monsieur Julien Bargeton ton du groupe RDPI et vous avez six minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. De quoi parle-t-on. Du harcèlement et essentiellement en fait du harcèlement entre pairs, puisque c'est la forme la plus répandue de la violence en milieu scolaire qui est caractérisé par un usage répété de la violence physique des moqueries des insultes ou des humiliations. Cela concerne et cela a été rappelé à peu près 800.000 à 1 million d'élèves par an, soit potentiellement 10% des élèves qui sont concernés et avec les 20. L'avènement du numérique, hé bien ce cet harcèlement se prolonge via les réseaux sociaux et y compris la sphère privée n'y échappe plus. Alors depuis 2017. Le gouvernement les gouvernement a pris. Vraiment la mesure de cette difficulté de ses graves difficultés qui d'ailleurs se sont marqués par un drame récent que vous avez tous ceux cités avec le jeune Lucas. Depuis 2018, je vous rappelle que les portables sont interdits à l'école et au collège avec une proposition de notre collègue Richard Ferrand d'ailleurs qui avait été adopté en procédure accélérée et c'est évidemment une forte une forte. Lutte contre le cyberharcèlement que bien sûr de lutter contre l'utilisation trop précoce et trop massive de ce genre d'instrument par nos enfants cet cet élément-là été le premier est extrêmement important en 2019 la loi pour l'école de la confiance est venu en effet créé ce droit à une scolarité sans harcèlement, aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. La même année, le gouvernement a annoncé l'extension des horaires de la plateforme net écoute dédié au cyber, harcèlement. Le plan de lutte contre le harcèlement phare a été souvent cité par les orateurs précédents et par vous Monsieur le le ministre il est désormais obligatoire dans tous les collèges et toutes les écoles élémentaires. Depuis la rentrée 2022. Il implique à la fois les adultes et puis les enfants notamment avec les élèves ambassadeurs ainsi que les parents qui sont associés. C'est donc un dispositif 360 degrés qui concerne toute la communauté éducative. L'année dernière la proposition de loi de notre collègue Erwan Balanant a créé un nouveau délit de harcèlement scolaire qui sanctionne des élèves ont aussi les étudiants ou les personnels des établissements scolaires et universitaires qui sont reconnus coupables de harcèlement. C'est désormais passible de 10 ans de prison et de 150.000 euros d'amende en cas de suicides ou de tentatives de suicide de la victime du harcèlement. Il y a donc une panoplie pour lutter contre le harcèlement et qui a été complété ces dernières années, depuis 2017 et bien sûr cela paraît insuffisant parce que la situation est toujours dramatique et ces phénomènes ne sont pas encore trop répétitif et donc effectivement d'autres d'autres changements sont vraisemblablement nécessaire. Alors il y a une proposition de loi, une proposition de loi de notre collègue. LR Marie Mercier qui qui pose le principe de la mesure d'éloignement du harceleur pour protéger la victime. C'est une question importante. L'éloignement systématique qui doit-il concerné. Est-ce que c'est pas une double peine s'il concerne aussi la personne l'enfant qui a été. Victime il y a eu aussi une proposition de loi de notre collègue Sabine von on voit donc que le Parlement se saisit dit largement Monsieur le Ministre. Vous avez apporté des éléments de réponse. D'ailleurs ce matin peut-être souhaiterez-vous les compléter lors de ce débat. En matière d'avancer sur la façon dont sont traitées les auteurs de harcèlement dans les établissements scolaires et puis peut-être qu'il faudrait se pencher sur des méthodes complémentaires, certains pays sont en avance sur ces sujets, je pense aux pays scandinaves qui ont souvent un temps d'avance. Sur ces considérations, ils les ont pris à bras le corps, depuis longtemps, notamment des méthodes comme la préoccupation partagée ou encore le programme finlandais, un programme qui s'appelle qui va couler. Qui est mis en place en 2006. Depuis 2006 donc ça fait longtemps et qui était organisé autour de discussions systématique de jeux de rôle il y a une systématisation de la lutte contre le harcèlement scolaire dans tous les établissements finlandais. Il serait aussi bien de faire un peu de parangonnage pour voir en Europe notamment comment ont pu avancer d'autres pays, on le voit, donc nous avons beaucoup avancé sur la question du harcèlement. Les faits reste encore trop grave et trop nombreux et je ne doute pas qu'ensemble nous construirons des nouveaux outils des nouvelles armes pour lutter contre ce fléau. Merci beaucoup. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre pour répliquer. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur sénateur Bargeton. En effet, le programme phare que dont nous parlons. À une inspiration qui êtes qui est finlandaise et lorsque j'ai évoqué. Les la mesure et l'évaluation de ce. Programme. J'aurais du mentionner le cas de la Finlande, où il a donné de, de bons résultats. Je, j'attire votre attention sur le fait que ce programme a une dimension pédagogique et il ne vise pas d'emblée à à sanctionner. Il vise plutôt à mener le le le harceleur l'enfant harceleur à à reconnaître la gravité de ses actes et à participer par la suite d'une mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative à l'égard des faits de harcèlement et en effet, parfois on a d'anciens harceleurs qui sont. Au 1er rang en quelque sorte des élèves ambassadeurs pour se mobiliser contre les situations de harcèlement et en ce sens l'école maintient bien sa mission première qui est une mission pédagogique mais il faut reconnaître parfois que. La dimension pédagogique ne suffit pas que la situation peut être si dégradé entre des harceleurs ou un harceleur et puis les élèves harcelés que la séparation entre les élèves devient la solution ultime. Cela est possible dans le secondaire. Bien sûr puisque les conseils de discipline peuvent. Scolarisé un élève en dans un autre établissement que celui d'origine, cela n'était pas possible et n'est pas possible dans le primaire, puisqu'il n'y a pas de conseils de discipline. C'est pourquoi nous proposons de passer par une voie réglementaire et non pas par une voie. Législative par la voix de la loi. De manière à dans certains cas et en dernier recours été. Toutes les solutions ont été envisagées. De déplacer l'élève par. Indépendamment de l'avis des représentants légaux et. Selon. Une procédure que je détaillerai si la question m'est posée. Je vous remercie. La parole est à présent madame Sabine et que pour le groupe socialiste et vous avez 3 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cela a été dit, près d'un million d'élèves subissent chaque année une forme de harcèlement durant leur scolarité. D'une violence parfois telles qu'elles poussent certains enfants à attenter à leurs jours. Il est intolérable. Monsieur le Ministre, que les fondements du vivre ensemble soit ainsi et que les jeunes soient éprouvé à l'âge où ils font leurs premiers apprentissages dévoilant leur fragilité propre à l'adolescence. Bien sûr il ne s'agit pas de dire ici que rien ne se fait au sein de l'Éducation nationale. Même si le programme phare s'est généralisé à la rentrée 21, nous devons encore constater la difficulté à franchir le mur de l'administration scolaire et la tentation du pas de vagues au sein de certains établissements. La lutte contre le harcèlement scolaire. Passe aussi par les initiatives locales, associatives ou institutionnel dans mon département du Pas-de-Calais par exemple j'ai animé avec les services de l'État, de la police de la gendarmerie de la justice, de l'éducation nationale Une réunion visant à améliorer l'accueil, la protection, le suivi des élèves victime de harcèlement scolaire ainsi que la prise en charge des auteurs de ces faits délictueux. Je me réjouis de la mobilisation de tous ces acteurs, bien sûr, mais cela reste encore insuffisant et la question du harcèlement scolaire révèle encore de grandes failles qui doivent être comblées. Je viens donc de déposer, avec mes collègues sénateurs socialistes, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement afin de compléter l'arsenal juridique existant notre PPL se veut pragmatique simple et concrète. Elle prévoit notamment d'imposer aux réseaux sociaux une nouvelle obligation de sensibilisation des usagers de renforcer le poids des adultes correctement formés sur le sujet au sein de l'école et que les auteurs puissent puissent être exclue au lieu de la double peine qui s'impose aux victimes forcés de quitter leur établissement pour échapper à leurs bourreaux et je me félicite Monsieur le Ministre, que vous ayez d'ores et déjà repris cette disposition très importante. En tout état de cause la clé de tout, c'est l'augmentation du nombre d'adultes effectivement présents dans les établissements comme le réclament les sénateurs de notre groupe à chaque discussion budgétaire depuis maintenant 6 ans, il est impératif. Monsieur le Ministre, d'augmenter les postes de personnels médicaux sociaux de psychologues dans les établissements scolaires personnel qui joue un rôle essentiel dans la prévention, la détection et la prise en charge des cas de harcèlement. Pour que la parole des enfants, des adolescents se libèrent ceux-ci doivent se sentir écouté compris protéger c'est par la présence suffisante de personnes formées et à l'écoute que nous pourrons espérer le fléchissement de ce fléau insupportable. Merci. Monsieur le Ministre pour réponse pour 2 minutes. Merci madame la. Présidente madame la sénatrice. Vent. Je vous remercie d'abord pour le rapport et votre travail sur le sujet que vous avez réalisé avec madame la sénatrice. Mollo. Je note au passage que votre proposition de diffuser au mieux les numéros 30, 18 et 30 20 que nous avons repris cette proposition lorsqu'elle sera inscrite dans les carnets de correspondance et surtout les environnements numériques de travail il y a une campagne d'affiches qui qui sont déjà réalisés et que j'ai pu voir presque systématiquement sur dans les couloirs des des établissements scolaires. On n'est plus à l'époque du pas de vagues. À l'évidence, nous sommes très mobilisés sur cette question, on a passé un cap quand même depuis un certain temps, même s'il y a du travail à faire à propos du des élèves harceleurs que nous allons éloigner je veux ici remercier. La sénatrice Mercier de la proposition qu'elle a fait à propos des élèves harceleurs. Nous proposons donc de les éloigner indépendamment de l'avis des parents ou des représentations ou des représentants légaux lorsque la situation est devenue intenable ce que la sécurité. Des élèves harcelés en l'occurrence ou de l'élève harcelé et mise en cause. Cela suppose l'accord du maire de la commune, voire des 2 s'il y a. Une scolarisation dans une commune voisine. Il faut procéder avec avec discernement en la matière puisque nous avons affaire à des enfants des enfants entre 6. Et 11 ans, que parfois les situations entre harceleurs et harcelés ne sont pas si claires avec des échanges si j'ose dire entre la situation des uns et des autres mais il faut pouvoir envisager cette possibilité lorsque la situation est bloquée. D'où le sens de la proposition que j'ai fait. Merci, vous avez une minute pour répliquer, chers collègues. Oui vous avez raison il faut agir avec discernement monsieur le Ministre, mais il ne faut pas, disons, faciliter la vie. Au harceleur au détriment. Du harcelé. Merci la parole est à présent à madame Céline Brulin, du groupe communiste. Vous avez 5 minutes, chers collègues.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, le harcèlement. Le harcèlement scolaire est un fléau. Un élève sur 10 subit chaque année une forme de harcèlement ou de cyber harcèlement c'est un drame car il entraîne des enfants vers des actes extrêmes. Face à ces situations, nous ne sommes pas totalement démunis, même s'il n'existe pas de remède miracle. Le Sénat a ainsi fait 35 propositions dans le cadre d'une mission d'information qui a été rappelé tout à l'heure, la loi du 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire a également donné quelques outils il convient je crois. Grâce à ce débat et je remercie la collègue qui l'a initiée d'en faire un bilan afin de vérifier que les réponses en matière de prévention de détection de soutien aux victimes et à leurs familles sont opérant. La loi, inscrit dans le code de l'éducation, la lutte contre le harcèlement scolaire permettant de mieux appréhender de punir ce phénomène dans son article hein il est instauré une information sur les risques liés au harcèlement scolaire délivrées chaque année aux élèves et parents d'élèves comment cela se traduit-il dans les établissements scolaires. Avec quels moyens. Son article 7 prévoit également la remise d'un rapport relatif aux frais de consultation et de soins engagés par les victimes. Monsieur le Ministre, ce rapport a-t-il été produit. Pouvez-vous nous en donner les éléments ce texte prévoyait aussi la CDI sation des assistants d'éducation qui constitue un des rouages d'alerte et de prévention essentielle au sein des établissements. Le décret a tardé à être pris. Hé bien qu'il soit désormais pris certaines académies continue visiblement de ne pas appliquer cette disposition. Quand est-ce que cette mesure sera généralisé. J'aimerais également rappelé la conviction que j'ai plusieurs fois exprimé ici d'une revalorisation du statut des AESH qui leur garantirait entre autres une véritable formation initiale et continue notamment en matière de harcèlement, le handicap pouvant constituer un motif et j'mets évidemment beaucoup de guillemets autre avancée de cette loi, mais qui d'après les remontées de terrain, se révèlent encore insuffisantes, le renforcement de la formation et de la sensibilisation de l'ensemble des personnels éducatifs. Quel est le contenu de cette formation initiale. Qu'en est-il pour la formation continue, le programme phare qui a été évoqué à plusieurs reprises, a été généralisé, vous l'avez dit vous-même c'est une bonne chose sauf que en effet sa généralisation a été lancée avant même le retour d'expérience des 6 académies. Or leur expertise permettrait je crois d'améliorer ce programme. Je pense par exemple la constitution d'une équipe d'au moins 5 personnes par collège ou par circonscription pour le 1er degré en rappelant d'ailleurs que ce déploiement se fait à moyens constants. Alors que les personnels ont déjà de nombreuses missions et on pourrait même dire de plus en plus de missions à effectuer et que les suppressions de postes risque de fragiliser. Ce travail là aussi vous évoquez régulièrement la baisse démographique pour justifier ces suppressions de postes mais la France reste un mauvais élève au regard d'autres pays européens en matière de taux d'encadrement, que se passe-t-il quand un des membres de l'équipe n'est plus en poste, il faut alors recommencer tout le processus. Ce qui est dommageable. Même chose avec les 10h de formation pour tous et tous les élèves du CP à la 3ème qui les assurent comment et avec quels outils lors de votre audition dans le cadre de la préparation du PLF 2023 nous vous rappelions et cela a été fait aussi à l'instant la situation critique de la médecine scolaire qui est elle aussi un maillon essentiel de la lutte contre le harcèlement, c'est de notoriété plus que public, les effectifs ont fondu comme neige au soleil encore plus en milieu rural et nous manquons également de psychologues pour les Rased vous indiquiez lors de cette audition de voir rencontrer le ministre de la Santé pour envisager une autre structuration de la médecine scolaire et envisager des alternatives qui permettraient de répondre aux impératifs de médecine de prévention et de détection. Quelles sont ces alternatives, où en est-on aujourd'hui du travail que vous proposiez d'initiés. Enfin le harcèlement scolaire a changé de dimension avec le poids pris par les réseaux sociaux qui n'offrent effectivement aucun répit aux victimes les frontières de l'école sont maintenant largement dépassé. Et il me semble que les plateformes doivent davantage assumer leurs responsabilités. Pourquoi ne pas avoir retenu l'idée d'une contrainte pour les réseaux sociaux de présenter régulièrement des vidéos de de prévention et de sensibilisation au système Enfin, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit ce matin. Sur le fait que un enfant harceleur serait écarté. Plutôt que la victime qui jusqu'à présent l'était. Avez-vous consulté les associations d'élus, puisqu'en effet il faudrait l'accord du maire dans l'école d'accueil qu'il y a aussi, je suis désolé de de venir sur ce sujet trivial, mais des conséquences financières puisqu'il y a une participation. De la commune. Dont. L'habitant l'enfant habitant doit aller vers une autre école et je voudrais savoir si vous avez pris le soin de consulter les associations d'élus, sur ce point, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, vous avez 2 minutes. Merci madame la présidente, madame la sénatrice brûle hein vous avez. En effet fait allusion au programme phare et à la loi du 2 mars. 2022 2022 qui place la question de la formation en leur coeur et de fait nous avons. Intensifié les programmes de formation, d'abord en les systématisant. Au niveau des Inspé pour les professeurs stagiaires ou pour les CPE CPE stagiaire et puis nous avons organisé séminaires nationaux et avec des déclinaisons académique pour d'abord former les formateurs, si je puis dire, afin que les choses se diffuse ensuite au niveau des écoles et des établissements. C'est un processus lent parce qu'il y a beaucoup de monde a former sur le sujet. 5 personnes par établissement scolaire. Du côté du secondaire 5 personnes par circonscription. Du côté du primaire. C'est un travail que nous menons. Sur plusieurs années. En parallèle de cela il y a la sensibilisation des familles c'est aussi quelque chose d'important. Les familles ont un rôle à jouer et donc en début d'année scolaire. Nous insistons sur le fait que les écoles et les établissements doivent sensibiliser les familles connaître les numéros 30, 20 et 30 18 en particulier, vous avez fait allusion à la médecine scolaire, j'en ai parlé moi-même on attend le rapport des 3 inspections générales afin de faire des propositions et je serai heureux de venir en parler devant vous, si vous le souhaitez. Quant aux. Plateformes. Je suis en accord avec vous. Elles doivent être responsabilisés. C'est d'ailleurs. À une réflexion et c'est d'ailleurs une un échange que nous avons eu lors de la visite. Opéré sur la plateforme. 30 18. Pardon le temps mais je reviendrai sur. La question des mères et des harceleurs et harcelés je excusez-moi pour ce retard. Je vous en prie monsieur le Ministre. Vous souhaitez répliquer. La parole est donc à présent à monsieur Jean hein gré du groupe Union centriste et vous avez 8 minutes, chers collègues. Bien, madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La communauté éducative et démunie. Elle est démunie car elle est affaiblie par un phénomène incompris de tous, pourtant bien présent. Le harcèlement. Aujourd'hui le harcèlement scolaire fracture notre jeunesse en deuil nos familles et brise notre République. En s'attaquant notre République. Aussi dépassée que désarmer le harcèlement remet en question sa légitimité. Une légitimité, pourtant construite à travers les siècles de Napoléon à Jules Ferry en passant par Julie victoire Daubié l'école républicaine, de par sa capacité à s'adapter au aux circonstances parfois aux crises a toujours su aller de l'avant. Mais aujourd'hui cette légitimité et menacé menacé par la souffrance de millions d'élèves. Chers collègues, il est difficile de comprendre la nature humaine, la psychologie et les rapports de force qui s'opère entre les élèves. Nous observons avec tristesse et colère, les conséquences funestes de ces abus. Presque un million d'enfants un million d'enfants subissent du harcèlement scolaire en France en 2021, 22 enfants ont fait le choix de renoncer. De renoncer de la pire des manières vivant une souffrance insupportable. Il ne se sentait plus d'exister alors ils ont fait le choix de ne plus souffrir. Chers collègues, nous constatons avec regret la faible prise en charge de notre système éducatif à résoudre ce phénomène. Difficilement cernable. Le harcèlement prend plusieurs formes moral, physique sexuelle et n'oublions pas le racket. Le harcèlement d'une manière générale est un phénomène qui s'accroît et se complexifie avec les réseaux sociaux. Le semblant d'anonymat qui le permet. La tendance à suivre les effets de meute et la volonté de ses distincts du groupe font des réseaux sociaux le lieu propice et privilégié ou harcèlement. Le harcèlement scolaire est partout de l'école à la maison en passant par les transports en commun, 50% des collégiens se plaignent de la violence dans les transports, les effets de groupe ont longuement été étudié et font consensus dans la communauté scientifique. Il y a un leader des suiveurs des actifs et des passifs. Ce sont ces mêmes passif qui parfois se trouve au sein même du corps enseignant corps enseignant censé écouter et prendre des mesures qui finissent par ne pas agir ou agir trop tard. C'est l'un des principaux fléaux de notre système éducatif. Les victimes de harcèlement et leurs familles sont parfois confrontés à une parole qui est entendu, certes. Lorsqu'ils en ont la chance mais qui n'est pas toujours considéré, chers collègues. À quoi bon entendre lorsque nous refusons d'écouter. Il est difficile de reconnaître une situation, un élève est harcelé. Le harceleur agi de façon cachée et les formes que peut prendre le harcèlement sont souvent interprétés comme de simples chamailleries entre enfants. Les adultes ne s'attardent pas toujours ou pas assez sur certains phénomènes de micro-, violences, ils sont considérés comme banales voire normaux entre jeunes ou moins jeunes. Nous assistons à une perte de confiance de plus en plus grande entre les parents, les élèves et l'éducation nationale. Que dire des délais de traitement trop long au sein des établissements. Le délai doit donc être définitivement et clairement afin de ne pas laisser les familles et les victimes en suspens pendant des mois mois durant lesquels le harcèlement perdure ou s'intensifie. La prise en charge des signalements au sein des établissements restent floues. Les procédures de signalements ne sont pas harmonisées à certains égards, elles sont même inadapté. Je le répète, chers collègues, nous sommes en face n'a fait domaine profondément humain qui mérite une réponse de l'État. Pourtant, il faut reconnaître les avancées en la matière, l'éducation nationale s'est dotée de moyens considérables pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le programme phare a le mérite d'exister, il demeure insuffisant ce programme rend les élèves acteurs de la lutte contre le harcèlement sur la base du volontariat. Une procédure en apparence à monsieur le ministre, il y a 2 mois, je vous ai interpellé au sujet du suicide du petit Lucas suite à cette intervention de famille de famille de mon département dans les Vosges ont contacté pour faire part d'une faille notoire failles qui se transforme en cauchemar pour les victimes les élèves harceleurs animé par une soif de ne de domination intègre le programme phare. Pierre qui pour rappel est censé protéger les victimes, que se passe-t-il. Monsieur le Ministre. Il n'est plus question de prévention, il faut des réponses concrètes. Il est nécessaire de responsabiliser des établissements ou harcèlement. Nous devons faire de l'école un lieu de vivre ensemble exemplaire la prise en charge des victimes est fondamental prioritaire, il faut en même temps encadrer efficacement les harceleurs. De nombreuses méthodes existent pour prendre en charge efficacement le harcèlement je pense notamment à la méthode farce ta noble animal proche et puis casse. Monsieur le Ministre, j'ai cité quelques méthodes. Quelle est votre méthode. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, vous avez 2 minutes pour répliquer. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur engrais. Il y a 2 écueils au fond à éviter. Dire que rien ne change dans l'éducation nationale que. Ce dont on parle n'est que du vent ou à l'inverse, bien sûr, expliquer que le programme phare que les dispositions qui ont été prises ces dernières années aurait tout changé miraculeusement. Nous sommes sur un sur un chemin et je reconnais avec humilité. Devant vous mesdames et messieurs les sénateurs, que nous avons du travail à réaliser. Du travail à réaliser. Pour réduire. Ce phénomène catastrophique qu'est le harcèlement. 1er point la formation des. Enseignants et des adultes. Dans les établissements et dans les écoles c'est un point très important. Et comme je l'ai indiqué, ça prend du temps et bien entendu compte tenu de, de la masse. Des enseignants et des adultes. Mais j'observe tout de même qu'il y a une prise de conscience d'une manière générale dans les communautés éducatives. Prise de conscience qu'on observait pas de l'avis général, il y a quelques années, les délais de traitement sont peut être long, peut être trop long, méfions-nous, à l'inverse des procédures expéditives. Il y a en la matière possibilité par exemple pour les chefs d'établissement ou pour les Dasen de procéder à des mesures de sauvegarde des mesures par lesquelles on écarte. Temporairement. Un élève harceleur sans préjuger de la suite qui pourra être donnée à la procédure et puis je voudrais insister sur ce point, c'est que, en dépit de la démarche pédagogique qui est celle du programme phare et qui est essentiel. J'insiste là-dessus. Il faut également envisager des sanctions, les sanctions, ça fait partie de la pédagogie d'une manière générale, que ce soit par le biais des conseils de discipline où que ce soit par le biais. Du transfert de lève de l'élève harceleur. Dans le 1er degré suite à une procédure que nous voulons régler par la voie réglementaire. Merci, monsieur le Ministre, vous avez une minute pour répliquer chers collègues si vous le souhaitez. Oui merci madame la présidente, monsieur le le ministre-j'entends vos propos sur le travail que vous avez entamé, notamment avec les préconisations. Du Sénat c'est un travail qui sera long, vous venez de le dire. Suite à l'interpellation que vous avez fait sur le suicide du petit Lucas de familles qui sont venus me voir dans le département des Vosges là Dasen à nous a aidé à aider les les familles comme vous venez de le, de le dire, je pense que cette sensibilisation cette prise de conscience de la part des familles. Suite au travail que nous faisons de manière collective doit doit aider mais si vous voulez, moi je suis toujours quand même étonnée qu'on qu'on puisse venir voir un parlementaire pour des problèmes internes à l'éducation nationale, c'est ça qui m'a un peu choquée depuis la la question que vous avez posée concernant le suicide du petit Lucas et concernant les sanctions dans vos propos conclusif. Je suis tout à fait. D'accord. Je pense qu'il faut avoir des sanctions. Accrues et j'ai presque envie de reprendre la phrase d'un de vos collègues ministres, il faut être gentils avec les gentils et méchants avec les méchants. Je vous remercie. Merci la parole est à présent à Madame. Esther Benbassa du groupe né non inscrits, vous avez 3 minutes chers collègues pour vous exprimer. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 7 janvier dernier Luca âgé seulement de 13 ans a mis fin à ses jours. Si c'est si les causes directes de son passage à l'acte reste encore à confirmer les conséquences du harcèlement scolaire dont il a été victime pendant des mois ne peuvent pas être nié comme lui chaque année plus de 800.000 enfants souffrent d'harcèlement scolaire et 26% d'entre eux ont des idées suicidaires. 77% des jeunes déclare avoir subi des violences à l'école, qu'elles soient morales ou physiques, les conséquences psychologiques de ce que trop considèrent comme de simples rêveries subies pendant l'enfance sont multiples, perte de l'estime de soi tendance dépressive vulnérabilité relationnel, que ce soit dans un contexte professionnel relationnel ou amoureux à un âge où ses enfants manquent encore de discernement ou et ou très peu parviennent à parler de ce qu'ils subissent le soutien des services scolaires et d'une nécessité évidente. Comment expliquer l'escalade de violences qu'a subie le petit paraissent il y a quelques semaines. Comment expliquer que sa mère n'est pas même été prévenue par la direction de l'établissement scolaire, il y a urgence à mettre en place des protocoles adaptés afin de déceler au plus tôt. Ces situations et d'éviter que de nouveaux drames ne se produisent. Mais il ne faut pas oublier que le harcèlement scolaire ne commence pas et ne cesse pas aux portes des écoles la rue et les réseaux sociaux sont également le lieu de calvaire pour des milliers de de jeunes certes des peines sont prévues pour les auteurs de harcèlement scolaire. Mais ses enfants en ont-ils seulement conscience face à la hausse des cas, le programme phare des grilles d'évaluation du danger. Un numéro d'écoute et d'être sur le harcèlement sont-ils suffisants. Les initiatives de certains établissements et collectivités sont louables à l'heure où la sensibilisation des enfants doit être une priorité, ces violences ne doivent plus être ignoré, ni banaliser, Monsieur le Ministre vous assurer que la prévention et la lutte contre le harcèlement entre élèves et l'une de vos priorités. Les enseignants doivent plus que jamais être préparées attentives les parents alertés afin que l'école puisse redevenir un lieu d'ouverture d'esprit dans lequel chaque enfant, quel qu'il soit puisse s'épanouir sans. Je vous remercie. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Benbassa. Un mot peut être sur les les chiffres dont nous disposons, qui ne sont pas complètement stabilisé sur les questions de harcèlement. Les mesures varient selon les outils de mesure et puis aussi, selon la définition que l'on donne au harcèlement combien de situations. De violence. Réelle. Physique ou symbolique d'insultes entre ton dans la catégorie du harcèlement puisque le harcèlement suppose des actes répétés à à l'égard d'un élève. Et donc là il y a une une il y a il y a un peu de flou. Si vous voulez, mais peu importe la réalité est là et il faut bien s'y attaquer déceler les situations de harcèlement, le plus rapidement possible. C'est évidemment un des objectifs de notre mobilisation, c'est un des objectifs du programme phare j'attire votre attention sur l'importance des élèves, des élèves ambassadeurs comme nous les appelons qui sont souvent les mieux à même de repérer le changement de comportement par exemple d'un de leurs camarades. Changement de comportement alimentaire un, un élève qui s'isole. Qui change dans son attitude, dans son rapport au travail. Dans son rapport aux autres voilà des signes qui peuvent laisser penser qu'une situation de harcèlement et est en cours et donc nous comptons beaucoup sur la mobilisation des élèves et puis il faut ensuite traiter ces situations. Dans un 1er temps quand la situation est prise suffisamment tôt. C'est dans le cadre de l'établissement ou de l'école. Que la situation peut être résolue dans un 2ème temps il arrive malgré la première tentative que la situation de harcèlement perdure et à ce moment-là les autorités académiques. Les autorités départementales de l'Éducation nationale peuvent intervenir et. Avec des psychologues, ainsi que des personnels de santé qui sont associés et enfin dans un 3ème temps dans des cas extrêmes, une sanction peut intervenir selon les modalités que j'ai précisé. Merci, monsieur le Ministre, Esther Benbassa, vous avez une minute pour répliquer si vous. Le oui oui je je voudrais aussi attirer votre attention sur ce qu'on a lu récemment à propos de violence sexuelle à l'école entre des enfants de 6 ou 7 ans, c'est quand même là aussi une autre facette du même problème merci. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue Monsieur Bernard Fiolet du groupe RDSE. Et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Un an après la promulgation de la loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Où en sommes-nous. L'ajout de cette loi dans l'arsenal législatif visait à garantir aux jeunes une scolarité apaisée. Elle visait d'une part, à mieux prévenir les actes de harcèlement. La prise en charge des victimes et d'autre part à en améliorer le traitement judiciaire. Prévenir les faits passe notamment par une formation continue de toutes les personnes qui entourent les élèves au sein et en dehors des établissements sur les sujets relatifs au harcèlement. Je salue le succès du programme phare rendue obligatoire depuis la rentrée 2022 dans les collèges et les écoles élémentaires. En plus de construire. Une communauté protectrice autour des élèves d'associer des instances démocratiques scolaire telles que le comité d'éducation à la santé et de mieux former les élèves à raison de 10h par an le programme mobilise aussi 10 élèves par établissement en leur confiant le rôle d'ambassadeur. Cela responsabilise les élèves notamment dans les établissements. Plus et permet aux victimes de se confier plus facilement. Je salue aussi la poursuite de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire se déroulant depuis 2015, chaque 1er jeudi après les vacances de la Toussaint. Elle permet de sensibiliser les élèves par des expositions et des manifestations. Le s'affairent Internet dès fête sa 20ème édition cette année et rassemble grâce au travail de la Commission européenne et de internet sans crainte. Plus de 150 pays et de nombreuses associative. Je salue également l'organisation des campagnes vidéo ou des prix. Non au harcèlement organisées dans de nombreux établissements. S'ajoutent les numéros encore trop peu connue. Vous l'avez dit, monsieur et la plateforme digitale dédiée à la lutte contre le harcèlement qui a recensé plus de 170 déclaration à ce jour. Mais force est de constater que la prévention ne suffit pas. Il faut prévoir des solutions pour punir les faits lorsque le harcèlement a été commis et constater. Le nouveau cadre législatif et réglementaire a permis de créer un délit, ouvrant la voie à des poursuites à l'encontre de tout Arcelor. Un quantum de peine nécessaire proportionnée et adaptée a démontré son efficacité, notamment dans les récentes mises en garde à vue. Le harcèlement scolaire ne passent plus seulement par la parole. Ou la maltraitance physique il sévit dorénavant sur les réseaux sociaux qui poursuivent la victime jusque chez elle. Nos méthodes de sanctions doivent s'adapter. La loi a permis une avancée en considérant ces derniers comme des éléments constitutifs de cette nouvelle infraction. Nous devons aller plus loin. Il est temps d'intensifier et d'axer notre réflexion sur les méthodes de régulation des réseaux sociaux en veillant à respecter le secret des correspondances. La liberté d'expression et la sécurité pour nos enfants. Il faut également que les victimes ne subissent pas le préjudice du déplacement secondaire ce colère alors que les harceleurs conserverait de bénéfice du maintien dans le même établissement. Mais ce matin même monsieur le Ministre, vous nous avez. Peut être rassuré dans ce domaine. Certes, les pouvoirs publics n'ont cessé depuis 2010 de se mobiliser dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Il ne saurait, toutefois, se désengager. Je regrette que les dernières études disponibles remontent à 2021. Nous ne pouvons évaluer les premiers résultats de cette loi, promulguée l'an dernier comme je regrette que le gouvernement n'ait pas remis comme annoncé dans un délai de un an un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes ou par les odeurs, les auteurs En gardant un oeil sur les résultats. Poursuivons le travail engagé notamment dans le secteur du digital. Vous avez raison à propos de cette mobilisation annuelle ça compte, que ce soit le Safer Internet dès le 6 février ou que ce soit au mois de novembre, chaque année. La mobilisation autour du prix non au au harcèlement qui a. Un vrai retentissement dans les établissements scolaires. J'ai pu le mesurer moi-même. Vous avez également raison je pense du côté des réseaux sociaux. Nous devons. Les responsabiliser. La plateforme 30 18 est en lien avec les principaux réseaux sociaux pour bloquer. Des comptes avec des propos injurieux ou des photographies qui n'ont pas à circuler mais. Nous attendons que les réseaux sociaux soit plus proactif et se mobilisent encore plus. Sur ces questions. du côté des des élèves harceleurs. En effet nous j'ai fait donc cette annonce relatifs à une modification du code de l'éducation. Donc une voie réglementaire pour pouvoir. Transférer des élèves harceleurs plutôt que les élèves harcelés. Il était normal que ce soit les élèves harcelés qui doivent quitter. Un établissement par la force des choses plutôt que les élèves harceleurs mais. Nous insistons aussi sur le fait que cette décision si elle doit intervenir et en dépit de la vie, donc des représentants légaux des parents. N'intervient qu'en dernier recours lorsque d'autres solutions auront été épuisés mais je crois qu'il ne faut pas l'écarter. Il s'agit moins d'une sanction en réalité que d'une mise en sécurité des élèves qui sont harcelés et. Dans une situation où à l'évidence les procédures de conciliation ne fonctionne plus. Merci, vous avez une minute pour répliquer, chers collègues. merci madame la présidente. Monsieur le Ministre vous me répondez que vous attendez beaucoup des réseaux sociaux qui se règle. Moi je pense qu'il ne faut pas attendre passivement des réseaux sociaux qu'ils nous offrent toutes les solutions à ces risques de harcèlement. Je crois qu'il faut qu'on soit contraire un peu plus proactif et on attend justement de l'autorité. De l'État d'assurer cette sécurité. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Marie Mercier pour le groupe Les Républicains. Et vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Que se passe-t-il donc dans nos cours d'école à part jouer à son activité préférée. Pourquoi parler de l'enfer des récréations. Parce que dans ce petit monde là se. Et enfermé, on y trouve parfois du raquette des conflits de l'intimidation mais aussi du harcèlement. Un million à l'école, ça fait un million de familles. Ça fait combien de larmes. La victime, vit un calvaire. Mais son agresseur est en souffrance aussi forcément. Tout le monde est perdant. Les enfants, les parents, les familles, les enseignants et les chefs d'établissement. C'est compliqué. Le harcèlement toujours c'est une violence répétitive fondé sur des rapports de domination et de discrimination d'âge, de sexe, de religion qui a pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime qui se sont de plus en plus isolé. Détruite abandonner. Les conséquences du harcèlement sont graves, tant elle porte atteinte à l'intégrité de ses enfants, elles peuvent parfois conduire au pire. Il est urgent que le drame subi par ses enfants soient rapidement admis et sérieusement pris en considération sous tous ses aspects. En la matière, la prise en charge préventive et bien entendu la meilleure des choses que le harcèlement ne commence pas ou soit repéré et gérer au plus tôt. Ce sont les programmes phares mais quand il est trop tard, il installe c'est au monde adulte de prendre toutes ses responsabilités pleine et entière, la victime doit être protégé avoir foi en notre justice est de son côté le harceleur doit réaliser que ces actes sont répréhensibles et être lui-même accompagné dans sa souffrance finaux qui. Citoyens seront-ils demain. La proposition de loi. J'ai déposé le 21 février visant dans le cas d'un harcèlement scolaire a posé le principe d'une mesure d'éloignement du harceleur. Pour protéger la victime a profit de poser un principe simple, ce n'est pas la victime de fuir de quitter l'établissement et son environnement pour échapper à son harceleur, ce n'est pas à sa famille de s'adapter de s'adapter à ce changement mais au petit harceleurs. Les maires me disent, signer les dérogations avec la boule au ventre disons c'est encore faisant qui gamin qui va être obligé de partir. J'ai voulu donner aux établissements scolaires une référence sur laquelle s'appuyer pour agir et je remercie les 215 collègues sénateurs qui ont bien voulu signé mon texte et ceux qui le partage puisqu'ils l'ont repris. Il existe bien sûr une procédure disciplinaire applicable aux élèves qui relève du pouvoir réglementaire et du règlement intérieur des établissements. Aujourd'hui, rien n'empêche un conseil de discipline d'exclure un élève auteur de faits de harcèlement, force est de constater que la plupart de temps, cela ne se fait pas. Il s'agit donc bien d'affirmer une position de principe de guider et de soutenir l'. Selon dans leur prise de décision dans la mesure de trop nombreux des moyens âge montre que les jeunes victimes subissent la double peine. Monsieur le mini. Je me réjouis que vous soyez emparé de cette idée. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt. Pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire la nécessité reste d'agir en amont en leur reconnaissant en le nommant et en évaluant l'efficacité des dispositifs mis en place. Aucun enfant ne devrait avoir à quitter une école protéger les enfants. Et notre devoir comme celui de leur transmettre des connaissances dans un milieu apaisée qu'relève. Lors, hein. Insouciance et qui leur laisse leurs rêves. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Pour votre mobilisation sur cette question, c'est l'occasion pour moi de vous remercier très vivement pour votre. Proposition de loi qui a d'ailleurs été signée sur tous les bancs très largement par. 215 de vos collègues. En matière. De d'enseignement primaire comme vous le savez, il n'y a pas de procédure disciplinaire, il n'y a pas de conseils de discipline. D'où l'impasse que nous avons connu récemment dans le cas du jeune Maëlle. Puisque. La. Le transfert ou le déplacement. De l'élève harceleur été soumis à l'accord des représentants l'légaux à à l'accord de la famille avec la proposition que je fais de modification du code de l'éducation. Cela pourra passer on pourra passer outre l'avis des parents. Avec l'accord du maire qu'ont concerné donc je pense que c'est une avancée tout à fait importante, on inverse finalement la situation puisque c'est le harceleur qui part et non pas le harceler. Il faut admettre que c'est une question de justice tout simplement et que on pourra avancer quand il est trop tard comme vous l'avez dit, il faut pouvoir agir et pouvoir déplacer l'élève C'est une solution de dernier recours, mais il faut pouvoir envisager cette solution dans le premier degré, comme dans le second degré et donc c'est quelque chose que nous allons faire et encore une fois, je vous remercie de votre mobilisation sur cette question. Merci. Si vous le souhaitez répliquer. Mais merci. Monsieur le Ministre, oui effectivement vous proposez exactement en tout point ce que j'ai proposé de, de Nasri dans le code de l'éducation. Je voudrais vous prévenir de quelque chose, j'ai fait de nombreuses auditions et à l'intérieur même de l'éducation nationale, on m'a dit oh ben si ça devient compliqué, on n'écrira plus jamais harcèlement on mettrait autre chose. Je trouve que ça ce serait pas digne. De l'éducation nationale. Et. Merci la parole est à présent Monsieur Yan Chantrel du groupe socialiste et vous avez 3 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons tous et toutes étaient profondément touchée par le suicide du jeune Lucas qui subissaient quotidiennement harcèlement et moqueries sur son orientation sexuelle. Depuis ce drame, quelles sont les mesures que vous avez prises pour mettre fin aux brimades quotidiennes sur subies par une partie de de nos enfants. Votre volonté d'éradiquer ce fléau que constitue le harcèlement scolaire se vérifiera par vos actions, sur deux leviers essentiels. Plus de moyens humains à l'école et un changement de la culture scolaire qui prévaut dans d'autres pays, chacun le sait, la meilleure façon de lutter contre le harcèlement scolaire, c'est d'augmenter la présence en personnel pour encadrer les élèves. Toutes les recherches démontrent que plus les effectifs sont réduits dans l'établissement et dans la classe plus le harcèlement diminue. Or la France a les classes les plus chargés de l'Union européenne au collège l'effectif moyen approche 26 élèves c'est très au-dessus de la moyenne européenne située sous la barre des 21. Plus d'une classe sur 10 dépassent désormais les 30 élèves, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et pourtant depuis son arrivée au pouvoir. Emmanuel Macron n'a fait qu'empirer. Cette situation dramatique. Depuis 2018, le second degré a perdu 9322 enseignants et la saignée continue puisque votre ministère annonce de nouvelles suppressions de postes pour la rentrée 2023. À ce terrible bilan s'ajoute l'abandon de la médecine scolaire qui a déjà été évoquée par des collègues. La France compte aujourd'hui un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves et un médecin scolaire pour 16.686 élèves, loin, très loin de la préconisation de votre ministère de un pour 5000. Comment prétendre lutter contre le harcèlement scolaire, quand on réduit à ce point les moyens de l'école. Le second levier, c'est celui de la culture et de l'organisation scolaire qui prévalent dans notre pays. Face au fléau du harcèlement, la manière dont on conçoit et organise l'école peut le favoriser ou le décourager. On a trop tendance à prendre le problème sous l'angle de la discipline avec une approche purement punitive et a délégué la lutte contre le harcèlement au CPE plutôt que de développer une approche collective, c'est en amont dans notre culture et organisation scolaire qu'il faut aller chercher les ressources pour lutter contre le harcèlement face une école de la concurrence entre individus du classement et de la distinction qui créent des rivalités contre la pression des notes et le stress des examens défendons un modèle qui prône des valeurs de solidarité et de coopération de bienveillance, de tolérance et d'inclusion un modèle aussi ou la santé mentale n'est plus un tabou. Un modèle scolaire qui place la mixité en son coeur pour développer une approche positive de l'autre ou l'altérité. La différence ne constitue pas un danger, mais une chance pour aller dans le sens vous nous aviez justement promis ici même, Monsieur le Ministre des annonces sur la mixité scolaire pour le 20 mars. Nous les attendons toujours. Où en est-on. Merci Monsieur le Ministre pour répondre. Merci madame la présidente, monsieur le Sénat. Auteur Chantrel depuis. La catastrophe la mort du jeune Lucas. Nous avons intensifié en particulier les programmes de lutte contre la et haine anti-LGBT. J'ai eu l'occasion d'en parler, nous préparons activement la journée du 17 17 mai et nous avons généralisé les les observatoires qui sont des bons points d'appui dans chaque académie. Pour. Se mobiliser pour sensibiliser. Au haine anti-LGBT qui ont des effets catastrophiques dans nos écoles. Vous avez mentionné la question des effectifs et là je suis obligé d'apporter un bémol à votre propos, il n'y a pas de lien si évident que cela entre les situations de harcèlement et puis les effectifs dans le cas du jeune Maëlle par exemple la classe, qui est la sienne n'a que 10 élèves et donc on est dans une situation qui n'est pas une situation de surcharge en ce qui concerne la médecine scolaire bien entendu que je partage le constat je l'ai dit, mais nous avons des postes qui ne sont pas pourvus. J'ai en mémoire la situation du département des Vosges. Qui. A. 10 postes de médecins scolaires et sur ces 10 postes, huit ne sont pas pourvus, huit sont vacants, et donc on pourrait en rajouter. Cinq ou six que ça ne changerait rien à la situation et donc on a un problème de fond qui est celui. qui vient du fait que les étudiants en médecine ne choisissent pas la médecine scolaire ne choisissent pas non plus la médecine du travail, donc c'est une réflexion de fond sur l'organisation de la médecine scolaire et sur ses Liens avec la médecine de ville qui est en jeu, enfin je souscris bien sûr à l'approche collective que vous soulignez, c'est la formation de tous les adultes, pas seulement la vie scolaire mais également les professeurs mais également toutes celles et ceux qui interviennent auprès des élèves qui peut faire fonctionner qui fait fonctionner le dispositif hein.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En France et cela étages a été évoquée. Près d'un enfant sur 10 serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire. Et ces dernières années, le harcèlement en ligne est venue amplifier ce phénomène. En 2021, ce sont 20 enfants et adolescents qui ont perdu la vie à cause de ce fléau. On considère qu'il y a harcèlement scolaire quand un jeune est victime d'une agression répétée délibérée souvent effectués en meute. C'est également un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. De caractère répétitif des agressions crée souvent un sentiment d'isolement et d'abandon dès harcelé qui deviennent incapables de trouver des réponses pour s'en sortir. Le harcèlement pénalisent durablement le parcours scolaire de la jeune victime et peut entraîner des conséquences psychologiques très lourdes allant jusqu'au drame du décrochage scolaire à des conduites autodestructrice voire suicidaire. Dans un monde où Internet à quand par nos vies et plus encore celle de nos adolescents. Le harcèlement en ligne ou cyber harcèlement sur les réseaux sociaux dans les forums, les jeux vidéo multiforme ou sur un blog, est devenue à le véritable danger. C'est le type de harcèlement qui est le plus destructeur pour les victimes car via les réseaux sociaux, les agressions ou brimades peuvent frapper leur victime à tout moment de la journée de la nuit et quel que soit l'endroit où elle se trouve. De plus le harceleur peut se servir d'un pseudo et ne pas dévoiler son identité. Alors, quelles mesures pour lutter efficacement contre la cyber harcèlement et ainsi casser cette spirale de violence. Le comité d'éducation à la santé à la citoyenneté et à l'environnement, le CES CE a commencé à sensibiliser les chefs d'établissement à ces problèmes de harcèlement. Cependant ce dernier montre ses limites avec beaucoup de dispositifs lister les un manque de moyens humains et financiers pour les appliquer. Depuis la rentrée 2022, le ministre de l'Éducation nationale que vous êtes arrêté un plan de prévention du harcèlement entre élèves avec le programme phare dont vous avez déjà parlé, devenu obligatoire dans nos établissements. Celui-ci combine plusieurs actions et dispositifs incluant un large éventail d'outils variés et concret. Se basant sur 8 piliers pour notamment éduquer pour prévenir des problèmes de harcèlement former une communauté protectrice de professionnels intervenir efficacement sur les situations de harcèlement. Pour une réussite de ce dispositif, il faut impliquer, élèves et personnels travaillant en collaboration avec les parents et des partenaires associatifs, mettre à disposition une plateforme numérique dédiée et créer une équipe de 5 personnel formé et une équipe d'élèves dans ambassadeur. Au niveau académique de superviseurs sont des personnes ressources pour les établissements et sur le plan national et de lignes dont vous parliez, le 30 20 de 30 18 qui propose un soutien aux victimes de harcèlement. Les responsables des établissements scolaires doivent doivent être vigilants à détecter tout harcèlement. Mais il est également indispensable que les harceleurs prennent conscience de leurs actes et des conséquences judiciaires et financières qu'ils encourent ou leurs parents lorsqu'ils sont mineurs. Cette année, notre collègue Marie Mercier déposer une proposition de loi visant à poser le principe de l'éloignement du harceleur pour protéger la victime et c'est une très bonne chose enfin j'évoquerai pour ma part plusieurs pistes de réflexion et d'action qui pourrait être mises en place. Le renforcement du programme phare avec la prof, formation continue des du groupe des 5 personnes de l'établissement secondaire ou par les par circonscription pour le primaire, une obligation des plateformes de contrôler et de supprimer les conflits les contenus délictueux. Qui soit d'ordre sexuel ou de harcèlement l'exclusion automatique du harceleur de l'établissement lorsque la situation de harcèlement est avérée. Et le développement de la médecine dont vous avez parlé tout à l'heure avec des professionnels qui soient formés à détecter le mal-être d'une victime de harcèlement le le monde médical et du vous avez du mal à trouver des médecins pour le la prévention scolaire mais la prévention par l'information est également est primordial. Et je crois que dénoncer un comportement délictueux de harcèlement doit être entrevoir pour tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre.

dans les différentes déclinaisons de la mobilisation que nous menons et j'ai déjà indiqué à quel point nous sommes sur le chemin. Rien n'est. Complètement réalisé mais nous avançons et nous progressions

des photographies ou des propos en quelques heures, de manière à ce que. Les élèves concernés soient. Protégés. J'ai pu écouter. Lors d'une visite. Au 30 18. Des conversations entre eux des collégiens ou des familles qui appelle paniqués parce que il y a telle ou telle photo qui circule et puis les personnes qui répondent, il y a des techniciens, il y a des psychologues. On prend en charge les élèves ils je salue évidemment le travail qui est réalisé en la matière. Je voudrais aussi mentionné un point qui complète votre propos dans la généralisation du programme phare hein on on est à 60%, il y a 86%, on n'est pas du tout à 100 pour % mais tout de même ça progresse. Le fait que ce programme donc sera étendue au lycée. À partir de la rentrée prochaine en sachant que les cas de harcèlement. Du côté des lycées sont moins nombreux hein, c'est plutôt du côté. Du cycle 3 et du collège que les situations de harcèlement sont les plus nombreuses mais il n'y a aucune raison de ne pas non plus se mobiliser. Du côté des lycées et c'est ce que nous allons faire pour le dire plus rapidement. L'éducation nationale se met en marche et se met en en mobilisation parfois comparé à. Une grosse bête de l'ère glaciaire. Moi je vois que l'éducation elle s'est bougé sur des questions importantes comme celles du harcèlement. Merci. Vous avez une minute pour répliquer, chers collègues.

passer et que les parents comme les enseignants comme toute, toute personne doit. Défendre prendre qu'il n'y ait plus jamais d'enfant harcelé merci. Merci la parole est à présent notre collègue Madame Sylvie Robert du groupe socialiste et vous avez 3 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme le rapport d'information sénatorial sur le harcèlement et le cyber harcèlement de 2021 l'avait démontré ce phénomène violent n'a été appréhendé reconnue que tardivement en France alors même que des travaux de chercheurs avaient commencé dès les années 70 pour autant avec le développement du numérique et l'explosion de l'usage des réseaux sociaux ces formes ont évolué alors cantonnées à l'enceinte de l'école. Le harcèlement scolaire se prolonge désormais sur les plateformes numériques l'amplifiant dramatiquement et le rendant plus sauvage et potentiellement dangereux. D'ailleurs 2002 1009 Michel va rêve dans ce rapport sur le cyber harcèlement soulignait le rôle joué par l'anonymisation et il affirmait même que le cyber harcèlement justement par ses caractéristiques et son objet pouvait avoir des effets particulièrement dangereux et durable. Ainsi la loi du 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire a été une première étape. Elle a notamment assigné aux fournisseurs d'accès. Internet la lutte contre le harcèlement scolaire comme objectif et a établi une obligation de modération des contenus de même nature sur les réseaux sociaux. Néanmoins il apparaît souhaitable et pertinent d'aller plus loin dans cette régulation par les plateformes, même si cette dernière ne sont pas responsables des faits de harcèlement mais constitue plutôt des vecteurs par lesquels le harcèlement se matérialise. Sur ce point, le rapport précité effectuer une série de préconisations. Tout en rappelant la difficulté du cadre juridique, national et européen. Parmi ces propositions figuraient l'obligation par exemple pour les réseaux sociaux de présenter de manière explicite et compréhensible par les jeunes utilisateurs des extraits des principales conditions d'utilisation singulièrement celles relatives au cyber harcèlement l'obligation pour les réseaux sociaux de présenter périodiquement à leurs utilisateurs une courte vidéo de sensibilisation sur les bons usages du numérique sur la prévention du cyber harcèlement et les moyens pour les victimes de réagir sur cette seconde recommandation un consensus semble émerger suite à l'adoption du Digital Services Act au niveau européen. Lesquels renforce la responsabilité des plateformes d'ailleurs Marc collègue Sabine vendent Egg a déposé une proposition de loi dans ce sens. Celle-ci est au frais utilement notre arsenal juridique, législatif et complèterait habilement la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique qui a lutté contre la haine en ligne, qui je crois va être prochainement débattu dans notre hémicycle. Ainsi, Monsieur le Ministre, vous qui êtes engagés sensible à la gravité du cyber harcèlement y seriez-vous favorable, je vous remercie. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Robert. Je vous remercie également pour. Vos propos qui témoigne de la mobilisation du du Sénat tout entier finalement sur cette question et je suis tout entier avec vous sur cette question aussi. À propos du cyber harcèlement j'ai mentionné la plateforme 30 18 j'ai mentionné la responsabilité des plateformes je suis tout à fait ouverts et disposés à avancer sur cette question. Bien entendu que l'état a une responsabilité en la matière et donc je suis. Je suis ouvert au travail commun. Avec avec vous pour avancer, progresser et réduire le fléau du cyber-, harcèlement. je voulais remercier monsieur le Ministre de sa réponse. Je pense qu'on a beaucoup de travaux à venir dans le, dans le domaine du cyber harcèlement et singulièrement même dans le domaine du numérique et je pense que ce sera une responsabilité collective de pouvoir avancer ensemble effectivement, merci beaucoup. Merci la parole est à présent à notre collègue Madame Sabine Draxler pour le groupe Les Républicains et vous avez. Trois minutes. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. La médiatisation récente de plusieurs suicides d'enfants a révélé à ceux qui l'ignoraient encore ce qu'était le harcèlement scolaire et ses effets à court terme. Ce que l'on sait moins. C'est que la santé leur travail plus tard ou la parentalité de ceux qui auront subit fait subir ou été témoin de ces violences en seront marquées toute leur vie. Anxiété sociale pour les victimes. Abus de pouvoir au travail ou en famille pour les agresseurs, sentiment d'impuissance pour les témoins le harcèlement scolaire explique de nombreux mots à l'âge adulte. Dépression. Violences intrafamiliales chômage ses conséquences sanitaires humaines et financières sont énormes pour la société. L'éducation nationale a pris conscience de la nécessité d'agir mais il me semble, il semble à l'enseignant spécialisé que j'ai été que la mise en place de programmes tels que Far ne peut être efficace qu'à la condition que des personnels des professionnels dédiés soit présent en appui des enseignants et auprès des élèves pour bien connaître et suivre les situations individuelles. Sans moyens humains ce dispositif resteront des coquilles vides, des méthodologies pour la plupart théorique souvent impossible à mettre en oeuvre faute d'équipes spécialisées pour les accompagner. Malheureusement, vous le savez Monsieur le Ministre, les écoles en zone prioritaire bénéficient de moyens encore conséquent. Mais dans la ruralité les postes spécialisés sont supprimés les uns après les autres. Plus de médecine scolaire plus de psychologue, plus d'enseignants spécialisés quasiment partout. Ceux qui restent sont submergés peu reconnu pour ce qu'ils font dans l'impossibilité de remplir leur mission est de répondre à la masse des demandes d'aide. Je pense qu'il s'agit là d'un mauvais calcul, car ces et ces économies, à court terme auront ont déjà des conséquences humaines et sociales désastreuses. Je le vois chez moi, en pleine campagne où les enseignants sont livrés à eux-mêmes et où les violences intrafamiliales explosent. Monsieur le Ministre, je vous pose la question, vaut-il mieux prévenir ou guérir vaut-il mieux créer des postes d'enseignants spécialisés ou des postes d'intervenants sociaux en gendarmerie. nous dit que la France compte suffisamment d'enseignants peut être mais il ne faut pas négliger la ruralité ne plat négligé des territoires que le pense préserver et qui ne le sont en fait plus du tout. Chez moi dans le sud de l'Alsace. Il ne reste que 3 personnel spécialisé pour 108 communes. Les enseignants, les élus et les familles se sentent abandonnés et je crains qu'il n'ait raison. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Draxler. Non ils ne sont pas abandonnés. Ça c'est quelque chose que je peux vous assurer d'abord parce que. Et j'ai eu l'occasion d'en parler devant. Vos collègues. Nous avons lancé un plan ruralité avec un engagement pluriannuel à partir de cet Automne pour donner de la visibilité. En matière de postes sur 3 ans pour ce qui concerne les écoles dans les territoires ruraux. Donc nous allons. cette cette visibilité aux maire pour éviter d'une année sur l'autre des changements brutaux de la carte scolaire. Par ailleurs, en matière de moyens humains, les zones. Les territoires ruraux sont relativement favorisées par rapport aux territoires urbains et c'est une bonne chose, bien entendu, puisque la question de l'éloignement fait que. La densité des écoles est moindre et donc nous avons un taux d'encadrement qui est meilleur dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, mais cela ne répond pas entièrement à votre question sur. Le harcèlement. Nous avons des moyens et des moyens, par exemple en matière de formation, la formation, que ce soit au niveau national, au niveau académique ou. Au niveau départemental. Ça coûte, ça représente des moyens et nous sommes évidemment déterminés à faire de telle sorte que ces moyens soient prorogés par ce que nous devons réduire à l'évidence et de manière absolument déterminante. Les situations de harcèlement. Encore une fois, nous sommes sur un chemin il les territoires ruraux ne sont pas oubliés. Merci vous pouvez répliquer à une minute, chers collègues. Monsieur le Ministre, dans certains secteurs en France il n'y a même plus de psychologues scolaires pour, pour évaluer les élèves en situation pour lesquels il y a une suspicion de handicap. Il y a plus d'enseignants spécialisés pour attraper des enfants qui serait pourtant rattrapable. Quel gâchis. Et quel coût aussi à venir dans quelques années pour accompagner les adultes qui seront devenus et qui seront dans l'incapacité de s'insérer dans la société, des coûts qui seront et qui seront déjà autrement plus élevés que que les quelques postes économiser. Merci la parole est à présent à Madame Toine bourrin pour le groupe Les Républicains et vous avez 3 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le harcèlement scolaire blesse broie brise et vol ce que la vie offrent de plus précieux, l'enfance. Ce terreau fertile où pousse les goûts l'apprentissage et les prémices de la conscience morale civique et donc sociale. Dans ce pays où l'on prétend combattre l'endémie d'un mal par un numéro Vert. Il est temps de mettre un coup d'arrêt à une spirale que le développement des technologies rend bien souvent infernal. Pour y parvenir, Monsieur le Ministre. C'est une culture de la vigilance qu'il nous faut instituer une culture qui se pense et se déploie au plus près du terrain, c'est-à-dire des victimes potentielles ou avérées. Il s'agit de détecter rapidement d'agir en local pour laisser les enfants le moins longtemps possible en situation de harcèlement. Car les premiers témoins sont les enfants eux-mêmes ils sont spectateurs libérant leur parole expliquons que l'idée n'est pas de dénoncer un harceleur mais de signaler un élève harcelé. C'est une assistance à personne en danger. À cet égard les applications intra-. Collèges et lycées type Pronote pourrait être utilisée comme plateforme interne d'alerte permettant aux témoins de signaler un élève en difficulté. Tout en préservant leur anonymat. 1er rempart dans l'accompagnement psychosocial nous devons également redresser une médecine scolaire en grand danger. Oui, je le répète une médecine scolaire. Abandonné. Nous comptons seulement un médecin pour 12.000 élèves. Une situation que Dominique Bussereau qualifié d'indigence devant le Sénat, lors de sa dernière audition. Plus encore, il convient de traiter ce fléau dans son intégralité le programme phare dont vous avez annoncé le déploiement au lycée n'est qu'une réponse partielle à un problème global. Ce qu'il nous faut comme en Finlande depuis plusieurs générations. C'est un bouleversement culturel l'avènement d'une société de grands témoins non de la suspicion, mais de l'attention portée aux autres où chacun est le maillon d'une chaîne de valeur, trop souvent ignorées. Chez nous, le respect de l'autre l'interaction sociale et la compréhension des émotions d'autrui. Plus qu'un programme. La Finlande a développé cette culture de la vigilance que le temps long et surtout les moyens humains comme financiers font infuser au quotidien avec des résultats surprenants marqué par la baisse de plus de 40% du phénomène. Enfin, comment peut-on penser lutter contre le harcèlement scolaire en faisant l'économie de son volet cyber. Nous avons le devoir d'éviter la dissémination des comptes la multiplication d'identité les identités factices et des comptes fantômes qui prospèrent grâce à l'anonymat et au pseudonyme Qu'attendons-nous pour corréler l'identité numérique à l'identité réelle des utilisateurs de réseaux sociaux. Techniquement c'est déjà possible. Alors Monsieur le Ministre, les militaires qui savent mieux que personne, traiter l'urgence ont une formule que je fais mienne être à l'heure, c'est déjà être en retard du retard, nous en avons à rattraper la France le peut comme la Finlande, la fait. Merci madame la présidente. Merci madame la. La sénatrice évidemment je. Je partage vos préoccupations sur les questions de de cyber harcèlement permettez-moi un mot sur le cas de, de la Finlande, que vous avez cité justement dans le cas de la Finlande, le programme qui va. Qui a donné de, de bons résultats. Ça a mis 10 ans pour parvenir au résultat. Que l'on, que l'on sait. Donc ça a pris du temps aussi. En Finlande. Quant au programme que nous avons déployé, il y a, il est beaucoup plus récent. Bien entendu, nous espérons avoir des résultats plus rapidement en évaluation internationale en tout cas le les regards internationaux qui sont portés sur nos efforts. Salut. La qualité de ce que nous faisons. On a un problème plutôt en cours de déploiement, je dirais hein on n'est pas à 100 pour %. Loin de là mais. Les les efforts que nous faisons sont salués. Et nous espérons mettre moins de 10 ans pour parvenir à des résultats comparables à ceux de la Finlande, l'expérience internationale est évidemment très utile. Pour ce qui concerne. Ce que nous faisons. Du côté des écoles, des collèges et des lycées. Merci. Si vous souhaitez répliquer une minute. Juste une petite précision, une petite. Chez le ministre a, c'est que les résultats du programme finlandais sont bien meilleurs que les 40% que j'évoquais au bout de 10 ans les 40% que j'évoquais ce sont des résultats qui ont été. Chiffrées évaluer au bout de 2, voire 3 ans. Merci monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, vous avez 5 minutes pour vous exprimer, si vous le souhaitez maman.

Merci madame la présidente, je vais m'exprimer brièvement car. Et je pense que nous avons. N'ont pas fait le tour de cette question, comment pourrions-nous mais enfin. Aborder un certain nombre de questions importantes. Je me permettrais simplement Mesdames et messieurs les les sénateurs. De. Récapituler quelques points, d'abord la question de la formation puisque ce cette question est revenue à plusieurs reprises nous avons concentré nos efforts sur les équipes au sein des écoles et des collèges et notre objectif est effectivement celui de former tous les personnels comme le prévoit d'ailleurs la loi du 2 mars 2022 à commencer par la formation systématique des professeurs stagiaires qui a commencé. Nous allons donc mobiliser encore davantage les Inspé et les écoles académique de formation continue. Nous devons aussi. Suivre qualitativement et quand est. Les actions menées et. J'ai indiqué que nous avons encore des marges de progression puisque 86% des collèges et 60% des écoles sont actuellement inscrits dans le programme. L'objectif, c'est évidemment 100% et l'extension du programme. Au lycée dès la rentrée prochaine. Comme le recommandent les sénatrices. Mélo et Vanek dans leur rapport d'information de septembre 2001. Nous allons mettre en place la systématisation à chaque rentrée scolaire, de la communication des numéros d'urgence le 30 18 et le 30 20 dans les carnets de correspondance et les supports numériques. Enfin. À propos. De la situation de l'de l'élève harceleur. si le rôle de l'éducation nationale et de prévenir d'accompagner et de protéger les élèves, il faut le reconnaître certaines situations ne peuvent se régler qu'en séparant les élèves harcelés de leur harceleur souvent pour mettre fin rapidement aux souffrances causées par le harcèlement, les parents de l'élève harcelé font le choix de le changer d'établissement et je comprends. Nous comprenons le sentiment d'injustice qui peut naître de cette situation puisqu'il n'est pas possible dans le 1er degré, contrairement au second degré qui dispose d'un conseil de discipline de déplacer un élève dans une autre école sans l'accord des parents, nous mettons en place des actions éducatives en fonction de la gravité de la situation, y compris donc dans les cas extrêmes. Lorsqu'un élève fait peser du fait de son comportement répété. Une menace grave sur la sécurité des autres élèves Nous allons porter une évolution des textes réglementaires pour instaurer une procédure permettant de déplacer dans une autre école un élève auteur de harcèlement de harcèlement et ceci sans l'accord des représentants légaux. C'est l'obligation de mise en sécurité de l'élève qui justifie cette exception bien entendu nous avons affaire à des élèves de 6 à 10 ans. Donc nous devons être prudents car nombre de cas de harcèlement ne sont pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais. Le le déplacement de l'élève harceleur et tout, tout de même. Essentiel Essentiel même si toute procédure d'exclusion doit être entouré des garanties indispensables aux droits de l'enfant qu'il soit l'élève harcelé ou l'élève harceleur. Si vous me permettez je terminerai mes propos en ayant une pensée. Émue pour tous les élèves victime de harcèlement scolaire. Notre débat je crois leur rend hommage. Et je sais que nous sommes tous ici pleinement engagée pour trouver des solutions afin de prévenir ce phénomène et les drames encore récent qui viennent nous rappeler douloureusement qu'il nous reste encore à faire. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre pour conclure le débat. La parole est à monsieur Max Brisson. Pour le groupe des Républicains. Madame la présidente de ce Ministre, mes chers collègues. D'abord, merci Monsieur le Ministre pour vos propos de faim et merci d'ailleurs pour toutes les précisions et les annonces qui ont nourri cet échange. Je crois que le groupe Les Républicains a eu raison de demander ce débat. Il a généré du bien compréhensible. Consensus. Cela risque de ne pas être tout à fait le cas dans le débat qui va suivre. Donc nous avons goûté et je pense que le sujet le mériter. Je remercie Alexandra Borchio-Fontimp d'avoir posé fortement tout à l'heure les termes du débat et d'avoir largement repris comme beaucoup d'entre vous. Les travaux de la Haute Assemblée notamment à la cause à l'occasion de la mission d'information de nos collègues Sabine Vanek et Colette Mélot plusieurs drames sont hélas venu rappeler récemment l'urgence à intensifier la lutte contre ce fléau. Beaucoup ont parlé de Lucas. Qui s'est suicidé. Après avoir été harcelée dans son collège et sur les réseaux sociaux en raison de son homosexualité. Je voudrais rappeler moi ce lycéen qui après avoir subi un harcèlement dans son ancien collège a assassiné récemment son enseignante dans son nouveau lycée il est hasardeux bien sûr de faire la moindre corrélation mais le drame, Saint-Jean-de-Luz et dans toutes les têtes. Beaucoup ont dit. Qu'au-delà de ces cas extrêmes qui émaillent l'actualité qui a aussi une réalité ordinaire quotidienne vécue par de nombreux enfants. Beaucoup ont justement rappelé que le cyber harcèlement prolonge dans la sphère privée, y compris le week-end le harcèlement et que depuis le confinement. Les cas sont de plus en plus nombreux. Pour autant. Comme l'indiquait déjà notre mission sénatoriale nous manquons d'appareil statistique d'enquête précise récente et régulière. Par ailleurs, il faudra aussi que nous menions assez rapidement une évaluation des effets du programme phare ainsi que du dispositif pénal issu de la loi du de mars 2022, il s'agit d'un préalable essentiel pour un plan d'action plus efficace. En 2021 notre mission Puente la détection comme un axe majeur. Pour progresser, nous avons beaucoup parlé de besoins, de formation des personnels. Le 1er niveau de lutte contre le harcèlement pas défait par la compréhension du phénomène, et la communication. Le principe d'une formation initiale et continue de l'ensemble des acteurs concernés a été inscrit dans la loi du 2 mars 2022, mais semble loin d'être appliquée dans les faits, vous venez de le dire et vous venez de réagir sur le sujet 2 tiers des enseignants dénoncent encore un manque de formation. Ainsi qu'une absence de prise en considération par leur hiérarchie. Vous avez réagi tout à l'heure sur le pas de vague.

Beaucoup l'ont dit avec un temps plus ou moins conciliant. Il est nécessaire d'identifier plus rapidement les cas de harcèlement. Nous butons ici. Sur le manque criant de médecins scolaires d'infirmières, de psychologues, pourtant les mieux à même de repérer la détresse de l'enfant et de recueillir sa parole. Nous attendons donc le plan que vous avez annoncé et sa mise en oeuvre et nous aurons des propositions à vous faire sur le sujet. Après le repérage d'un cas de harcèlement. Le traitement de la situation est essentielle. Les retours que nous avons des associations et des familles montre encore que des progrès peuvent être réalisés que les victimes et leurs parents ne se sentent pas suffisamment écoutés et soutenus généraliser le programme phare, manque de moyens humains et financiers et repose sur des dispositifs qui ne sont pas encore assez explicite pour assurer une vraie prise en charge dans les. Établissements scolaires et une meilleure orientation vers les intervenants extérieurs. Par ailleurs on nous avons beaucoup parlé d'un propulsion de loi de notre collègue Marie Mercier, proposition de loi que nous soutenons fortement et Alexandra Bourgeot la répéter, vous venez de faire des annonces, elles sont les bienvenues. Nous attendons des mesures précises. L'essentiel est de toute façon de régler la question en conclusion, Monsieur le Ministre, nous attendons que les recommandations du Sénat que la proposition de loi de notre collègue Marie Mercier soient réellement prises en compte dans le programme phare et deviennent surtout effective sur le terrain, nous serons donc pratiquement attentif dans les prochains mois à la mise en oeuvre de tout ce que vous avez annoncé ce matin et répété cet après-midi la mobilisation ne doit pas fléchir le Sénat vous accompagnera la sérénité de tous nos élèves à l'école est en jeu. Merci cher collègue. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi pour une école de la liberté de l'égalité des chances et de la laïcité, présenté par Monsieur Max Brisson et plusieurs de ses collègues. À la demande du groupe des Républicains. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Max Brisson que nous allons appeler à nouveau. Sur ce plateau. Chers collègues, vous avez 10 minutes. Pour ce faire.

Première mission en volume l'an dernier nouveau qui ont un budget de 60 milliards d'euros. Et pourtant et pourtant la performance d'autres systèmes éducatifs ne cesse de se dégrader, production d'illégalité décrochage dans les classements internationaux lacunes dans l'acquisition des savoirs fondamentaux, enquêtes et rapports nous alerte sur la dramatique, baisse du niveau en mathématiques et en sciences ou sur les difficultés croissantes des élèves en lecture et en compréhension. Simple ces évaluations inquiètent un peuple tout entier. Sans qu'on puisse les en blâmer, année après année, les parents canon les moi hier font fuir à leurs enfants les plus mauvais établissements. L'évitement est devenue au sport national. le nombre de candidats au métier d'enseignant font le ministère recrute en urgence des contractuels bombardé professeur en 48 heures et affectés dans les établissements les plus difficiles. Le métier de moins en moins attractif et nous doutons Monsieur le Ministre, que la seule revalorisation des salaires aussi nécessaire qu'elle soit remplace une réponse structurelle. L'éducation nationale est en crise. Pourtant pourtant l'attachement à notre école demeure son redressement et espérer s'il y a des divergences. C'est sur des réponses à apporter pour la majorité des acteurs et sont essentiellement financières. Entre 2012 et 2017 11 % de hausse du budget de l'Éducation. Entre 2017 et 2021, 22 21 % d'augmentation. C'était une nécessité. Assurément, les résultats ont il était à la hauteur. Certainement pas. Depuis trop longtemps. Crédits et moyens supplémentaires. Seront les remèdes exclusif à la dégradation de notre école. Ne nous y trompons pas, il masque l'impuissance l'impuissance à réformer un système trop vertical trop uniformes et oublieux des particularités. On dépense beaucoup. Alors qu'on ne repense jamais en profondeur l'organisation de notre système éducatif. Impuissance à laquelle la rue de Grenelle a trop souvent répondu par plus de contrôle plus de procédure plus de circulaires plus de mer mise dans la vie des des établissements et par une GRH qui in fine et s'est coupé de la réalité des conditions d'exercice du métier d'enseignant. Ces dernières années aux rares. Ministérielle qui dans le passé. Fixer un cadre et des objectifs généraux ont succédé l'avalanche des circulaires. La multiplication des injonctions l'enchevêtre ment des contrats d'objectifs et disons-le le plaisir d'un verbiage plus ridicule que précieux. Alors qu'en Europe la tendance générale conduisait à donner plus de souffle, plus d'autonomie au système d'éducation. En France verticalité centralisation uniformisation épuise désormais toutes les initiatives et décourage les meilleures idées, tout cela bien sûr au nom des grands principes d'unité d'égalité. Alors que notre système scolaire produit ségrégation et inégalités. Le coeur de cette proposition de loi et d'en d'en finir avec cette asphyxie bureaucratique et d'engager une rupture avec le conservatisme ambiant. Arc-bouté sur de Maxime qui font Florès au ministère, on l'a déjà fait et c'est impossible pourtant. Rapport après rapport, la Cour des comptes nous le dit les systèmes scolaires les plus performants sont ceux qui donnent le plus de place à chaque établissement fédérant à ce niveau la communauté éducative autour d'un projet co-meurt, qui encourage les enseignants à être novateur. Et à améliorer leur performances et celle de leurs collègues. Tout est dit. Ce sont bien la liberté et l'autonomie qui font défaut. Je vous propose donc de poser les fondations d'une plus grande autonomie des stades saumon scolaire à travers la création expérimentale sur la base du volontariat des établissements publics autonomes d'éducation. Ces établissements auront la possibilité de contractualiser avec les recteurs et les collectivités territoriales, leur organisation pédagogique les dispositifs d'accompagnement des élèves, l'affectation des personnels. La location et l'utilisation des moyens. Le recrutement des élèves une contractualisation non pas piloté par le haut encadré corsetée adeptes du copier/coller mais bel et bien initiée par les équipes pédagogiques pour s'adapter aux réalités de chaque établissement, bref le contraire de ce qui a été initié jusqu'alors et qui se poursuit aujourd'hui en effet, Monsieur le Ministre, l'école du futur, l'école, faisons la ensemble le Fonds pédagogique pour l'innovation demeure malgré le discours présidentiel sur l'autonomie marqué au fer rouge du pilotage par l'eau. Ces initiatives sont à leur tour empêtrée par une application restrictive enserré rabougrie parfois même en porte-à-faux avec l'objectif initial en dépit de l'intention sincère de donner plus de souplesse et de sous aux établissements. À l'inverse, l'expérimentation des établissements publics autonomes retournera elle toute sa place tout son sens, tous ces moi hier au projet pédagogique d'un établissement tout en continuant de l'inscrire dans un cadre national qui innerve depuis 2 siècles. Notre système éducatif. L'expérimentation s'appuiera également sur les contrats de mission qui permettront d'aller d'aérer le cas hein. Hier des professeurs de rompre avec leur linéarité. Et donc pour l'institution de soutenir l'envie que beaucoup ont d'innover, de changer. Bref, l'envie de véritablement servir mes chers collègues, nous sommes dans cet hémicycle tous partir sensible à la spécificité des territoires et chacun d'entre nous sait d'expérience qu'aucune école aucun collège. Aucun lycée ne se ressemblent. Qui mieux que le professeur c'est adapté ses enseignements aux élèves. Qui mieux que le directeur le principal ou le proviseur peut définir les besoins de l'établissement dont il a la responsabilité. Voilà l'esprit de cette expérimentation donner une plus grande liberté au collège aux écoles au lycée au directeur au chef d'établissement et aux professeurs c'est incontournable pour promouvoir le mérite et l'égalité des chances. Je sais que le débat clivant et alors l'autre mot elle ce texte apporte un début de réponse et celui de l'acquisition des savoirs fondamentaux, elle vacille parce que l'école s'éparpille le temps effectif de leur enseignement se réduit alors que les programmes se densifie bigarrée d'une multitude d'éducation à de l'institution scolaire, il est désormais moins attendu l'instruction qu'une réponse aux multiples défis sociétaux Pierre Louette de l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètre pas qu'appelait de ses voeux Janzé. Pour répondre à cette baisse du niveau. Je vous propose donc de créer un service public de soutien scolaire et de généraliser l'accès de tous les élèves à des cours de soutien, plus de démarcation entre ceux dont les familles ont les ressources pour payer ses cours et ce qui ne les ont pas le service public de soutien scolaire s'appuiera, entre autres sur des professeurs volontaires, y compris retraités réunis sous la forme d'une réserve éducative. La question de la formation des professeurs doit également être posée enseigner dans le premier ou le son degré, ce n'est pas le même métier, la formation ne peut être identiques. Cette proposition de loi vous propose de dissocier la formation des enseignants du 1er et du second degré. Il ne s'agit pour moi ni de revenir sur la mastérisation, ni sur le lien avec l'université, mais d'arrêter de se payer de mots et de redonner en faire la mère à l'éducation nationale dans la formation des professeurs des écoles en dernier lieu, mes chers collègues, vous le savez. Nous sommes vigilants sur la question de la laïcité. L'école doit oh vous me re-, cet outil de rassemblement fondé sur une stricte laïcité. C'est le sens des dispositions sur la neutralité des accompagnateurs scolaires et sur le port d'une tenue d'établissement, renforçant le sentiment d'appartenance et le vivre ensemble. J'espère que sur ces sujets comme sur les autres nos débats seront à la hauteur des enjeux. Conscient que ce qui se joue dans l'établissement. Loin des postures dogmatiques. Pour terminer je veux saluer très chaleureusement notre rapporteur, Jacques Grosperrin pour son travail et la mise sur pied de ce texte amendé lors de son passage en commission. Mes chers collègues, nous devons certaines pas les mêmes solutions à proposer.

les propositions qui figurent dans ce texte repose sur des convictions fortes et sur une passion immodérée pour l'école de la République. Monsieur Masson, vous faites un rappel au règlement. Madame la présidente, j'avais sous et j'avais demandé la parole tout à l'heure, en application de l'article 44 alinéa 6 du règlement puis je crois que vous ne m'avez pas vu mais je vous remercie madame la présidente de. M'avoir permis de m'exprimer. Lorsque nous avons débattu de ce texte en commission il y a 2 articles qui manifestement ont paru. Les plus importants et qui ont été l'objet du plus grand nombre de d'intervention et surtout des interventions les plus passionnés et je crois que c'est vrai, ce sont les articles sur la laïcité sur les articles fondamentaux de ce texte de loi. Et je suis quand même quelque peu surpris que les deux articles les plus importants étaient été placé à la fin, complètement à la fin du texte. Parce que quand on présente hein. Une proposition de loi, mise à part pour la la loi sur les retraites ou l'article 7 avait été déjà bien décalé par le gouvernement. Mais l'exemple du gouvernement sur les retraites des ne doit pas être repris de deux, c'est je dirais que c'est le mauvais exemple. Mais quand il y a des articles importants, c'est quand même normal qu'on les places en tête des débats et en début de loi et donc. Pour pallier ce problème. Je voudrais en application de l'article 44 Alia aligner à six. Demander une priorité pour les articles 10 et 11 et pour qu'il soit traité en premier. Dans, lors de nos débats. Voilà, madame la présidente. Merci, cher collègue, acte donner de votre rappel au règlement, ce que je vous propose, c'est d'inscrire votre demande de priorité après les prises de parole du rapporteur, Jacques Grosperrin. Et la réponse. L'intervention de de Monsieur le Ministre, si cela vous convient parfaitement. Monsieur le rapporteur. Parole vous est donnée pour. Cinq minutes. madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Ce texte part d'un constat. L'institution scolaire est en souffrance. Nombreux sont nos concitoyens, être inquiet. Un Français sur 2, pense que l'école fonctionne mal et les 2 tiers des Français sont pessimistes sur leur avenir. Cette proportion atteint 80% chez les enseignants, cela traduit un mal-être profond. L'école de la confiance a cédé la place à l'école de la défiance. Pourquoi, parce que l'école n'arrivent pas à atteindre les objectifs que lui assigne la nation. En 1er lieu la France reste l'un des pays où l'origine sociale des élèves conditionne plus leur parcours scolaire. Malgré les moyens importants en faveur de l'éducation prioritaire, les écarts entre les élèves scolarisés en REP ou REP plus et se scolarisés hors de ses réseaux varie peu. La politique sur laquelle est bâti l'éducation prioritaire introduit également une dichotomie des moyens entre les établissements relevant de celle-ci et ceux qui n'en font pas partie. Or, 70% des élèves socialement défavorisés ne sont pas scolarisés en REP. Cela crée parfois un sentiment d'abandon pour tous ces élèves et pour toute la communauté pédagogique concernés. a ailleurs. L'école ne semble plus être capable de transmettre les savoirs fondamentaux. Les élèves français de CM1 sont surreprésentés parmi les élèves européens les plus faibles en mathématiques ou en sciences. Les évaluations intergénérationnel mettent également en lumière une baisse de la maîtrise des savoirs fondamentaux, en 40 ans sur une même dictée. Les élèves de CM2 de 2021 fonds signification. Typiquement plus de fautes que leurs prédécesseurs de 1987.

3ème cause de défiance l'éducation nationale. Elle a du mal à se déployer une politique nationale qui tiennent compte de la diversité des territoires. Le rapport de nos collègues Laurent Lafon et Jean-Yves Roux sur les nouveaux territoires de l'éducation. A mis en lumière l'absence pendant longtemps de la donner. Ruralité dans les statistiques de l'éducation nationale. Cela conduit à une politique scolaire rural par défaut. Or les parcours scolaires poste collègue collège et post-bac d'une partie des jeunes ruraux sont marqués par des écarts à la moyenne, voire des difficultés d'ampleur comparable à celle qui caractérise les élèves de l'éducation prioritaire. Plus d'un Français sur 5 âgés de moins de 20 ans, vit aujourd'hui dans un territoire rural. Monsieur le Ministre. Votre circulaire de rentrée en juin 2022, prône une enquête une école engagés pour l'excellence. L'égalité, elle le bien être mon groupe partagent les mêmes objectifs, les moyens de les atteindre en revanche diverge cette proposition de loi porte notre vision de l'école. Je tiens d'ailleurs à remercier mon cher collègue, Max Brisson. L'auteur de ce texte. Il doit permettre au Sénat de débattre avec vous Monsieur le Ministre et avec l'ensemble des groupes politiques, projet contre projet, de l'avenir de l'école. Les nombreux amendements le montre, l'école est une priorité partagée pour chacun de nos groupes. Ce texte se structure autour de 4 axes. Il souhaite tout d'abord renforcer l'autonomie des établissements scolaires. Aujourd'hui l'uniformité nationale formelle sa commode de larges inégalités réelles de traitement des élèves. La politique éducative centralisé descendante en provenance du ministère n'arrive pas à répondre aux besoins des élèves du territoire. L'article 1er de la proposition de loi ouvrent la voie à une expérimentation. Elle permet aux écoles et aux établissements scolaires volontaires de contractualiser avec le recteur pour accroître leur autonomie. Les collectivités concernées peut faire également partie du contrat. Le texte prévoit pour les écoles qui souhaiteraient participer à cette expérimentation d'acquérir au préalable le statut d'établissement public. C'est pourquoi chacun ici connaît bien sûr le lien fort qui unit la commune à son école, il faudra répondre à l'inquiétude des élus locaux. La commission a rendu nécessaire l'accord préalable des conseils municipaux ou intercommunaux lorsque la compétence scolaire a été transformé avant tout changement de statut de l'école. L'article deux confère au directeur de l'école une autorité hiérarchique sur les enseignants. Notre commission a souhaité illimité ce dispositif aux écoles à partir d'une certaine taille. Le seuil de 9 classe dans l'école me semblait intéressant. Cela concernerait environ 20% des écoles publiques. aujourd'hui des écoles accueillent plus d'élèves que certains collèges dans lequel les chefs d'établissements disposent eux de cette autorité hiérarchique. En revanche, il nous a semblé opportun. À ce stade de conserver pour les écoles plus petites qui ont des équipes qui pédagogiques plus restreinte, la seule autorité fonctionnelle pour les directeurs d'école. J'en profite. Monsieur le Ministre, pour vous demander quand seront publiés les décrets d'application de la Loire, il a Rilhac il y a quelques mois. La proposition de loi vise également assurer l'égalité des chances entre les élèves. Pour cela, elle crée un service public de soutien scolaire qui pourra s'appuyer sur la réserve éducative. Plusieurs amendements de la commission ont permis de préciser les conditions de participation à ce service public. En terme de diplôme de probité et de neutralité. Ce texte renforce la politique éducative en faveur des territoires ruraux plutôt qu'un copier/coller aux écoles et aux établissements scolaires situés dans une zone de revitalisation rurale des dispositifs qui existent en éducation prioritaire nous préférons créer. Des territoires ruraux à besoins éducatifs particuliers. Pourquoi ce choix. La commission parce que les zones de revitalisation rurale sont un dispositif fiscal qui arrive à chez errance fin décembre 2023. Mais parce qu'aussi un déploiement automatique des dispositifs de l'éducation prioritaire dans les territoires ruraux, a peu de sens. Je pense par exemple au dédoublement des classes de grande section au CE1. Au final, comme l'a montré le rapport de Pierre Mathiot et Daria Nabeshima, la principale problématique des élèves des territoires ruraux et celle de l'orientation de l'autocensure et de l'égalité des chances et la poursuite des études plutôt dans le secondaire. Nos collègues Max Brisson Annick Billon, elle m'a écrit Pierre Monnier. Dans leur bilan des mesures éducatives du précédent quinquennat ont montré combien la réforme du lycée été difficile à mettre en place dans les lycées de petite taille. L'article 9 prévoit un accord du conseil municipal avant la fermeture d'une classe dans une commune rurale. Monsieur le Ministre, nous avons entendu vos propos et ceux de la Première ministre et sur une pluriannualité de la carte scolaire et une meilleure concertation avec les élus locaux Ces prévisibilité pluriannuel est demandée par les élus locaux depuis de nombreuses années. La commission de la culture et le Sénat seront particulièrement attentifs à la mise en oeuvre de cette mesure. 3ème axe de ce texte, l'amélioration de la transmission des savoirs fondamentaux, en réformant la formation des s'enseignants du 1er degré. Ce texte propose de transférer à des écoles supérieures du professorat des écoles sous tutelle du Ministre de l'Éducation nationale, la formation des enseignants du premier degré. Enseigner dans le 1er degré, demande des compétences spécifiques en termes de pluridisciplinarité de transmission des savoirs fondamentaux faire classe à des élèves du primaire et différent de faire cours à des collégiens ou à des lycéens. De manière générale, je me réjouis que ce texte soit l'occasion de débattre avec vous des modalités de recrutement et de formation des enseignants. La commission a souhaité sécuriser les jeunes préparant au sein de ses nouvelles écoles au concours d'enseignants du 1er degré et faciliter leur réorientation en cas d'échec. Au concours ou d'abandon de la formation enfin. Le texte souhaite encourager le développement d'un sentiment d'appartenance dans les établissements. C'est un thème cher à notre collègue Céline Boulay-Espéronnier. Il veut également qui a formé l'importance de la laïcité à l'école, notamment lors des sorties scolaires. Celles-ci sont une projection de la classe hors les murs. D'autres thématiques relatives à l'organisation du système scolaire nous paraît importante à débattre dans le cadre de cette proposition de loi. Je pense à la question des jardins d'enfants. Ces derniers peuvent à titre dérogatoire et uniquement jusqu'à la rentrée 2023 2024. Prendre en charge l'instruction des enfants de 3 à 6 ans. Déjà, lors de l'examen de la loi pour une école de la confiance, nous avions protesté sur tous les bancs de cette assemblée contre la fin des jardins d'enfants comme alternative reconnue à la maternelle. Nous ne comprenons toujours pas ce choix du gouvernement. Aussi la commission propose de pérenniser au-delà de la rentrée 2023 2024. Cette possibilité d'instruction des 3 6 ans par des jardins d'enfants qui existait avant l'entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance.

La bivalence offrent de nouvelles perspectives de carrière. Surtout, elle permet de limiter des affectations de personnels, partagés entre plusieurs établissements et une meilleure intégration au sein de l'équipe pédagogique de l'établissement. Mes chers collègues. Ce texte se veut résolument ambitieux afin de changer en profondeur l'école il. Également de la volonté du Sénat de continuer à faire de l'éducation, la première priorité de la nation. Je vous remercie.

Madame la présidente. Monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, monsieur le rapporteur, Jacques Grosperrin. Monsieur le sénateur, Max Brisson. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Cette proposition de loi témoigne de l'intérêt que la chambre haute Marc à la politique publique d'éducation et je tiens à vous en remercier. Votre proposition de loi traite de sujets à la fois structurants et d'une grande actualité pour l'éducation nationale et donc pour l'ensemble de la nation. La gouvernance des écoles et des établissements. La formation des professeurs, l'accompagnement aux apprentissages des élèves. Les conditions de la continuité du service public de l'éducation dans les territoires. Voilà des questions essentielles. Nous partageons de nombreux constats mais nos solutions pourront nous allons le voir, ne pas être les mêmes. Sur la question de l'autonomie des écoles et des établissements d'abord j'observe que votre proposition existe assez largement dans les faits, pour le second degré. En effet, les collèges et les lycées sont des établissements publics autonomes et contractualisent avec l'autorité académique, certes, il en va différemment des écoles qui n'ont pas la personnalité juridique. Pour autant, je ne suis pas certain que nos maires soient prêts à renoncer à cette compétence patrimoniale de l'échelon communal, vieille de près de 200 ans, puisqu'à l'issue puisqu'issu pardon de la loi Guizot du 28 juin 1833. Cette loi imposée aux maires d'entretenir dans leur commune une école et d'y loger un ou plusieurs instituteurs afin d'instruire tous les enfants. J'ai vu que vous avez avancés en commission sur ce sujet et il ne me semble pas opportun en l'état, d'aligner le fonctionnement de nos écoles sur les établissements du second degré. Il ne faut pas je pense laisser croire à nos élus que nous les écartes rions de décisions importantes qui concernent les enfants de leur commune. Au passage je me permets de rappeler mon attachement à faire vivre les communautés éducatives locales via notamment la démarche entreprise par le président de la République dans le cadre du Conseil national de la refondation. Ne vous méprenez pas cependant sur la portée de mon propos, je ne suis nullement en train de vous dire que le gouvernement n'est pas ouvert à une évolution de la gouvernance du 1er degré. En témoigne la Loire Illac de décembre 2021. Mais il faut avancer progressivement. Si l'on souhaite voir prospérer ces réformes pour répondre à votre question monsieur le sénateur, les décrets seront prêts pour la rentrée. Ils ont été soumis aux organisations syndicales, il y a 10 jours, ils passeront au CSA le 16 mai. C'est pourquoi je défends l'autorité fonctionnelle des directeurs d'école qui donne à ces derniers, le rôle de pilote de son école de leur école, tout en conservant l'esprit d'un travail collectif entre tous les professeurs de l'école, c'est un marqueur culturel fort de notre école primaire. De la même façon j'ai engagé avec ma collègue, Sylvie Retailleau Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une réflexion pour que nos professeurs des écoles soient mieux armés et formés pour répondre aux exigences désapprentissage. Là encore, il me semble que nous ne différons pas substantiellement sur l'objectif. J'ai d'ailleurs plusieurs fois. Devant vous, eu l'occasion de m'exprimer en ce sens. Mais je ne saurais souscrire en l'état tout à fait à votre proposition qui risquerait d'écarter les professeurs d'une formation universitaire et de l'obtention du diplôme du master. Quant à l'accompagnement des élèves. Non, là encore, nous partageons l'objectif d'un soutien scolaire à tout élève qui en éprouvent le besoin. C'est dans ce sens que je poursuis la politique entamée par mon prédécesseur et c'est dans ce sens que j'entends conduire la transformation du collège. Aujourd'hui le collège n'est pas suffisamment en capacité de remédier aux principales difficultés scolaires des élèves. De lutter contre les inégalités et de cultiver l'exige l'excellence des élèves. C'est dans ce sens que la classe de 6ème sera transformé l'année prochaine afin que les fragilités des élèves puissent être corrigée. C'est dans ce sens que je rendrai dès la prochaine rentrée scolaire le dispositif devoirs faits obligatoire afin que chaque élève puisse être au-delà des heures de classe soutenu dans ses apprentissages accompagné pour réviser s'entraîner et fixer les acquis vu en classe. Cette égalité des chances, mesdames et messieurs les sénateurs, à laquelle je viens de faire référence doit exister dans tous les territoires, y compris en effet en ruralité. Vous le savez avec la Première ministre lors de notre déplacement dans la Nièvre. Il y a quelques jours nous avons annoncé des mesures qui ne sont pas si éloignés de vos propositions. Mais. Il faut bien avouer que maintenir contre vents et marées et contre la réalité des évolutions démographiques des classes ouvertes. N'est pas pédagogiquement viable. Mon devoir en tant que ministre de l'Éducation nationale et d'assurer l'accès à l'enseignement à tous, partout sur le territoire mais pas à n'importe quelle conditions. Pluri-annualité des moyens instance de dialogue préfet Dasen élus locaux pour coordonner l'action publique valorisation des regroupements intercommunaux pédagogiques sont autant de propositions qu'attendent les territoires, les élus, les parents, les élèves. Et vous j'espère mesdames et messieurs les sénateurs, puisque vous avez souvent évoqué ces questions avec moi. À une solution égalitaire qui consisterait à geler les moyens partout. Nous préférons une solution équitable, équilibrée qui prenne en compte l'éloignement, la qualité d'enseignement. La vie pédagogique en pluri-annualité. Nous devons mettre fin aux incohérences qui oppose l'état dans son rôle d'aménageur du territoire à l'État qui organise l'instruction de nos enfants. Les 2 sont intimement liés car l'école si elle doit être impérativement accessible pour tous nos enfants doit être aussi un lieu de vie pédagogique qui garantit la réussite de nos élèves. C'est pourquoi nous devons mener avec tous les, les acteurs élus, agents de l'État. Un travail de dentelle afin que l'organisation de l'école puisse répondre aux particularités de chacun des territoires. Sur la question de l'application de la loi de 2004 aux parents accompagnateurs. Je ne vous surprendrai pas en vous indiquant que de manière constante. Tous les gouvernements se sont opposés à cette disposition. Je rappelle que les parents en l'occurrence n'agissent pas en qualité d'agent de l'État, le Conseil d'État s'est déjà prolongé prononcé sur ce sujet. Les parents accompagnateurs ne sont pas soumis au principe de neutralité, mais sont bien évidemment interdits de tout prosélytisme. De surcroît, je ne pense pas qu'éloigner les parents de l'école soit souhaitable tout au contraire. Sur l'uniforme et j'en terminerai par là pour que nous puissions échanger et ce sera évidemment avec intérêt et plaisir. C'est une possibilité qui existe déjà en outre-mer les établissements qui l'ont souhaité l'ont inscrit à leur règlement intérieur. Le gouvernement est opposé à une obligation nationale qui ne règle ni le sujet du harcèlement ni les différences sociales et encore moins les atteintes à la laïcité l'uniforme serait immédiatement contourner par différents accessoires. je ne veux donc pas uniformiser les élèves. Je souhaite qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent aux règles de vie, des établissements et au-delà. Aux valeurs et aux principes de la République. C'est par l'instruction. Il la pédagogie. Que notre école y parviendra. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Conformément à l'article 44 alinéa 6 du règlement je suis saisi comme vous l'avez entendu tout à l'heure par monsieur Jean Louis Masson d'une demande de priorité d'examen des articles 10 et 11 afin qu'il soit examiné avant l'article. 1er. Aucune explication de vote n'est admise, quel est l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. je pense que ce texte, le coeur du texte, c'est avant tout. On l'a dit la ruralité c'est la formation des enseignants. C'est l'expérimentation sur l'autonomie des enseignants, c'est le vivre-ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure donc je pense qu'il n'a pas utile. Il faut examiner ce texte avec les articles. À la suite les uns des autres. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis madame la présidente. Je mets donc aux voix. Cette demande de priorité avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Cette demande n'est pas adopté. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à madame Monique de Marco du groupe des écologistes pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe Les Républicains d'abord inscrit à l'ordre du jour cette proposition de loi qui porte sur une institution républicaine capital pour le vivre ensemble. On le sait, l'école est un sujet de clivage politique important et ce texte a le mérite de proposer très clairement une autre vision inspirée de la réforme opérée en 2010 au Royaume-Uni. Et évidemment le consensus sera difficile à trouver. Si nous pouvons rejoindre une partie des constats justifiant cette initiative parlementaire. Nous souhaitons nuancé le regard critique porté sur la performance globale je cite entre guillemets médiocre du système éducatif français. Il faut tout de suite rappeler en effet que les évaluations internationales auxquelles il est fait référence ne porte pas sur l'intégralité des mousses, des missions dévolues à l'école. On les retrouve énumérés à l'article IV et de votre proposition. J'en cite quelques-unes seulement apprentissage d'un socle commun de connaissances, protection de l'environnement enfin. Intégration des élèves en situation d'handicap. Lutte contre les discriminations, prévention de la radicalisation et laïcité laïcité il y a encore, laïcité. On le voit bien, depuis sa fondation. L'école de la République est devenu le rendent pas de tous les maux de la société. Et les enseignants sont la ligne de francs destinés à affronter toutes les crises et ce dans des conditions de travail que l'on connaît. Je rappelle ainsi qu'en 2020, les élèves sont en moyenne 18,4 par enseignant dans l'enseignement primaire en France contre 13,6 dans l'ensemble de l'Union européenne. En remettant en perspective les résultats des enquêtes de comparaisons internationales avec l'ensemble de ses missions. Il y avait des moyens alloués. On peut considérer que nous ne s'en tire pas si mal. Pendant des décennies le métier d'enseignant s'est complexifié sans revers utilisation substantielle de rémunération pour ceux qui l'exercent mais aussi de reconnaissance. Monsieur le Ministre, certaines des déclarations que vous avez fait devant la semaine nationale pourrait considérer avec certaines propositions de nos collègues et les républicains. A lieu. Annualisation ruralité. S'agit-il d'une initiative partagée. Ou un test. Monsieur le Ministre, allez vous inscrire ce texte à l'Assemblée nationale puisque le gouvernement va amender ce texte si qui à mon sens, serait un signe. Après des années blanc coeur il me semble absolument prioritaire de restaurer la la confiance des enseignants dans l'institution. La dépression figurent parmi les premières maladies professionnelle des enseignants. Nous proposions pour cela de créer une communauté enseignante plus du primaire au secondaire, en y associant les AESH. Il faut selon nous multiplier les trajectoires de carrière il améliorer les perspectives professionnelles des personnels de l'audit que si on. Des moins bien traités. Nous souhaitons également discuté de la possibilité d'un système de du tutorat qui permet aux enseignants de tous niveaux et de toutes fonctions d'obtenir un soutien bienveillant tout au long de leur carrière. Après la censure de l'article 40 pour ses à des arrangements. Il ne reste rien de nos propositions et nous ne pouvons que nous opposer par exemple à la création des écoles supérieures du professorat. Je reste donc très opposés au système d'auto d'autonomie des écoles prévus aux articles 1 2 et 3 de la proposition de loi et au système de contractualisation. Qui a dit réinscrire dans ces contrats, que le contrat républicain de donner à chaque enfant une égale de chances d'épanouissement intellectuel. La question de la mixité sociale est insuffisamment traitée. L'existence. Difficultés rural ne sont pas avérés, selon les syndicats enseignants. Je rappelle que dans le secondaire et REP plus concentre les populations les plus défavorisées et ces sujets nécessiterait un véhicule législatif à part entière. Enfin après l'assassinat de Samuel Paty nous semblait essentiel de préserver la vie scolaire en Irak qui vont pas incessamment les polémiques autour du principe de laïcité, nous proposerons la suppression des articles 10 et 11. À l'heure où le ministère n'est pas en mesure de garantir des remplacements d'assurer des recrutements ni de formation continue de qualité qui répondent aux besoins des personnels. Quel est le sens d'un tel projet. En conclusion, cette proposition de loi qui oublie nos langues régionales. Menace le faible équilibres de l'éducation nationale accélérer la privatisation aurait un coût considérable à la charge des familles. Elle creuserait les inégalités entre établissements. Parce que nous souhaitons une école coopératives et citoyenne. Un service public juste et accueillant pour toutes et tous, nous voterons pas cette proposition de loi, je vous remercie. La parole est à présent à notre collègue monsieur Julien Bargeton du groupe RDPI et vous avez six minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le président de la Commission, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Alors quand on fait une proposition de loi au Sénat, en général on a 2 choix. On fait une proposition de loi qu'on espère mener à bout. Consensuel vous avec des positions possibilité de convergence. Alors là on aurait pu faire par exemple une loi sur les écoles de la ruralité ou une loi sur la formation des enseignants. Où il y a un 2ème choix celui que vous avez retenu, qui est de faire une proposition de loi vaste qui retranscrit un programme politique c'est noble, c'est. Mais vous savez qu'elle ne prospère rapa. Vous savez qu'elle ne prospère rapa vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, c'est une proposition de loi qui se veut clivante. Vous avez annoncé la couleur, si j'ose dire, à partir de là évidemment elles ouvrent beaucoup de choses mais comme elle ouvre beaucoup de choses sur l'école, mais partout et ben il y a eu plein d'amendements sur Parcoursup, les AESH. La formation continue de nos, nos collègues de l'Union centriste de l'éducation sexuelle à l'école. Évidemment puisque c'est une et une loi qui prétend embrasser l'ensemble mais qui ne le fait pas et donc ça ouvrait la porte à ceux-là c'est un peu dommage, je pense qu'on aurait pu avancer ensemble sur certains sujets précis. Du coup, elle a aussi pour conséquence de revenir sur certains débats récents hein donc elle revient. Ça a été dit sur la neutralité pour les accompagnants scolaires sur également l'enseignement en famille et puis également sur le port de l'uniforme à l'école. Je note d'ailleurs que l'Union centriste. Une proposition de loi d'une collègue d'Union centriste visant supprimer. Cet article, c'est bien que là aussi vous avez tellement cliver que finalement vous avez cliver aussi au sein de la majorité sénatoriale. L'autre conséquence de cette loi, c'est que du coup alors que vous êtes parfois critique là-dessus, elle n'attend pas les évaluations ou les concertations pour procéder à des propositions or parfois le Sénat dit ben il faudrait quand même d'abord évaluer les dispositifs et concertée. C'est le cas par exemple sur l'autorité fonctionnelle de l'avoir il a qui qu'on vient de voter ou sur l'autonomie. Il y a une expérimentation en cours et l'autonomie pédagogique, l'établissement il y a. Il y a une expérimentation à Marseille on pourrait attendre. Bah, d'avoir un peu les résultats du lancement de ses propositions avant de d'y, d'y revenir. Et d'ailleurs notre rapporteur dans sa sagesse s'est senti obligé de restreindre légèrement les dispositifs dans les 2 cas puisqu'il a restreint l'autorité fonctionnelle à certaines écoles et qu'il a également restreint. La l'autonomie. En en prévoyant parce qu'il avait été oublié peut-être d'associer quand même davantage les élus locaux, ce qui prouve bien là aussi que c'est une loi qui veut peut être trop trop embrasser et puis elle arrive dans un timing particulier. Le ministre l'a dit il y a un plan qui a annoncé sur les écoles rurales et ça il y a aussi le Sénat qui a lancé une mission d'information sur l'autonomie des établissements. Peut-être aurait-il fallu attendre que il y ait vous êtes dans cette mission d'information donc vous auriez pu attendre vous-même les conclusions de vos propres. De vos propres travaux. On a l'impression quand même que cette proposition de loi cherche à préempter jalons après Jâlons tous les sujets et d'une façon même s'il y a des choses intéressantes parfois précipités et un peu brutal pour employer les termes et puis elle ne répond pas à son objet. Vous dites que ces lois vont pour la liberté, égalité des chances. Il y a quand même peu de dispositifs sur l'égalité des chances, où est la mixité sociale dans ce texte ou hé oui il y a il y a un article sur le soutien scolaire et d'ailleurs j'ai. Nous ferons des propositions. C'est un sujet intéressant. Mais au-delà de ça, la mixité sociale dans l'urbain. Vous avez fait le rural mais du coup ben non vous avez pas fait l'urbain et cetera et cetera donc finalement et il y a d'autres sujets qui ne font pas abordé le privé et nos collègues du coup dépose une série d'amendements qui viennent montrer finalement que. Elle ne correspond pas à son objet. Je voudrais juste rappeler quand même si si je ne le fait pas, vous m'en voudriez parce que personne ne le ferait que le dédoublement de classes dans les repérer plus en CP et se hein. Ces 300.000 élèves et que ça va atteindre grandes sections de maternelle. Le système devoirs faits ah les résultats. C'est 10,10 points d'amélioration sur les mathématiques et le français dans les zones concernées, l'école. L'école inclusive 430.000 élèves porteurs de handicap contre 320.000 au début 2017 les cordées de la réussite. 200.000 élèves sont ainsi accompagnées de la 4ème à la terminale. Bref, il faut quand même aussi rappeler un certain nombre de dispositifs. Ce qui n'empêche pas de les de les compléter et de proposer des améliorations mais il est bon aussi de repartir de de ce qui existe, ces propositions de loi, elle a une vocation politique d'ouvrir un débat je dirais parfois d'ouvrir des polémiques alors que je pense que l'école mérite de la confiance et de l'efficacité. C'est dans ce sens que nous entrerons dans le débat. Vous avez voulu en faire un sujet clivant. Il faudrait aussi se dire comment ce débat peut faire de l'école un lieu de rassemblement. Merci beaucoup. Merci la parole est à présent à notre collègue Madame Marie-Pierre Monnier du groupe socialiste pour 9 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 10 avril 1870 le Ferry prononcer les mots suivants dans l'enceinte du Palais Bourbon. Ma prétention et de vous montrer que l'égalité d'éducation n'est pas une auto pis. Que c'est un principe qu'en droit, elle est incontestable et qu'en pratique, cette utopie apparente et dans l'ordre des choses possibles. C'est d'abord à cette exigence d'égalité, que nous devons nous attacher quand nous évoquant l'école de la République, pas à celle de la performance trop souvent porté aux nues comme si l'école était une entreprise. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est un condensé des propositions mises en avant par la droite depuis des décennies pour transformer une institution qu'elle estime défaillante, autonomie des établissements scolaires renforcer jusqu'à l'extrême autorité hiérarchique, les directeurs d'école remise en cause du Cadre de la fonction publique pour les recrutements enseignants uniforme obligatoire. Je souhaite en 1er lieu rappeler que loin des discours à la mise sur le sujet. La dernière étude de l'Insee publiée en 2022, établie à 74% le niveau de confiance de la population dans l'institution scolaire. Bien sûr, tout ne va pas bien, mais nous considérons pour notre part que ce dans notre école a besoin c'est de moyens à la hauteur pour fonctionner dans de bonnes conditions et non pas de telles mesures qui ont vocation à la faire basculer dans une logique libérale et concurrentielle, bien loin des principes républicains. J'entends déjà mes collègues du côté droit de cet hémicycle me répondre que des moyens on en donne déjà bien assez mais je souhaiterais à ce titre partagé quelques éléments de comparaison à l'échelle européenne. D'abord dans son rapport consacré à l'Europe de l'éducation, publié en décembre 2022. La direction de l'évaluation de la prospective et de la performance pointe que la France est le pays de l'Union européenne, dont les effectifs par classe sont les plus élevés. Les élèves scolarisés en élémentaire en France sont en moyenne 22 par classe contre 19,3 dans le reste de l'UE. Au collège, l'effectif moyen approche 26 élèves alors que la moyenne européenne est situé sous la barre des 21. La France est aussi l'un des pays de l'UE où les enseignants doivent assurer un nombre d'heures de cours. Parmi les plus élevés. Et ce alors que leur salaire est inférieur à la moyenne européenne. L'évolution de nos dépenses en matière d'éducation mérite également d'être scruté avec plus d'attention dans un contexte où l'on entend dire et qu'elle serait un puissant fond la dépense intérieure de l'éducation a atteint un pic de 7, 7 du PIB au milieu des années 90, elle évolue aujourd'hui de moyenne. En moyenne autour de 7% de. Mais depuis les années 80, l'État s'est progressivement désengagé des dépenses au profit des collectivités territoriales, dont la part dans les dépenses d'éducation est passée de 14 100 100.981 23 % en 2021. J'ajoute que quitte à nous poser des questions sur l'efficacité du budget alloué à l'éducation nationale nous pourrions nous interroger sur les sommes attribuées spécifiquement l'enseignement privé sous contrat, financé à 73% par de l'argent public est-il bien normal que dans une ville comme Paris. Les établissements privés disposent de plus d'heures d'enseignement rapportées au nombre d'élèves que leurs homologues du public. Pour en revenir au détail des articles que contient ce texte plusieurs constitue pour notre groupe. Une ligne rouge. Nous aurons à coeur de défendre tout au long de cet examen leur suppression l'article. Qui prévoit l'expérimentation d'une autonomie renforcée des établissements scolaires du 1er et second degré. Va à l'encontre de notre vision républicaine de l'école qui doit être la même pour tous les élèves sur l'ensemble du territoire et répondre au même programme c'est objectif le cadre expérimental dans lequel il s'inscrit et par ailleurs fragile juridiquement, il ne me semble pas possible que les établissements publics autonomes de l'éducation soit créé pour une durée temporaire. Article 2 instaure une autorité hiérarchique pour les directeurs d'école certes circonscrit suivant le nombre de classes à la suite de l'examen en commission. Nous avions déjà eu l'occasion de l'affirmer. Lors de l'examen de la loi Rilhac. Nous sommes attachés au fonctionnement collégial des écoles du 1er degré, celui des pères parmi les pères. Nous reviendrons d'ailleurs par voie d'amendement sur la notion d'autorité fonctionnelle voter alors qu'il introduit une première brèche sur le sujet. La mise en place des contrats de mission entre recteurs et enseignants proposée à l'article 3 s'inscrit dans un cadre dérogatoire au droit commun de la fonction publique qui n'est pas acceptable. qui impactera l'ensemble du ben scènes de recrutement bien au-delà des seuls établissements concernés et ne résoudra d'ailleurs en rien le manque d'attractivité de certains établissements ont certains territoires. L'article 10 étant le principe de neutralité et l'interdiction du port ostensible de signes religieux aux participants occasionnels du service public de l'éducation. Mon groupe s'est toujours opposé à une telle extension de ses obligations aux accompagnateurs et accompagnatrices de sorties scolaires. J'ajouterai que le sujet de la laïcité à l'école mérite une autre approche visant une meilleure appropriation et adhésion de nos élèves à ce principe fondamental. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre de la formation des enseignants. D'autres dispositions de ce texte moins clivante ont le mérite de soulever des problématiques pertinente. Même si nos différents parfois sur les réponses apportées. Ainsi, nous considérons que la formation initiale des enseignants du premier degré peut être revue et améliorée dans son déroulement. Il ne nous semble pas opportun de mettre fin à la culture professionnelle commune. Entre 1er et second degré que permettent les spé. Et et l'eau et d'éloigner la formation des enseignants du premier degré du monde universitaire et de la recherche. L'article 6 pose les jalons d'un service public de soutien scolaire. C'est un signal positif qui répond à un besoin social fort qui ne peut être laissée à la main du privé. Nous aurions souhaité l'encadrer davantage afin de garantir la qualité de la l'accompagnement proposées aux élèves au regard des exigences et de la continuité dans les apprentissages nécessaires. Nous considérons en effet qu'il doit être pour le second degré assurée uniquement par des professeurs et ce en l'intégrant à leurs heures de service nos amendements en ce sens ont malheureusement été jugée irrecevable en raison des charges supplémentaires engendrés. Il est vrai que tout bon service public nécessite un investissement de la part de l'État. L'article 7 qui prévoit la mise en place d'une réserve éducative pour nourrir ce service public nous paraît redondant par rapport à la réserve citoyenne de l'éducation nationale déjà existantes tant il conviendrait plutôt de dresser le bilan. L'article 8, fortement remanié en commission interroges sur les difficultés propres aux élèves scolarisés en milieu rural. Six son périmètre et sa portée sont devenues floues, il a le mérite d'aborder un sujet rarement évoqué et pourtant cruciale. Nous partageons les la préoccupation exprimée par l'article 10 dans l'ensemble de nos territoires ruraux les alertes se sont multipliées concernant les fermetures de classes prévues à la prochaine rentrée. Dans la Drôme ne comptant plus de 40 fermetures de classes et les plus douloureuses dans les communes rurales. Je ne peux que rejoindre mes collègues qui regrette ces fermetures en raison de l'application d'une logique purement purement comptable, je le répète, les choix faits au PLF ont des conséquences. J'espère pouvoir donc compter sur eux lors du prochain vote pour revenir sur les suppressions de postes enseignants opéré ces dernières années en ce qui concerne l'article 11 qui prévoit l'obligation d'une tenue vestimentaire uniforme. Nous considérons que, qu'il n'est pas la bonne réponse à apporter aux inégalités sociales et scolaires. Si nous souhaitons nous attaquer sincèrement à ces sujets, la mixité sociale constitue la vraie porte d'entrée si je me réjouis toujours de l'opportunité d'un temps de débat au sein de notre hémicycle sur l'école. Ce texte me laisse toutefois un goût amer car il me semble que ces propositions ne sont pas à la hauteur des enjeux auxquels est aujourd'hui confrontée notre école de la République, pourtant essentiel pour nos enfants et l'avenir de notre pays, si nous souhaitons réellement être dans une approche moins vertical et plus proche du terrain. Nous devrions en 1er lieu écouter les préoccupations des personnels qui s'efforce de la faire vivre au quotidien. La parole est à présent à madame Céline Brulin, du groupe communiste pour cinq minutes, chers collègues. Si Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le seul et maigre mérite de cette proposition de loi et de montrer que de véritable projet de société sous-tendent la vision de l'école dans notre pays, pour notre part, nous portons une vision clairement de gauche, celle d'une école ayant pour l'objectif, l'égalité des chances et la justice sociale. Celle d'une école qui offrent le plus haut niveau de connaissances à des enfants qui deviendront ainsi quel que soit leur parcours ultérieur des citoyens et des travailleurs conscients et responsables. Celle d'une école qui apporte plus à ceux dont le Patrimoine culturel est moindre, ce qui est intrinsèquement lié à la condition sociale. Et le temps n'émousse pas cette conviction, au contraire. Face aux bouleversements technologiques et scientifiques qui peut résumer l'éducation un socle minimal de connaissance. Face aux enjeux démocratiques qui peut raisonnablement considérer que nos jeunes doivent être plus formés à l'obéissance qu'apprendre à développer leur esprit critique et leur capacité à se forger une opinion solide éclairée par l'histoire, par exemple, hé bien les auteurs de cette proposition de loi dont la vision est clairement de droite et même réactionnaire la blouse devenant l'uniforme. L'Autorité devenant hiérarchique le recentrage sur le lire écrire compter frappant jusqu'à la formation des enseignants. La main invisible du marché. Son cortège de concurrence et l'idée selon laquelle seuls ceux qui seraient privés serait efficace on également pris toute leur place dans cette proposition de loi mais mes chers collègues, vous n'êtes pas à une contradiction près, car votre proposition consiste de fait a créé une forme de séparatisme, alors qu'il faudrait renforcer l'école de la République. De même. Vous dites vouloir libérer les énergies. Si c'était les innovations alors que vous vous acharnez à encadrer les pratiques professionnelles des enseignants jusque dans les moindres détails, même à titre expérimental la contre à. La contractualisation que vous envisagez conduirait inévitablement à une école à la carte d'un service public national motivée par une obligation de manque de moyens alloués par l'État nous bascule yeux nous basque le rayon Vert une myriade d'école sur le modèle des écoles privées soumises à des objectifs particuliers qui conditionnerait programme moyen horaire et recrutement des enseignants a sorti de votre obsession d'une réduction massive de la dépense publique alors qu'il faut considérer l'éducation comme un investissement dans l'avenir. Cela ne pourrait conduire qu'à une mise en concurrence des établissements, ainsi que des disciplines. Mais la France ne veut pas plus d'école à la carte que de République à la carte contradiction toujours vous écarter la question des moyens comme réponse au besoin de renforcer l'école de la République en pointant par exemple l'éducation prioritaire pour finalement la revendiquer en ruralité. Ou alors vous considérez que les sorties scolaires. Ce sont des temps de classe hors les murs au seul motif de contrecarrer la liberté religieuse des parents de confession musulmane. Pour les autres, cela vous gêne beaucoup moins mais vous refusez systématiquement nos propositions pour qu'à ce même titre elle soit encadrés par des personnels pédagogiques et en même temps plutôt que de faire du soutien scolaire, un objectif de l'éducation nationale avec des moyens de rattrapage des dispositifs individualisé, vous en, vous entendez le laisser dans les mains d'une réserve éducative inévitablement cette mission pèserait sur les collectivités territoriales, tout particulièrement celles qui parce que leurs habitants rencontrent davantage de difficultés sociales, culturelles et scolaires en font déjà beaucoup plus que d'autres en matière éducative vous prétendus remèdes sont finalement pire que le mal. Depuis 1989, l'autonomie des établissements publics locaux d'enseignement ne cesse de croître. Cela a-t-il permis de résorber les inégalités. Absolument pas. La plus récente réforme celle du lycée conduite au nom de cette volonté d'offrir des marges de choix et de la liberté les renforce au contraire vous le savez-vous qui comme moi avaient dans vos départements des lycées offrant tous les enseignements de spécialité ou presque quand d'autres se contentent du minimum, les uns étant plutôt. Dans l'hypercentre des grandes métropoles, les autres se trouvant plutôt dans les quartiers populaires et les zones rurales. Pensez-vous vraiment que c'est en faisant porter la responsabilité de l'ensemble de la de de l'institution sur les agents de première ligne qu'on parviendra à faire face à la crise de recrutement des enseignants que que nous connaissons aujourd'hui poser la question, c'est y répondre. Quant au contrat de mission censée amener les enseignants les plus expérimentés dans les zones les plus difficiles. Leur échec risque d'être aussi pas tant que celui du dispositif Éclair. D'autant que le mouvement mais à force d'un autant conclure le chocolat et un réseau de lui non plus. Cette proposition de loi est dangereuse et nous la combattrons comme il se doit. La parole est à présent à notre collègue Madame la Présidente Annick Billon du groupe Union centriste pour huit minutes. On va baisser. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Je voudrais tout d'abord remercier l'auteur du texte, Max Brisson. Jacques Grosperrin également le rapporteur pour le travail précis et riche qui nous donne l'occasion d'avoir un débat de fond sur l'éducation. Ce texte témoigne toute l'attention que vous portez que nous portons à l'éducation nationale et la volonté d'élever notre école, nos élèves nos enseignants. Nous en avons besoin. En effet, alors que les dépenses en matière d'éducation sont supérieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Le système éducatif français peinent à produire des résultats satisfaisants. L'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social. L'école ne lisent plus ne codirige plus les inégalités. Pire les creuse parfois. Sur le niveau des élèves. L'étude internationale teams 2019 permet de constater que les élèves français de CM1 sont sur-représentés parmi les élèves européens les plus faibles. Au lieu de 25% attendus dans le quartier inférieurs, ils sont 45% en mathématiques et 41% ancien. 15% des élèves français soit un sur 7 ne maîtrisent pas les compétences élémentaires en mathématiques alors qu'ils sont seulement 6% au niveau européen. En janvier 2023, la Cour des comptes publié un rapport mobiliser la communauté éducative autour du projet d'établissement. Des égalités du système éducatif. Les rapports sur la mixité scolaire dans les établissements, tout comme les analyses des résultats aux examens nationaux démontre à quel point l'univers n'uniformité nationale peut s'accommoder de larges Zine égalité le silence soudain m'a perturbé. Le brouhaha finalement été utile tout à l'heure. Merci l'institution scolaire est en souffrance et de nombreuses interrogations persistent sur sa capacité à répondre aux objectifs qui lui sont assignées. Selon le rapport de notre collègue Jacques Grosperrin. Plus d'un Français sur 2 et 3 enseignants sur 4 pensent que l'école fonctionne mal. 2 Français sur 3 et 8 enseignants sur 10 sont pessimistes sur l'avenir de l'école. Lors de d'autres rapports sur le bilan des mesures éducatives du quinquennat avec mes colères, mes collègues Marie-Pierre Monnier et Max Brisson. Nous avions déjà tiré le signal d'alarme. Notamment sur la crise d'attractivité que connaît le métier d'enseignant appelé il y a encore quelques années. Le plus beau métier du monde. Lorsque nous avions rendu nos conclusions près d'un enseignant sur quatre se demandait s'il n'aurait pas dû choisir une autre orientation professionnelle. Le constat est rude et le texte que nous imaginons d'examinons aujourd'hui se veut une réponse à cette problématique. Il propose de faire évoluer les dispositions sur de nombreux sujets avec pour objectif sinon pour ambition de résoudre les difficultés de l'école et donner plus de liberté aux équipes éducatives. Par exemple il propose que l'autorité fonctionnelle des directeurs d'établissements de plus d'un certain nombre de classes trop soit transformée en autorité hiérarchique. Cela permettrait à l'école de mieux s'adapter à ses besoins spécifiques. Les contrats de mission proposée à l'article 3 du texte permettre aux enseignants de donner plus de souplesse à l'heure où à l'heure avec un S affectation et de permettre aux établissements de répondre à des besoins qui leur sont précis. La formation des enseignants est également abordé la PPL prévoit de séparer la formation des professeurs du second degré de celle de leurs collègues du 1er degré. Ceci afin de mieux préparer ces derniers aux apprentissage des savoirs fondamentaux. Nous saluons également l'amélioration et la meilleure prise en compte des collectivités territoriales avec la redéfinition de leur rôle dans l'élaboration des politiques relatives à l'éducation prioritaire. Certains territoires ruraux particulièrement en zone isolée ou subissant une crise industrielle ou post-industriel voit se cumuler des difficultés sociales qui peuvent avoir des effets et sur le, ce Ces difficultés ont été renforcés par la crise sanitaire que nous avons traversé ce sont des territoires à besoins spécifiques aussi. Nous saluons la création par le rapporteur de territoires ruraux à besoins éducatifs particuliers. Cette revendication était d'ailleurs porté par notre commission depuis plusieurs années. Le rôle des collectivités locales est également réaffirmé à l'article 9 du texte. Celui-ci propose une co-réflexion lorsque des fermetures de classes doivent intervenir dans les territoires. Nous nous réjouissons des améliorations apportées en commission sur ce texte. Nous avons notamment proposé qu'une condition de diplôme soit ajoutée aux conditions de recrutement des personnels qui formeront la réserve éducatif le niveau Baccalauréat sera requis. Nous avons par ailleurs souhaité renforcer le dispositif de formation des professeurs du 1er degré. Afin qu'elles soient alignées sur la formation des professeurs confesseur du second degré. De même, nous souhaitons que les étudiants bénéficient comme leurs homologues d'actions de formation complétant leur formation initiale. Le modèle des jardins d'enfants va perdurer grâce à un amendement notamment porté par le président Hervé Marseille supprimant les dispositions de la loi de l'école de de la confiance. Enfin, nous avons renforcé le rôle des collectivités locales en modifiant l'article 9 du texte en transformant le moratoire de un an. Initialement prévu à en une période de 3 ans pendant laquelle aucune fermeture de classe ne pourra intervenir si les conseil municipal se prononce lors d'un vote contre la fermeture de classe. Pour la séance, nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 11 qui concerne le port de l'uniforme. Dans les établissements scolaires. La majorité du groupe n'est pas favorable à une telle disposition. L'uniforme est souvent présenté comme l'un des deux leviers à activer en réponse aux inégalités sociales et pour favoriser la mixité scolaire. Or, aucune étude ne vient confirmer ce postulat. Si vous me permettez le port de l'uniforme n'est pas forcément la réponse à la bonne tenue de notre école. Le groupe Union centriste et dans sa majorité opposés à ce dispositif. Mes chers collègues, convaincu de l'importance de ce texte, le groupe Union centriste votera donc en sa faveur. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Madame. Esther Benbassa, des non inscrits pour 3 minutes, chers collègues. Deuxième fois oui. Oui, c'est la journée. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, aujourd'hui nous discutons d'une proposition de loi issu comme vous l'avez compris de la droite sénatoriale pour une école de la liberté de l'égalité des chances et de la laïcité. Si l'intitulé semble être. Porteur d'espoir et de renouveau. Le contenu, l'est moins. Ainsi, dès le 1er article, le ton est donné. Il est proposé d'accroître l'autonomie des établissements scolaires sous contrat qui aurait désormais la possibilité de recruter leurs élèves de choisir leur engagement, leur organisation pédagogique et de donner une liberté quasi totale au directeur de l'établissement. Avec ce mode de sélection des élèves vous réduisez leurs chances à certains d'accéder à les tiens. L'établissement scolaire de leur choix. Par ailleurs, les inégalités entre élèves ne cesse de s'aggraver le poids de l'origine sociale se se reflète inévitablement dans les résultats scolaires. Le système éducatif français ne parvient plus à prendre en charge les élèves les plus faibles. Selon la dernière enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves d'Air France est un des pays de l'OCDE qui affiche un très grand écart de réussite entre les enfants les plus défavorisés et ceux issus des familles les plus aisées et surtout éduquer c'est un chantier sur lequel il est urgent de travailler et pourtant les mesures proposées sont insuffisantes et ne semble pas répondre à cet impératif de réduction des inégalités scolaires de surcroît le texte, texte d'autres marqueurs indélébiles dans le de la droite. Comme l'interdiction du port du port du voile pour les accompagnatrices scolaires à l'Arctique neuve et le port obligatoire de l'uniforme à l'article 10, encore une fois le principe de la laïcité déformé aujourd'hui la laïcité seraient menacés partout en France et l'école en grave danger, que ce soit dans les assiettes à la cantine lors des sorties scolaires dans les cours de récré ou encore à la piscine. Tout prétexte c'est bon pour le définir le principe de laïcité à sa sauce et encourager le marché électoral qui est le vote de l'islamophobie cette stigmatisation permanente ne fait que renforcer le repli communautaire. C'est un engrenage vicieux que l'éducation nationale devrait endiguer à force de pédagogie de formation à la laïcité de dialogue, professeurs, élèves et professeurs, parents. Emmanuel Macron a déclaré le 16 mars dernier qu'il ferait de l'école sa priorité et faire de sorte que l'école soit ouverte à tous, émancipatrice libératrice inclusive ce texte ne répond visiblement pas à cette ambition, je voterai contre pour un texte qui fait des clins d'yeux à l'extrême droite et dans le contenu et sur l'année. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur le sénateur. Bernard Fiolet du groupe RDSE. Et vous avez 5 minutes chers collègues pour vous exprimer. Rebonsoir. Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président, monsieur l'auteur de cette proposition. Pourquoi la république n'est plus perçue comme l'idéal qui fait rêver. Parce que la promesse républicaine n'est pas tenu aussi, ne nous étonnons pas que certains se tournent vers d'autres promesses et cède aux emprise idéologique qui leur sont proposés. Monsieur le Ministre ici même devant vous il y a un mois je rappelais les voeux du président de la République. La principale injustice qui mine notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale et la réponse se trouve dans l'école. Vous nous aviez annoncé pour fin mars de nouvelles dispositions d'affectation des élèves plus équitable entre écoles publiques et privées. Qu'en est-il aujourd'hui. Cette proposition de loi pour une école de la liberté de l'égalité des chances et de la laïcité est une interpellation forte au constat accablant du modèle et de éducatif français. Classements internationaux catastrophique. Crise de recrutement des enseignants. À l'image des déserts médicaux. Il ne faudrait pas voir se développer des déserts de République des zones de non-droit. Les vérités scientifiques sont contestés par des croyances révélé les principes de la République sont ignorées et la laïcité bafouée. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader ce pan essentiel de notre société dont les ressources humaines sont la principale richesse. L'éducation devrait être la priorité de nos investissements. À quoi bon vouloir relocaliser réindustrialiser investir sans ressources humaines à hauteur et épanouie. Il faut également rétablir de l'autorité. Une autorité scientifique, indiscutable une autorité morale affirmé et comme marqueur. L'autorité de compétence des maîtres qui enseignent sous l'autorité des directeurs, chefs d'établissement. Cette absence de hiérarchie est des. De l'école publique par rapport à l'école privée. De nom de l'autonomie aux établissements. L'égalité n'a jamais été l'UNICEF Formister ni l'unicité. Elle est au contraire l'adaptation au terrain et aux circonstances et doit pour cela associer les collectivités locales, mairies, bien sûr, mais aussi les services médico-sociaux des départements, les régions pour l'orientation, les parents d'élèves et l'éducation nationale avec l'école comme chef de file. L'expérimentation d'établissements publics autonomes d'éducation va dans ce sens. Comme la réserve éducative proposées. Le périscolaire telle qu'il a été reçu comme une contrainte précipitée par nombre de collectivités n'est pas partout à la hauteur de l'enjeu majeur que constitue le temps d'accompagnement des enfants qui ne doivent pas être livrées aux réseaux sociaux au désoeuvrement avec les risques auxquels on les expose. L'encadrement des enfants par une communauté éducative doit être renforcée. Combien de parents font le choix de l'enseignement privé à cause de l'absentéisme non remplacés. Les enseignants doivent être soutenus respecter. Financièrement et socialement. Comme dit Jacques Perrin faire classe dans le primaire, ce n'est pas la même chose que faire cours dans le secondaire. Il faut une formation spécifique et adapté. Les écoles supérieures des professeurs des écoles qui nous sont propres poser pour succéder aux aux Inspé qui succédait déjà aux SP qui succédait aux IUFM ne serait-elle pas que nos regretté École normale alors, appelons un chat un chat et revenons aux écoles normales, auquel d'ailleurs le président de la République ne serait pas hostile. Pour enseigner les fondamentaux et affirmé les vérités scientifiques qui ne peuvent plus être contestée ou menacés ainsi que ceux qui les professent. Jean Pierre Houdin dans une enquête récente révèle que 50% des enseignants et particulièrement les plus jeunes s'autocensurent. Devant les menaces et les craintes de représailles. L'humilité du savoir est vécue comme une faiblesse par ceux qui le contestent. Ne cédons rien sur la laïcité. Ces principes et sur la neutralité qu'elle exige aussi bien sur les tenues vestimentaires des enseignants, des élèves que des accompagnants scolaires. Si la proposition d'uniformes d'école nous semble excessive. Elle réaffirme cependant qu'aucune culture aucune expression religieuse ne peut porter atteinte à l'émancipation et à la liberté des femmes par exemple. Le curé l'imam ou le rabbin ne peuvent remplacer l'instituteur et je suis heureux que nous partagions enfin tous cette affirmation de l'école de la République. Il enfin revoir la participation des communes au financement des écoles privées. Dans le contexte d'augmentation des charges de coût de l'énergie comme des salaires, une baisse d'effectifs d'une école pour cause démographique ou de mutation d'élèves dans le privé, renchérit automatiquement la participation des communes. Elle divise leurs coûts fixes par un nombre moins d'élèves et abonde ainsi les ressources de leur concurrence. Cela rend tout nouvel investissement supplémentaire d'ailleurs encore plus pénalisant. Les charges devraient être divisée par le nombre de places potentielles et non par le nombre d'élèves. Effectif. Je vous ai déjà alerté sur ce sujet, Monsieur le Ministre. Soutient ce cri d'alerte que nous vous adressons pour rétablir l'excellence de l'école de la République. Chers collègues. La parole est à présent à madame Céline boulet espère rogner du groupe les républicains. Et vous avez 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Plus que jamais, l'éducation et le pilier fondamental de notre société. Le système éducatif français fournit un apprentissage de qualité à des millions d'élèves chaque année. Malgré cela, la crise de l'école est un constat qui ne fait plus débat. Perte de confiance des familles et des élèves, manque de soutien auprès des personnels de l'Éducation nationale. Crise d'attractivité du métier d'enseignant. Baisse du sentiment d'appartenance. Autant de manifestations d'une institution affaiblie qui peinent à trouver un nouveau souffle. Il est clair que nous devons renforcer l'école davantage d'autonomie pour les établissements scolaires permettrait de mieux répondre aux besoins et aux attentes des élèves, des parents et des enseignants. Cela favoriserait l'innovation et l'expérimentation pédagogique en donnant des établissements davantage de latitude pour adapter les méthodes d'enseignement aux caractéristiques de leurs élèves et à leurs contextes spécifiques. Telle est l'objectif de la proposition de loi de notre collègue Max Brisson. Un objectif que nous partageons sans réserve. Je souhaite remercier chaleureusement le rapporteur, Jacques Grosperrin pour l'ensemble du travail réalisé. À l'heure où l'intégration des nouveaux outils technologiques. L'influence des réseaux sociaux viennent bouleverser les rapports à l'apprentissage et à la transmission des savoirs. Je suis convaincu que nous devons concentrer nos efforts pour contribuer à améliorer l'égalité des chances. Les mots, respect, autorité fierté d'appartenance altruisme ne sont pas des mots désuets. Il est temps de re sanctuariser l'école autour de ses valeurs. Il est temps de recentrer l'école sur les savoirs fondamentaux dont le 1er et le savoir-être avec pragmatisme et loin des positions idéologiques. Concernant l'article 11 de la proposition de loi visant à rendre obligatoire la tenue d'établissements scolaires. Je crois qu'il est temps de réévaluer le rôle de cette dernière dans l'éducation et de la considérer sous un nouveau jour dans l'école de 2023. Ce serait même un gage de modernité et d'efficacité et je vais m'en expliquer. Je vous précise que nous avons choisi le terme d'établissements plutôt que celui d'uniforme car ils mettent en avant l'autonomie des établissements, dans la mise en application de cette obligation, elle sera réalisée en concertation avec les parents, la communauté éducative et les élèves en fonction des particularités géographiques sociales et économiques locales en somme les spécificités des territoires. Si cette question a suscité beaucoup de débats en métropole. Ces dernières années. Je précise que les partisans de la tenue d'établissement à l'école républicaine sont majoritaires en France. En effet, un sondage CSA diffusé le 12 janvier 2023 évoquent 60% des Français sont pour. D'ailleurs elle a fait ses preuves dans les outre-mer. La tenue d'établissements permet de renforcer l'entraide et le sentiment d'appartenance. Pourquoi ce qui fonctionne dans le cas d'une association ou d'une équipe sportive ne fonctionnerait pas à plus grande échelle. Par ailleurs, elle sera un moyen de préparer les élèves à la vie professionnelle. L'enfant qui franchit le seuil de son école devient un élève, et entre dans une situation de travail. La tenue comme dans d'autres professions, aide au respect des règles. En matière de sécurité, ce qui est à prendre en compte elle minimise le risque d'éventuelle intrusion dans l'enceinte des établissements. Par ailleurs, la tenue d'établissement scolaire permet d'évacuer la question du port de signes ostensibles d'appartenance religieuse ou communautaire assurant une pleine application du principe de laïcité. C'est un outil de simplification, service de la communauté éducative qui est soumise à l'interprétation de tenue. Susceptibles d'être à caractère prosélyte. Monsieur le Ministre, là dessus, nous avons un désaccord car nier les vertus de la tenue obligatoire ce serait priver les enseignants d'un outil qui les protège. Pour preuve, en novembre dernier, votre ministère faisait savoir que depuis la rentrée scolaire 2022. Les atteintes à la laïcité était en forte hausse. Sans parler de toutes celles qui ne sont pas signalés. Dernier point et non des moindres, la tenue d'établissements scolaires est une mesure sociale. Elle permettra de limiter le diktat des marques coûteuse pour les familles pouvant conduire l'élève à l'exclusion au raquette et au harcèlement. Concernant le financement, l'État abondera pour les familles ne disposant pas de ressources suffisantes par le biais de l'allocation scolaire. Cette mesure aussi pourrait profiter à nos entreprises françaises et mettent en avant le Made in France, par exemple, c'est une piste qui à mon sens il faudra explorer. Pour conclure, ma conviction est que la tenue d'établissement est un outil efficace. Bien sûr, cet outil ne suffira pas à résoudre tous les maux de l'école, elle n'en a pas la prétention bien sûr, elle n'est pas une potion magique elle contribuera néanmoins renforcer une culture commune fondée sur le respect indispensable au ciment de l'école. La majorité des acteurs de l'éducation et des élèves que j'ai interrogé m'ont conforté dans cette conviction est cher Annick Billon cherche Julien Bargeton la meilleure évaluation pour moi c'est la consultation à grande échelle. Concernant l'ensemble de la proposition de loi de notre collègue Max Brisson. Notre groupe, vous l'avez compris la votera car elle a l'ambition de proposer de vraies solutions à des difficultés indéniable. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent monsieur Franck Menonville du groupe les indépendants et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidence. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La gravité de la crise que traverse notre école est réel. Une défiance s'installe peu à peu le niveau d'ensemble baisse. Et le métier d'enseignant attire de moins en moins. Pourtant, l'école et ces enseignants sont en première ligne pour transmettre à notre jeunesse la grande les grandes valeurs de la République citoyenneté. Laïcité, culture de l'engagement sont au coeur des missions de l'école. Acteur majeur de l'égalité des chances. Ce contrat liant la République et ses enfants et futurs citoyens est aujourd'hui à renouveler. L'école a aujourd'hui besoin d'un nouveau souffle et de nouvelles perspectives. C'est tout l'objet de cette proposition de loi qui s'attelle à ce vaste chantier. L'égalité des chances. Tout d'abord en proposant la création d'un service public de soutien scolaire. On fait nous. Constatant que c'est un vrai sujet de fracture sociale au sein des familles. Elle a d'ailleurs été exacerbées pendant la crise sanitaire et le confinement en 2020. Concernant les savoirs fondamentaux, le texte propose de réarmer les enseignements du 1er les enseignants du 1er degré en améliorant leur formation. Il prévoit ainsi la création d'écoles supérieures du professorat qui prépare aux concours et forment les enseignants et et forment davantage et mieux les assassins. Les enseignants stagiaires, cela représenterait donc une vraie avancée pour mieux préparer les enseignants du 1er degré pour l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Cette proposition de loi vise aussi à accroître l'autonomie des des établissements par voie d'expérimentation. Il est en effet essentiel de donner aux établissements, la capacité d'initiatives, d'innovations qui s'impose. Cela participe aussi à la mode. Ah la motivation des enseignants et peut être il faudrait sans doute s'inspirer des systèmes éducatifs des pays nordiques qui repose sur l'autonomie des professeurs et celui également du Portugal qui tente à décentraliser les processus de recrutement et à octroyer davantage d'autonomie aux uns, aux établissements. De plus, il me semble qu'il faut aller plus loin et réformer le statut des directeurs d'école en renforçant le rôle et notamment dans les écoles les plus importantes. Le texte n'oublie pas non plus la ruralité et défend avec conviction une approche différenciée en matière scolaire, les territoires ruraux nécessite des critères spécifiques et adaptées à leurs défis. Ce texte prévoit également qu'une décision de fermeture de classe sera soumise à l'avis du conseil municipal ou untel ou untel ou des conseils intercommunaux. Il est as absolument essentiel d'associer davantage les élus locaux dans ce processus car les conséquences. D'une telle décision tant humaines que financières sont lourdes pour les territoires en matière de laïcité. Cette loi entend étant notamment aux accompagnateurs, le principe de neutralité politique et religieuse lors des sorties scolaires. La laïcité est l'un des grands principes qui doit être réaffirmée dans l'école de la République en 2021, l'IFOP publié un rapport en partenariat avec la fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty l'enquête souligner fait important, 34% des professeurs en réseau éducatif prioritaires ont témoigné de perturbations lors des cérémonies d'hommage. Par ailleurs et selon le rapport de Jean Pierre Audin. Oh ben la moitié des professeurs déclare s'être auto-censurer pour éviter des incidents. Avec certains élèves, ces chiffres doivent nous alerter et nous engager à agir au plus près des difficultés dont témoignent les enseignants et à les soutenir dans l'exercice de leur noble mission nous devons cesser les petits renoncements du quotidien qui font reculer la République et son idéal. Mes chers collègues ensemble le nouveau devant engager un grand chantier pour refonder les bases de notre école républicaine, elle doit être émancipatrice, elle doit préparer nos enfants aux défis de demain et les guider sur les chemins ardus de la connaissance, nous devons mener à une vraie réforme structurelle pour que les établissements disposent d'une plus grande autonomie les et puis les équipes de plus de liberté et de capacités d'initiative pour ainsi mieux s'adapter aux besoins des élèves. Cette proposition de loi a le mérite d'en provenant d'proposer quelques premières pierres et d'ouvrir la porte à d'autres améliorations. C'est un très bon signal que notre assemblée s'emparent de ce sujet et qui nous tient à coeur et qui est le moteur de l'espérance républicaine pour tous ceux-là je salue donc le travail de l'auteur de cette proposition de loi Max Brisson et de le travail bien évidemment également du rapporteur, Jacques Grosperrin et notre groupe votera en faveur de ce texte. Merci. Merci, cher collègue, la parole est enfin monsieur Olivier Paccaud du groupe. Les républicains pour 7 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur. Très chers collègues. L'école passionne. Elle fait parfois cliver. Elle peut susciter la caricature et-ce. Notre pauvre. Max Brisson caricaturer un vieux réactionnaire, c'était quand même pas très gentil chère Céline Brulin, je ne dirais pas que vous êtes une bolchévique rose quand même. Mais. Réjouissons-nous débattre. Réjouissons-nous de ne pas penser la même chose. Réjouissons-nous d'avoir des visions différentes. C'est ça la démocratie c'est le débat et nous allons, après le repas débattre effectivement de visions différentes et de propositions pour. Réinsuffler un. Nouvel élan à cette école qu'il y en a tant besoin. L'école c'est le sanctuaire républicain. Par excellence. La République en France. Il est pour ainsi dire n'est son idéal. Il y a été cultivée si affermie et propagé à l'ensemble du corps social. Chez nous, l'école et la République sont consubstantiels. Hélas ce coeur battant de la République. Cet organe essentiel. De notre démocratie, celui-là même qui est censé insuffler toute sa vitalité, sa cohésion à notre société est malade. pardon depuis trop longtemps de Meaux nombreux souvent niée. Faute de diagnostic effectué attends. L'affection qui ronge l'école est devenue générale et ce sont toutes ces fonctions qui en sont atteints. Le tableau symptomatologie qu'si je puis dire. De cette maladie de l'école n'est guère reluisant. Et pour cause. Là où elle obtenait des résultats pédagogiques excellent donnant une instruction vaste et ferme à des générations entières de jeunes l'école peine aujourd'hui à inculquer à ses élèves les fondamentaux, lire, écrire, compter. Sans compter tous ceux qui sortent du système. Sans bagages ni diplôme. La dégringolade de notre pays dans les différents classements internationaux n'en est que l'insigne Illustration, cela a été dit. L'école est par ailleurs devenu l'institution où apparaît la première lézardes sur la cuirasse de l'autorité. La volonté de s'affranchir des règles communes. Il devient les légions. La figure tutélaire de l'enseignant et méprisé. Or. Comment tendre des générations futures, qu'elle tienne notre État et c'est loin en respect, si elles ne sont déjà plus capable d'obéir aux enseignants censé les faire venir à la citoyenneté. Par ailleurs, l'école et ça a été débattu tout à l'heure. Est devenue un lieu de souffrance et de violences pour les élèves. La cloche qui sonne la fin de la récréation n'interrompt plus la tragédie du harcèlement scolaire devenu permanent sous sa forme cyber brimades. Moqueries et autres persécutions ne sont plus contenue par les grilles fermées de l'école. Elle chemine par les écrans colportée par les réseaux sociaux s'insinue jusque dans l'intimité du foyer ne laissant plus la moindre trêve à leurs malheureuses victimes. Le tableau dépeint jusqu'à présent est déjà bien sombre mais comment pourrait-il en aller autrement quand les chevilles ouvrières de l'institution scolaire sont si mal considéré. Je veux bien évidemment parler des professeurs. Comment exiger d'eux qu'ils accomplissent. Ce qui s'apparente à un véritable sacerdoce républicain dans des conditions si navrante. Quand leur rémunération les classe parmi les enseignants, les moins bien payés d'Europe. Quentin constante opprobre jeté sur une profession bien souvent ingrate et aux difficultés mal connu. Les sessions de recrutement hâtive parfois par la voie douteuse du job dating les concours qui compte 2 à 3 fois moins de lauréats que de postes à pourvoir sont d'autres symptômes inquiétants de la crise dans laquelle s'enlise notre modèle éducatif. Se trouvera-t-il encore suffisamment d'enseignants compétents et dévoués devant nos élèves, à la fin de la décennie. Enfin, que dire de l'abandon des territoires ruraux par les politiques éducatives. Si d'aucuns ont pu dire de façon caricaturale qu'il existait une école à 2 vitesses, en opposant un enseignement public en difficulté et un enseignement privé prisée. Pour avoir conservé les qualités évanoui du premier. Alors, force est de constater qu'il existe également un enseignement prioritaire à 2 vitesses celui soignant les quartiers de la politique de la ville au détriment des non moins déshérités zones rurales. En politique d'éducation, comment tout c'est encore une fois les métropoles où les agglomérations et le désert français. Une répartition plus équitable des ressources de l'enseignant prioritaire ne serait que justice et permettrait surtout à l'école de retrouver certaines des pièces mécaniques manquante pour relancer le fameux ascenseur social disparu. N'oublions jamais ce chiffre édifiant. Et accusateur pour notre école. 70 pour des élèves relevant de l'éducation prioritaire n'en bénéficient pas. 70%. Depuis 6 ans, on nous annonce une réforme de la carte de l'éducation prioritaire qui ne vient pas. Or la république. C'est l'égalité des chances partout et pour tous, ce qui n'est plus le cas. Face à cette situation alarmante, la présente, proposition de loi entend prescrire un début de remède. Administré les premiers soins sans toutefois se contenter d'expédients. S'y-t-elle avec courage et ambition. On ne pourra que se réjouir des mesures qu'elle propose que ce soir la création d'un service public de soutien scolaire. Un partenariat réel avec les collectivités pour l'établissement de la carte scolaire. Une attention particulière portée aux territoires ruraux défavorisés, la possibilité pour les professeurs d'élargir leurs horizons via la bivalence encourager. Le respect d'une laïcité vigilante et cohérente. La volonté de sérénité. Le climat scolaire par le port d'une tenue vestimentaire commune. Une opportunité. Mes chers amis, nous est offerte d'enrayer la maladie de l'école de rétablir cette dernière dans la noblesse de ses missions et la vigueur de ses succès. Tâchons de nous en saisir. Car c'est dans l'école d'aujourd'hui et de demain que se forme la société du futur et que l'égalité des droits et surtout des chances peut prendre forme.